La séance est ouverte. Le compte-rendu intégral de la séance du mercredi 6 juillet a été publié sur notre site internet, nous n'avons pas reçu d'observation, il y en a-t-il en séance. Je n'en vois point le procès verbal et donc adopté. Madame la Ministre. Mes chers collègues. Mesdames et messieurs. Et. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris, c'était le 7 décembre dernier la disparition de notre collègue Catherine Fournier, sénatrice du Pas-de-Calais. Elle nous a quittés à l'âge de 66 ans, à l'issue d'une longue et cruelle maladie contre laquelle elle s'est battue avec un courage incroyable jusqu'au bout, elle a continué à s'intéresser aux travaux de notre assemblée, je me souviens personnellement avoir encore échanger avec elle à ce sujet dans ces tout derniers jours. J'étais présent à Fréthun à ses obsèques, ce fut une émouvante cérémonie d'adieux à laquelle assistaient de nombreux élus et habitants. ça servile et du Pas-de-Calais. Le don de soi et l'amour du prochain ont sans cesse guider la vie de Catherine Fournier. Né à Boulogne sur Mer, elle a grandi près de Calais a fretin communes dont son père que je salue ici René Hauchard fut longtemps maire. C'est sans doute dans cet environnement familial au cours des premières années de sa vie que se forgea sa vocation pour le service de l'intérêt général, sa passion pour l'engagement public et politique. Après un diplôme universitaire de gestion des entreprises et des administrations obtenu à Lille, Catherine Fournier il fit ses débuts professionnels dans le secteur des assurances mais dès 1988 à l'âge de 33 ans, elle était de retour à fretin où elle Fonda une entreprise gérant une résidence hôtelière sous formes pavillonnaires, elle fut longtemps chef d'entreprise et illustré, dans ses fonctions, déjà l'engagement en contribuant par exemple à travers l'édification de motel à loger des ouvriers et leurs familles, c'était la construction alors du tunnel sous la Manche. Mais ce don de soi Catherine Fournier on apporta surtout le témoignage le plus éloquent dans l'exercice de ses différents mandats et singulièrement son mandat de maire. 1995 7 ans après son retour à fretin élu la fierté de succéder à son père à la mairie, brillamment réélu à 3 reprises par la suite, avec toujours de très beaux scores 1er tour 2008 90 %. Et allait rester maire pendant 22 ans, elle y renoncera en 2017 après son élection au Sénat pour se mettre en conformité avec la législation sur le cumul des mandats pendant plus de 2 décennies elle mis toute son énergie et sa générosité au service des habitants de Fréthun elle oeuvra bout avec beaucoup d'efficacité pour l'emploi et l'aménagement du territoire, elle s'investit à fond dans le dossier de la gare internationale de Calais Fréthun, point l'entrée du tunnel sous la Manche, grâce à son action, la ville s'est métamorphosé en se développant autour de cette gare TGV international et des installations d'Eurotunnel profondément ont raffiné dans sa commune, Catherine Fournier l'été aussi à son département et à sa région, élue conseillère générale du Pas-de-Calais, de 2006 à 2008, puis conseiller régional à partir de 2015, aux côtés de Xavier Bertrand et contribuer au dynamisme économique de la région, elle exerce doute d'importantes responsabilités dans les intercommunalités, vice-présidente de la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis, puis vice-président de l'agglomération de Grand Calais Catherine Fournier ne fut pas seulement une élue locale exemplaire, elle fut aussi une grande sénatrice son entrée au Sénat en septembre 2017 marquera sa vie politique après avoir sillonné le Pas-de-Calais au cours de la campagne pour les élections sénatoriales alors de mairie en mairie, aux côtés de Jean-François Rapin et du regretté Philippe Rappeneau, elle a défendu avec passion au sein de notre assemblée sa commune le Calaisis, son département, le Pas-de-Calais, dès son arrivée, nous avons apprécié cette femme, souvenez-vous, souriante, chaleureuse, nous les premières interventions dans l'hémicycle, furent écoutés avec beaucoup d'attention et la. Au groupe de l'Union centriste et devint membre de la commission des affaires sociales. Particulièrement assidus aux réunions de commission, elle se plongea très rapidement dans les travaux législatifs et fut nommé dès juin 2018 corapporteur de l'importer un projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur le volet relatif à la formation professionnelle en octobre de la même année, elle devint présidente de la Commission spéciale sur le projet de loi relatif à la croissance, il a la transformation des entreprises, elle exerça cette lourde responsabilité avec pragmatisme et engagement, menant à bien dans des délais brefs, l'examen d'un texte fleuve et disons-le quelque peu hétéroclite qui a donné lieu à près de 360 auditions et déboucher sur la loi dit Pacte riche. De plus de 200 articles par sa maîtrise des sujets qui étaient souvent des sujets techniques par son sens du dialogue, elle sut immédiatement suscité l'estime et le respect de ses collègues et j'ai le souvenir de de ces interventions en conférence des présidents. En 2020, elle participa à la commission spéciale sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique. Elle s'appliqua également dans les travaux de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Avec 2 de ses collègues membres de la commission des affaires sociales, Michel Forissier, Frédérique Puissat, elle fut l'auteur d'un rapport d'information rapport remarqué par sa grande qualité sur le droit social applicable aux travailleurs des plateformes Elia a formulé d'intéressantes propositions pour améliorer la protection sociale de ces travailleurs se trouvent souvent dans des situations particulièrement précaire, elle s'est aussi mobilisé sur le sujet de la pénurie de médicaments, l'un des effets de la crise sanitaire, plaidant, alors pour une mutualisation européenne notamment de l'industrie pharmaceutique. C'est en outre beaucoup investi au sein de la délégation aux entreprises. à la suite du renouvellement de 2020 Catherine Fournier, rejoignez la commission des affaires économiques et la commission des Affaires européennes, dont les présidents Sophie Primas et Jean-François Rapin peuvent témoigner de la finesse de ses analyses et de sa bonne connaissance des dossiers économiques et sociaux lors des questions d'actualité au gouvernement le marquer une pub n'a cité, notamment sur les dossiers de d'apprentissage, mais aussi de l'impact de la pêche industrielle sur l'écosystème, ou encore sur le sujet du Brexit. Catherine Fournier a toujours eu à coeur de défendre son territoire, elle s'est battue avec acharnement pour que soit les arrêts de l'Eurostar à Fréthun, tout comme elle s'est battue pour les droits des pêcheurs français lors des négociations du Brexit. Sa dernière intervention l'autre mystique, c'était il y a un peu plus d'un an. Fut pour défendre la mise en place d'un statut adapté à la spécificité de la liaison fixe transmanche, à l'instar de celui des porcs et des aérodromes. Au fond, elle ne cède rien. Je repense à cette phrase du général De Gaulle, soyons fermes pur et fidèle au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des femmes et des hommes qui n'ont pas cédé. Catherine Fournier n'a jamais cédé et jusqu'au bout, jusqu'au bout de sa vie. Toute sa vie, elle aura conservé cette ténacité cette droiture. Bien sûr, passionné par la vie publique et politique, mais aussi par les voyages, la musique, c'était de la vie de tous ceux qui l'ont connu une femme compétente, courageuse, persévérant, mais aussi profondément bienveillante généreuse et charismatiques, oui vous oui vous voulez dire à cet instant, dans cet hémicycle. La voix encore ici, là, en face, en face de moi. Ah. Une sénatrice chaleureuse, une élue de proximité au fond une véritable humaniste qui avait une profonde empathie pour les autres. à ses anciens collègues, des commissions des affaires sociales, les affaires économiques des affaires européennes à ses amis du groupe de l'Union centriste, Monsieur le Président et et vous Valérie Létard qui m'avait accompagné au dernier jour de cette rencontre que nous avions dans l'église de de Fréthun, j'exprime une fois encore notre sympathie attristée à son père René, ancien maire de Fréthun à son époux, Jean Claude à ses enfants, Antoine et Anna, sa soeur Michèle à ses proches, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa vie et on partageait ses engagements je souhaiterais la part que le Sénat a pris et continue à prendre à leur deuil votre peine est aussi la note, c'est vrai, nous avions loué avec elle ses Liens d'estime et d'amitié qui c'est dès la première rencontre, elle restera présente dans nos mémoires. Je vais donner la parole. Ah Madame Agnès Pannier Runacher ministre de la transition énergétique qui va s'exprimer au nom du gouvernement, Madame la Ministre. Merci, merci, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs. Il me revient, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, le funeste honneur de rendre hommage à votre très regrettée collègue Catherine Fournier et je le fais, sous son regard bleuté où l'on transparaît, sa force de caractère, j'y reviendrai Catherine Fournier. Un nom qu'il porte en lui le vent du littoral et le bruit des emprunts de cette mer du Nord, Calais-mettant. Car elle était du Pas-de-Calais autant de naissance que de coeur et fier de cet héritage de naissance, d'abord, elle est née en 1955 à Boulogne sur Mer citadelle ouverte sur le monde, port de pêche et d'échanges de ce Detroit du Pas-de-Calais, puis elle a grandi non loin de là, dans sa commune rurale de Fréthun, une commune qu'elle ne quittera jamais, ou du moins pas longtemps, notamment pour ses études, qu'elle a effectué à Lille afin d'obtenir un DUT de finances comptabilité son diplôme en poche, elle est vite revenu à Freitas au coeur de ce territoire du Calaisis qu'mettant et elle a décidé d'y lancer son entreprise de tourisme qu'elle a géré jusqu'en 2004 années à laquelle elle a rejoint une société d'export en tant que chef d'entreprise, elle a beaucoup contribué au développement économique de ce territoire, notamment en travaillant en lien avec le Royaume-Uni. Mais la vie de Catherine Fournier, vous le savez tous sur ces bancs, c'était aussi. Peut-être même surtout la politique. La politique au service de son territoire au service des habitants de sa commune de son département. De sa région. Car elle était également du Pas-de-Calais, de coeur et d'engagement à 40 ans en 1995 comme une évidence, elle a repris le flambeau de son père René Hauchard le flambeau de la mairie et de ses 1300 habitants. Réélu à 3 reprises pendant 22 ans, Catherine Fournier a été une mère exemplaire, elle a fait naître une nouvelle école, un stade de football, un complexe sportif et de nouveaux logements, elle s'est engagée sur le dossier difficile de la gare internationale de Calais Fréthun, l'un des combats les plus marquants de sa vie, dorénavant, Bruxelles n'est plus qu'à une heure Paris une heure 30 et pour les véhicules Londres trente-cinq minutes ce succès, il doit beaucoup à sa ténacité, il y a son engagement constant sur le projet d'Eurotunnel. Cet engagement pour son territoire, elle a poursuivi au sein du conseil régional des Hauts-de-France en tant que membre de la commission au travail qui portait bien son nom, elle n'a eu de cesse de défendre ses convictions, notamment en faveur de la réindustrialisation et de l'emploi ces derniers combats politiques, elle les a amener ici au Palais du Luxembourg, où elle a été élue lors du renouvellement de 2017 en tant que sénatrice et membre du groupe de l'Union centriste au sein de la commission des affaires sociales des affaires européennes, des affaires économiques et enfin de la délégation aux entreprises jusqu'au bout. Elle fait saisie des sujets qui lui tenaient à coeur, celui de notre modèle économique et de nos entreprises avec la Commission spéciale sur la loi pacte. Ou sa rigueur, sa droiture, mais aussi sa bienveillance en ont fait une présidente apprécié et respecté de tous, c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai fait sa connaissance et que j'ai tout de suite apprécié sa manière de conduire les débats, ou encore celui des travailleurs des plateformes au travers d'un rapport exigeant et complet sur le droit social qui lui est applicable, mais aussi, toujours sur les sujets qui touchent à son territoire. La problématique du Brexit et du risque d'un Odile pour les pêcheurs de la Côte d'Opale par exemple. La fermeture de l'Usine Bridgestone de Béthune où, là encore, nous avons travaillé ensemble et où j'ai pu mesurer la sincérité de ces engagements et sa très grande humanité. Avec son concours, nous avions mis en place le tout 1er dispositif choc industriel qui a permis le reclassement de la grande majorité des salariés mais aussi le développement de plusieurs projets porteurs d'un nouvel élan industriel pour le territoire. Catherine Fournier incarner la belle politique, celle des convictions et des combats pour les autres. Toujours au contact de la réalité du terrain jamais dans la posture donnant une vocation universelle oh très locales, précise technique mais aussi audible et à l'écoute, accessible, elle portait en elle l'âme du Pas-de-Calais, l'âme de ces territoires, dans toutes ses composantes de la côte au bassin minier en passant par le Ternois et l'Audomarois, un territoire qui aura autant font j'ai forgé son caractère que ses convictions. Catherine Fournier était une femme que l'on n'oubliera pas, elle était attachante humaine mais aussi franche et sa forte personnalité nous aura collectivement marqués. Sur tous les bancs on a vanté sa capacité de coûte mais aussi sa fermeté et sa volonté de faire avancer les choses, en travaillant avec tous les élus de bonne volonté. C'est avec ce même courage cette même force qui a caractérisé sa carrière qu'elle a affronté la longue maladie, vous l'avez dit, monsieur le président, qui a fini par l'emporter Au nom du gouvernement. Et avec beaucoup de tristesse, en y associant plus particulièrement ceux de mes collègues, comme Olivia Grégoire, Gérald Darmanin, Bruno Lemaire qui la connaissait de longue date. Je tenais à adresser mes plus sincères condoléances et ma solidarité dans l'épreuve à son époux d'abord qu'il avait arrêté son activité pour l'accompagner jusqu'au bout. Il y a 6 enfants qu'elle aimait par-dessus tout à sa famille ensuite à tous ses proches et aux habitants du Pas-de-Calais 2 fretin pour qui elle s'est tant battu. Et enfin, à vous, ses collègues de l'Union centriste, mais aussi de tous les bords, avec qui allez-mettant en débattre et échanger. Souvenons-nous de son salaire de son sourire solaire. Souvenons-nous de ces valeurs. Souvenons-nous de ces combats, je vous remercie.

Et. Ainsi hommage à Catherine Fournier nous allons suspendre nos travaux pour quelques instants. Elle sera reprise de la séance à 15 heures 15 la séance est suspendue.

La séance est reprise. Chers collègues par courrier du 11 juillet je Guillaume Gontard, président du groupe, écologie, écologie, solidarité territoires demande que le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'État du Qatar le gouvernement de l'État du Qatar relatif au statut de leurs forces, inscrit à l'heure du jour, le mardi 19 juillet à quinze heures quinze soit examiné selon la procédure normale et non la procédure simplifiée. à tes données de cette demande et dans la dire discussion générale qui aura donc lieu, nous pourrons nous pourrions attribuer un temps de 45 minutes aux orateurs des groupes le délai limite pour les inscriptions de parole sera fixée à lundi prochain 18 à 15 heures. Il n'y a pas d'opposition à ce changement, il en est ainsi décidé. L'ordre du jour appelle. Une déclaration du gouvernement, suivie d'un débat en application de l'article 50 tirer hein de la Constitution sur le bilan de la présidence française de l'Union européenne, la parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à qui nous souhaitons la bienvenue. Monsieur

Monsieur le président, Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le président de la République et la première ministre m'ont fait un immense honneur en m'accordant leur confiance, alors que je m'exprime pour la première fois devant vous dans cet hémicycle, je peux vous assurer que je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne, tout comme la secrétaire d'État, qui est à mes côtés, Laurence Boone. Je vais aussi vous assurer que je souhaite associer pleinement le Parlement à l'action de mon ministère, on vous informant régulièrement de nos travaux en débattant avec vous comme nous le faisons aujourd'hui en vous rendant compte de nos résultats et de l'action de la diplomatie que je porte, sous l'autorité du président de la République et de la Première ministre, je n'aurais dans mon action qu'un seul impératif et qu'une seule boussole agir au service des Français. Car, alors que les ordres du monde et les crises à répétition ne cesse d'affecter, de plus en plus leur quotidien, je veux porter une politique étrangère qui contribue à apporter des réponses à leurs préoccupations et voilà l'esprit dans lequel j'entends travailler en tant que Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, je tenais à vous le dire d'emblée, et à vous le dire aussi clairement que je viens de le faire avant de dresser comme vous m'y invitez avec vous le bilan de 6 mois de présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je me réjouis beaucoup du débat sur ces 6 mois de présidence française parce que pour moi, parler d'Europe, c'est parler de notre souveraineté de nos valeurs de notre avenir, de notre capacité à garder en tant que Français et en tant qu'Européen, notre destin en main et donc pour le dire autrement, rester les auteurs de notre histoire collective que personne d'autre ne doit venir écrire à notre place. Nommé ministre au terme d'un parcours qui m'a, entre autres, emmenés de Romain oh je suis traité où fut signé le traité fondateur du 25 mars 1957 à Londres qui a fait le choix de quitter l'Union européenne, un choix que nous devons respecter mais que nous regrettons, je sais l'importance capitale pour l'avenir de nos nations et de nos peuples européens de ce projet politique majeur l'Europe dans ce contexte, je suis particulièrement fier de pouvoir affirmer que les résultats de ce semestre français à la tête de l'Europe sont des résultats historiques historique par leur portée mais historique, d'abord en raison des circonstances inédites dans lesquelles s'est déroulée cette présidence je pense bien sûr à la guerre déclenchée par la Russie, en Ukraine, au mépris du droit international, de ses propres engagements de la souveraineté de l'Ukraine et de la sécurité de notre continent. Ce choix funeste d'une agression, le 24 février signe le retour de la guerre, sur d'autres continents. Et là, bien sûr, profondément marqué notre présidence mais nous avons su y répondre collectivement en tant qu'Européens et c'était notre responsabilité de présidence française que de réussir cela, ils répondent collectivement, sans pour autant et je vais y revenir perdre le cap de ce que nous avions décidé de faire. Nous allons donc poursuivre l'agenda ambitieux que nous nous étions fixés en amont de ces événements ainsi au bout de 6 mois de présidence, je crois pouvoir dire que l'Europe de juillet 2022 n'est plus celle de décembre 2021. Elle est plus forte, plus souveraine et plus unie. C'est bien sûr le fruit des travaux de fond que nous avons menée, c'est également l'effet des urgences que nous avons eu à gérer. C'est le 1er volet de notre action sur lequel je veux insister, la réponse immédiate à la guerre en Ukraine que Vladimir Poutine a pris la responsabilité de déclencher le 24 février dernier aux portes de notre Union. L'Europe n'était sans doute pas préparé à affronter une mise en cause aussi brutale de l'ordre international et de ses propres intérêts stratégiques, pourtant, elle a su réagir avec force et unité à une crise qu'elle a tout fait pour désamorcer. C'est ainsi l'honneur de notre pays d'avoir pu mobiliser ses partenaires européens et internationaux pour y faire face, nous l'avons fait à titre national en prenant toutes nos responsabilités pour soutenir l'Ukraine dans cette guerre qu'elle doit gagner il y va de son avenir, mais aussi d'une c'est une nécessité pour que l'Europe retrouve la paix, une nécessité pour que les principes sur lesquels nous avons bâti notre sécurité collective depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale soit respectée. Mais nous l'avons fait également dans notre rôle de présidence à l'initiative de la France, l'Europe s'est en effet élevé à la hauteur des enjeux en 3 mois, tout d'abord, elle a pris à l'encontre de la Russie, une série de sanctions sans précédent. Au service d'un objectif clair : faire comprendre à la Russie qu'elle a choisi une impasse et asphyxié le financement de son effort de guerre. Alors, on a souvent coutume de reprocher à l'Union européenne, sa lenteur ou son manque de réactivité, or en moins de 48 heures, le premier paquet de sanctions était adopté à l'unanimité des 27 et notre main n'a jamais tremblé par la suite, ce qui a permis d'adopter tous les autres paquets de sanctions qu'elle souhaite individuelles financière ou commercial, nous en sommes aujourd'hui, vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs à six paquets et nous maintiendrons la pression autant que nécessaire et nous la renforcerons si cela est nécessaire. Les Européens ont aussi brisé ce qui était jusqu'ici un tabou majeur en Europe parce qu'il fallait en décidant de financer désarmement y compris armements létaux ces armements dont l'Ukraine a besoin pour se défendre. Et là aussi, il n'a pas fallu attendre longtemps car, dès le dimanche 27 février cette décision a été prise ce jour-là, les Européens ont activé. Le mécanisme la Facilité européenne de paix le mécanisme qui permet de dégager des ressources à cette fin et le message de l'Europe, ce jour-là était également très clair Le Temps de l'innocence stratégique est révolue, l'Europe est prête à faire face et elle sait faire face. Les pays européens ont également été au rendez-vous de la solidarité, de la fraternité en accueillant les millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens chassés par le conflit, à qui a été accordé l'autorisation de venir se protéger dans un pays de l'Union en bénéficiant de droits très concret, le droit au logement, au travail à la scolarisation des enfants aux prestations de santé. Nous avons pour cela utilisé pour la première fois une directive qui datait de 2001 permettant d'accorder ce qu'on appelle la protection temporaire Nous avons également mis en place un très vaste pont logistique pour apporter à l'Ukraine, l'aide humanitaire dont elle a besoin et nous avons, vous le savez, également appuyé la Moldavie voisine qui est directement touché par les conséquences du conflit. Nous avons enfin doter l'Union européenne des moyens de collecter des preuves des exactions et des crimes commis par l'armée russe en Ukraine, en renforçant le mandat d'euros juste parce qu'il ne saurait y avoir d'impunité pour les crimes de guerre. Ce travail indispensable est venu en complément de l'engagement des États qui, comme le nôtre ont soutenu et soutiennent encore le travail des autorités judiciaires ukrainienne et de la Cour pénale internationale. La réalité c'est que ces circonstances inédite et tragique ont confirmé à la fois la pertinence et l'urgence de l'agenda de souveraineté dont le président de la République avait donné l'impulsion dès 2017 dans l'amphithéâtre de la Sorbonne et qui a constitué le le fil d'Ariane de toute notre présidence, c'est le 2ème volet de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne qui s'est attaché à tirer toutes les conséquences de la guerre en Ukraine pour continuer et poursuivre le renforcement de notre souveraineté et contribue ainsi à consolider l'indépendance, la sécurité et la stabilité de l'Europe. Quelques mots à ce sujet au sommet de Versailles en mars dernier, l'Europe a affirmé sa volonté de rester maître de son destin, c'est-à-dire pleinement libre de ses choix. Libre de ses choix énergétiques, c'est l'ambition qui sous-tend la décision prise par les chefs d'État ou de gouvernement européen de sortir rapidement de notre dépendance au pétrole et il faudra également au gaz russe, la France, pour sa part, je n'ai pas besoin de souligner a toujours considéré son indépendance énergétique comme essentiel à sa souveraineté et ne peut que se féliciter des choix qu'elle avait fait dans le passé, libre de ses choix économiques aussi, la politique industrielle européenne ne se réduit plus aujourd'hui au droit de la concurrence avec des programmes paneuropéen dans le domaine de la santé de l'hydrogène ou encore des semi-conducteurs, nous bâtissons notre indépendance dans des domaines qui sont des domaines cruciaux pour notre avenir. Du fait des crises du fait de ces crises qui parfois nous réveille et qui souligne les vulnérabilités qui étaient les nôtres et nous engage à à réagir une prise de conscience se fait chaque jour un peu plus en Europe, l'Europe ne peut pas être un grand marché, un grand marché de consommateurs qui achèteraient des produits fabriqués ailleurs, si l'on veut être indépendant, il faut aussi être capable de produire soi-même, en particulier dans les secteurs critiques, mais pas seulement, je pense que chacun se souvient au début de la pandémie de la Covid 19 des difficultés qui étaient les nôtres à nous procurer ne serait-ce que masque ou gels hydro-alcoolique. Au sommet de Versailles est donc toujours au mois de mars dernier, l'Europe s'est mis à parler le langage de la puissance, c'est la condition de notre sécurité collective, comment en décidant de remédier au sous-investissement dans les capacités collectives, individuelles, de défense des Européens en se dotant d'une boussole stratégique qui est un véritable livre blanc de la sécurité de la défense européenne et qui vaut pour les 10 ans qui viennent, elle a pu être adopté par le Conseil européen des 24 et 25 mars dernier elle fixe des objectifs très concrets pour que l'Union puisse conduire plus facilement des opérations plus Agile qu'elle renforce sa résilience qu'elles investissent davantage encore dans sa défense et améliore encore sa coopération avec l'OTAN. Par ailleurs au Conseil européen des 23 et 24 juin l'Union s'est affirmer comme une puissance de stabilité sur le continent, il faut mesurer, je crois que l'histoire permettra de le voir clairement le caractère véritablement historique qui a été la décision prise par le Conseil européen, à l'unanimité d'octroyer à l'Ukraine et à la Moldavie, le statut de candidat à l'Union européenne. Cette décision du Conseil européen avait été préparée, notamment par le déplacement à Kiev le 16 juin du président de la République avec le chancelier allemand Scholz, le président du Conseil italien Draghi et le président roumain Ioannis déplacements effectués à la veille de la vie que devait rendre la commission sur les demandes de ces pays et déplacements qui a certainement contribué à forger le consensus au Conseil européen. Le choix fait par notre union a été d'envoyer à l'Ukraine, un message de solidarité vital pour elle comme un à la Moldavie, dont on sait qu'elles étaient fragiles et exposés, mais c'est aussi, je voudrais le souligner devant vous notre intérêt stratégique, car il n'y a plus de demi-mesure possible dès lors que la Russie avait choisi de se couper des principes du droit international et de s'isoler. Pour autant, une fois ce statut de candidat reconnu, nous le savons tous la perspective d'adhésion ne répond pas à elle seule au défi d'accueillir l'Ukraine et la Moldavie dans la famille européenne, ni ces pays ni les nôtres ne peuvent attendre pour renforcer une cohésion qui est plus nécessaire que jamais. C'est l'une des raisons pour lesquelles le président de la République a proposé de créer une communauté politique européenne au sein de ce forum, qui se substituera pas aux organisations existantes, l'OTAN, le Conseil de l'Europe, l'OSCE ou d'autres, nous pourrons bâtir des coopérations concrètes avec les pays candidats sur de nombreux domaines, mais nous pourrons aussi approfondir la discussion sur des sujets de sécurité entre non seulement les pays candidats, mais tous les pays européens par la géographie et par les valeurs. L'organisation par la présidence tchèque en octobre prochain d'une première réunion des chefs d'État ou de gouvernement donnera ainsi le coup d'envoi de cette nouvelle communauté. Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs cet agenda de souveraineté et c'est le 3ème volet de notre présidence, nous l'avons mis en oeuvre aussi bien sûr dans le cadre du programme législatif ambitieux que nous nous étions fixé à l'origine, et que nous avons mené à bien dans tous les domaines, je dois le dire. La tentation aurait pu être le 24 février 2 considérer qu'il n'y avait plus pour les Européens, qu'un seul sujet : l'Ukraine, la guerre en Ukraine, ses conséquences, la façon d'y répondre et nous avons au contraire estimé que cette guerre au coeur de l'Europe ne faisait que valider notre priorité la priorité qui préexistait et qui était au coeur de notre présidence, faire que l'Europe soit plus souveraine plus unie, plus proche de ses citoyens. Et ainsi, malgré la guerre nous avons accélérer nos efforts, nous l'avons fait d'abord dans le domaine de la transition écologique qui est pour nous tous, hein, un objectif stratégique l'accord obtenu au Conseil Environnement du 20 8 juin donc tout récemment, presque à la fin de notre présidence entre les États membres sur le paquet climat- fait font Fifty Five comme on dit souvent : Bruxelles. Et une avancée majeure qui doit assurer que nous réduirons de 55 % voilà notre ambition de 55 % nos émissions de CO2 dans l'Union européenne en 2030, par rapport à Cela confirme que l'Europe entend continuer à être sur la scène internationale, à l'avant-garde du combat nécessaire pour répondre à l'urgence climatique et cette transition écologique car tout est lié, elle est également indispensable pour que l'Europe gagne en souveraineté énergétique en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles. Cet agenda écologique se traduira par des bénéfices concrets pour nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Avec, par exemple, mais on pourrait citer d'autres exemples, celui-ci a été déjà fort médiatisée, la mise en place de chargeur unique à compter de 2024 pour tous les smartphones, ordinateurs portables et autres objets connectés, ce n'est pas un anecdotique parce que en effet réutilisé Un même chargeur pour tous les appareils que nous avons, nous remplaçons facilitera notre vie quotidienne, je n'en doute pas, mais ça permettra aussi d'éviter des milliers de tonnes de déchets électroniques chaque année 11000 tonnes selon les ONG qui ont évalué ce que ceux de la représenter par an. Enfin, un accord a été trouvé entre les États membres en vue d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour que nos efforts écologiques ne viennent pas donner un Avantage concurrentiel à ceux qui n'en font pas, c'est désormais au Parlement européen de se prononcer, je précise que l'enjeu est aussi environnemental car ce mécanisme est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les fuites de carbone, en effet, dès lors que ce mécanisme empêchera les risques de concurrence déloyale, une entreprise européenne n'aura plus de raison de se délocaliser à l'extérieur de l'Union pour espérer bénéficier de nos économies de nos employes et du climat, c'est donc un pas extrêmement important qui a été franchi l'Europe souveraine et c'est aussi affirmé dans le domaine social, l'Europe sociale, on en parlait beaucoup, il m'est arrivé de le faire dans d'autres circonstances, et d'autres temps, désormais elle prend corps et elle prend corps en pleine cohérence avec le modèle que la France a toujours défendu. Chaque travailleur européen disposera grâce la directive qui crée un cadre commun sur le salaire minimum d'un revenu minimal adéquat, je voulais souligner devant vous que c'est une avancée majeure, une véritable conquête sociale à l'échelon européen, ce socle européen des droits sociaux que nous appelons de nos voeux, qui était une promesse, hé bien il commence aujourd'hui à prendre forme et il prend forme. Je suis également fier que notre pays, il fait adopter après 10 ans de blocage une directive fixant un objectif clair aux entreprises, au moins 40 % de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises en Europe d'ici 2000 26 à échéance rapprochée, c'est une avancée considérable, pour nous tous et pas seulement pour nous toute une avancée considérable pour l'égalité entre les femmes et les hommes égalité dont le président de la République a fait pour son second mandat, comme il l'avait fait pour le premier, une priorité je voudrais aussi rappeler la proposition du président, annoncé le 19 janvier visant à inscrire le droit à l'avortement dans la charte européenne des droits fondamentaux. Le Parlement européen, vous le savez la reprise à son compte aujourd'hui et à l'heure, évidemment, où ce droit fondamental est remis en cause dans une démocratie aussi importantes que les États-Unis, l'Europe doit d'autant plus porter ce combat pour elles-mêmes et, au-delà de ses frontières. Nous avons également fait de pas de géant que je vais citer pour mieux réguler le numérique, je parle de l'adoption de ces 2 textes clés que sont l'acte sur les services numériques et l'acte sur les marchés numériques. Texte qui auront un impact majeur sur nos vies et celles des générations qui nous suivent, il s'agit bien sûr d'empêcher les comportements monopolistiques des grandes plateformes et les abus de position dominante qui existait, c'est pas tant, mais il s'agit aussi de les contraindre à la responsabilité et à la transparence sur la suppression des contenus illicites sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas permis hors ligne n'est pas permis en ligne. Car c'est peut être là, qui était l'une des principales menaces pour nos démocraties des réseaux sociaux sans loi, livrée à la loi de la jungle et avec ce phénomène, la remise en cause de la validité de la parole publique et la validité d'un débat éclairé entre les représentants des citoyens. Notre objectif désormais est que cet ex-européens deviennent des références mondiales en effet, c'est ma conviction que l'Europe en se donnant des règles pour même même de fait en train de contribuer à l'élaboration d'un véritable ordre public international du numérique. Le garage. Pourquoi est-ce que je vous dis cela parce que nous l'avons vu déjà depuis plusieurs années avec le fameux RGPD qui est repris, qui protège nos nos droits et qui repris aujourd'hui par de nombreux pays tiers et je ne doute pas qu'il en ira de même avec ses 2 autres textes majeurs que nous venons d'adopter, sous présidence française et qui répondent à des besoins fondamentaux. L'Europe souveraine, nous l'avons aussi fait en sortant définitivement l'Europe commercial de ce qu'on a pu appeler sa naïveté. Parce qu'elle considérait souvent le commerce du du seul point de vue économique, l'Europe a été longtemps, trop longtemps prête à accepter des règles du jeu asymétrique, le choix de l'ouverture, qui était le sien depuis toujours, devenez pour nombre de nos citoyens et de plus en plus synonyme de naïveté, ça n'est plus le cas, je voudrais citer 3 exemples

c'est un progrès majeur sur lequel nous avons travaillé depuis 15 ans, là aussi, vous me pardonnerez de faire référence à mon passé mais dans d'autres fonctions traitant également des Affaires européennes, je me souviens qu'il y a 15 ans, c'était déjà le combat du gouvernement de la France. De la même manière, autre exemple, les États subventionnant à outrance leurs entreprises et on peut penser là encore à la Chine, mais pas uniquement, venant ainsi faussé la concurrence au sein de notre marché intérieur seront sanctionnés par la Commission européenne, grâce à l'accord qui a été trouvé au Conseil au tout dernier jour de notre présidence sur l'instrument de lutte contre les subventions étrangères et 3ème exemple : nous avons promu également un renforcement des règles protectrices pour la santé des consommateurs via ce qu'on appelle des mesures miroir qui permettent d'imposer aux produits importés, les mêmes règles que celles que nous appliquons pour nos productions au sein de l'Union. et 3 exemples que j'ai choisi parce que il part, je pense, très concrètement à nos concitoyens à nos entrepreneurs et aux salariés de notre pays, la vérité et vous m'avez entendu sa référence au passé, par 2 fois, c'est que cela faisait longtemps que la France porter ces questions au plan européen, sans être toujours entendu, sinon nous serions rêver plus vite et certains des partenaires, vous vous en souvenez, je m'en souviens, en tout cas, voyez même une certaine forme de protectionnisme dans notre plaidoyer. Aujourd'hui les temps ont changé. Nous avons saisi l'occasion de notre présidence pour faire que il y a des résultats sur chacun de ces domaines, et les résultats sont là, l'Europe est désormais beaucoup mieux armées pour protéger et protéger réellement efficacement nos intérêts et nos emplois. Affirmer notre souveraineté, nous l'avons encore fait en renforçant l'espace Schengen et en débloquant les discussions sur le pacte Asile migration qui sont des sujets majeurs également l'espace Schengen, nous l'avons renforcée en réaffirmant son pilotage politique par la création d'un conseil des ministres Schengen qui se réunira régulièrement puis en revoyant les règles qui régissent la gestion des frontières internes et externes de l'Union, on sait qu'il n'y a pas de réponse nationale. Qu'qui soit suffisante pour faire face au défi migratoire et la réponse, elle est forcément aussi européenne et internationale et européenne d'abord, dès lors que nous partageons un même espace de libre-circulation pour nos concitoyens. Au sein de l'Union européenne, la seule réponse efficace et donc celle de la responsabilité renforcée des pays de première entrée qui a été rappelé et tout, tu dois bien sûr aller de Pair avec la solidarité des autres États vis-à-vis des pays tiers et singulièrement vis-à-vis des pays d'origine, il faut aussi une approche équilibrée, continuer à porter notre effort en matière de développement car on sait bien que c'est l'un des fondements majeurs d'. Cette Cette l'absence de perspectives pour de très nombreuses personnes des pays les moins développés, qui les poussent à entreprendre le voyage migratoire cette politique pourtant n'exclut nullement la fermeté dont il faut savoir faire preuve, par exemple lorsque certains pays tiers refuse d'admettre sur leur territoire de réadmettre les ressortissants qui sont entrés illégalement sur le territoire européen, et qui donc n'ont pas vocation à l'asile, selon notre droit et c'est cette logique fondée sur le respect de ses équilibres nécessaires indispensables même qui nous a permis d'obtenir en juin d'importantes avancées, en particulier s'agissant d'un contrôle renforcé des migrants à leur arrivée sur le territoire européen. Enfin, sous notre présidence, nous avons accompagné des travaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe, nous avions invité les citoyens à écrire le prochain chapitre de notre union, dans le cadre d'un exercice participatif qui a été un exercice inédit, les membres du gouvernement sont allés à la rencontre des Françaises et des Français, dans toutes les régions de France, entre mai 2021 et mai 2022 donc toute une année pour recueillir leurs propositions, ces propositions ont été présentées à l'échelon européen, le 9 mai vous avez entendu le président de la République et elles doivent maintenant trouver une réponse concrète, c'est l'une des priorités de la présidence tchèque qui prend le relais de la nôtre, la France bien sûr prendra toute sa part à la traduction de ses priorités, enfin c'est le 4ème et dernier volet de notre présidence, c'est aussi avec nos partenaires à l'extérieur de l'Europe qu'il nous faut aujourd'hui bâtir les conditions de notre indépendance et notre prospérité. Je vais souligner une évidence, une part de notre avenir se joue dans notre capacité à renforcer nos partenariats avec les grandes régions du monde dans un monde qui est plus que jamais globalisé, où les interdépendances sont soulignés, chaque jour, je pense en 1er lieu L'Afrique que la présidence française avait mise au coeur de la PFUE avec le sommet Union européenne-Union africaine des 17 et 18 février, nous y avons lancé tous ensemble européen un projet de refondation du partenariat entre l'Europe et l'Afrique car il est nécessaire. Projet centré autour des questions économiques, mais aussi de la formation et de la jeunesse nous resterons bien sûr au-delà de notre présidence, très engagée pour participer à sa mise en oeuvre, vous avez entendu la première ministre je pense dans son discours de politique générale, je pense également à l'indo-Pacifique, la France est présente, puisque la France cette aussi un pays du Pacifique et et de l'océan Indien, région vitale pour nos exportations et nos approvisionnements mais région qui fait face à la pression de la présence croissante de la Chine, c'est donc une nécessité absolue pour nous de nous impliquer en tant que puissance et nations du Pacifique, grâce à la présence et à la force de nos territoires ultramarins mais aussi c'est une chose nécessaire pour les grands équilibres du monde, c'est pourquoi nous avons organisé sous présidence française du Conseil de l'Union européenne le 1er forum ministériel UE- indopacifique à Paris le 22 février et qui a permis d'avancer sur 3 sujets de façon concrète des projets de sécurité et de défense de connectivité et de numérique et les enjeux globaux ont également été ciblés comme la 3ème priorité je me félicite que l'Union européenne est adopté cette stratégie, c'est une région clé une partie de notre avenir, séjour, là aussi, la présidence tchèque prendra le relais également bien sûr partenariat transatlantique, car nous savons qu'aucun des grands défis qu'ils soient numériques, j'en parlais beaucoup écologique commerciaux internationaux ne pourra être réglé sans une coopération étroite entre l'Europe et les États-Unis États-Unis qui mesure je crois aujourd'hui, combien l'Union européenne peut également être utile aux équilibres du monde et cet égard et le sommet de l'OTAN s'est tenu il y a quelques semaines, je me félicite que, sous présidence française, le sommet est permis. De pousser auprès de nos amis et alliés, une meilleure appréciation de la contribution de ce que l'Union européenne apporte à la défense et la sécurité de tous les alliés, le concept stratégique adopté lors du sommet de Madrid reflète reflète cette complémentarité cet équilibre et vous vous prononcerez bientôt mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs sur la ratification de l'accord autorisant la Suède et la Finlande à l'Alliance Atlantique, un choix qui était le leur, une adhésion qui renforcera notre sécurité collective comme elle renforcera la place des Européens au sein de l'Alliance, dernière région que je veux évoquer les Balkans occidentaux. Région stratégique et région encore trop troublé région stratégique qu'on ne doit pas laisser dériver loin de la famille européenne, a fortiori dans un contexte où des puissances tierces n'hésiteront pas, et on le voit déjà à occuper les vide politique et stratégique que nous aurions laissé. Les pays de la région sont sur le chemin de l'adhésion d'un chemin qui est exigeant et difficile leur marges dépend avant tout de même, mais notre intérêt, c'est de les accompagner, c'est pourquoi nous avons organisé en marge du dernier Conseil européen de juin, donc le 23 juin une réunion avec les chefs d'État ou de gouvernement des Balkans occidentaux pour réaffirmer leur perspective européenne et rappeler que la marche à suivre, de notre côté éclair du leur, elle doit l'être aussi, vous connaissez les difficultés qu'ont quelques pays à régler leurs sujets bilatéraux. Ces succès mes à mes messieurs les sénatrices et sénateurs, je voudrais aussi dire à qui nous les devons d'abord bien sûr au président de la République qui a mis, depuis sa première élection 2017 qui a mis le rap au coeur de son projet politique et qui a porté l'agenda et la vision de notre présidence, mais je veux aussi saluer au au-delà du chef de l'État, l'action de tout le gouvernement. Autour de Jean Castex, puis autour de la Première ministre Élisabeth Borne ça lui aussi celle du secrétariat général des affaires européennes du secrétariat général de la présidence française, celle de tous les ministères et de tous leurs agents qui ont été mobilisés pendant des mois et des mois, hé bien avant le début de la présidence française pour concevoir ce que nous ferions puis animé la présidence réussir ces négociations, faire vivre le projet européen ça, lui aussi, tous les territoires qui ont vu les collectivités se mobiliser tous les citoyens qui ont participé au débat sur l'Europe et partout la société civile qui s'empare, et je m'en félicite, peu à peu du projet européen et, enfin, je veux saluer bien sûr avec Laurence Boone, l'action déterminante de mon prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, qui, à ma place, a conduit pendant 5 mois, les travaux de la présidence française et celle de Clément Beaune ils ont mené, ils ont mené la PFUE à bon port et enfin comme Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ayant succédé à Jean-Yves Le Drian je veux dire, bien sûr, et je souhaite leur dire solennellement devant vous ma fierté du travail qui a été accompli par tous nos diplomates et agents du Quai d'Orsay à Paris à la représentation permanente auprès de l'Union européenne à Bruxelles et dans toutes nos ambassades en Europe et partout dans le monde, voilà ce que je voulais vous dire mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs sur cette 13ème présidence depuis le début de la construction européenne, alors, le 30 juin j'ai symboliquement passer le témoin, le relais le bâton comme l'on dit, mais je mets des guillemets, s'il vous plaît, n'ayez pas mauvais esprit à la présidence tchèque à mon collègue Jan Lipavsky. Nous pouvons être fiers, je crois, de laisser à la présidence tchèque, une Europe qui n'hésitent plus à affirmer sa souveraineté qui ose défendre ses intérêts stratégiques, économiques, ce qu'il faut de clarté de fermeté pour se faire respecter, mieux qu'auparavant, la fin de la présidence française, puisqu'elle est derrière nous depuis le 30 juin ne signifie pas que nous abandonnons non on les priorités qui sont les nôtres, bien au contraire, vous pouvez compter sur ma détermination sur celle de Laurence Boone si ça tout le gouvernement pour faire en sorte que les résultats de la présidence française et sème bien au-delà de ces six mois, nous travaillons très étroitement avec nos partenaires d'abord partenaire tchèque puis suédois au sein de ce qu'on appelle le trio de présidences puisque nous formons un trio et nous travaillons aussi avec tous nos autres partenaires au 1er chef, l'Allemagne, puisque nous sommes 27 ensemble dans la même aventure, en n'oubliant jamais que notre devoir est de bâtir au service de nos concitoyens une Europe encore plus forte encore plus soudé encore plus durable, en un mot plus souveraine, je vous remercie. J'ai le plaisir de saluer dans la tribune d'honneur, une délégation de sénateurs du groupe d'amitié France-Espagne, la délégation est conduite par son président Monsieur Pio Garcia Escudero ma caisse qui présida le Sénat espagnol de 2011 à 2019 est accompagnée par son excellence Monsieur victorieux Redondo quand, ambassadeur de France, de l'Espagne en France pardon et par nos collègues Michel Meunier et François Bonhomme, président et vice-président du groupe d'amitié lors de sa visite en Loire-Atlantique, la délégation est notamment visité chantiers navals de Saint-Nazaire, elle sera reçue demain en audience à la présidence, avant une série d'entretiens institutionnel, la coopération bilatérale entre l'Espagne et la France, nous le savons et solide, que ce soit en sécurité en politique énergétique ou encore dans les domaines scientifiques et universitaires, la présence de nos homologues espagnols à l'occasion de ce débat sur le bilan de la présidence française du Conseil de l'Union est un signe fort des Liens d'amitié qui relie nos deux pays elle revêt une portée symbolique que je me permets de souligner, mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à la délégation espagnole la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour. La parole est

La parole est maintenant au président Jean-François Rapin. Monsieur

Madame Bruno nous a quitté, mes chers collègues, le gouvernement a dressé son propre bilan de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en forme de panégyrique, cela n'étonnera personne, si l'on s'en tenait au dossier de presse qui l'a publiée, nous pourrions rester là et notre séance n'aurait pas lieu d'être, mais permettez-moi de gratter le vernis, car tout ce qui brille n'est pas de l'or, il est de notre responsabilité de ne pas passer sous silence les zones d'ombre et les angles morts de cette présidence française, elle s'est donc déroulée au 1er semestre 2022 malgré et nous l'avions déploré la concomitance d'échéances électorales importantes pour notre pays, c'était un choix du président de la République qui aurait pu demander un report de fait, même si nos diplomates ont pu arracher des accords in-extremis au conseil, ce fut au plan politique, une présidence tronqué. La France a manqué de temps pour convaincre ses partenaires sur certains dossiers, je pense, notamment, notamment au texte sur le financement des partis politiques européens et la transparence de la publicité politique que le président de la République affichée comme une priorité pour renforcer la démocratie en Europe. Je ne nie pas que dans l'ensemble, les grands dossiers européens est avancé sous présidence française, mais ces avancées tiennent autant, voire plus, à la Commission européenne, c'est la commission qui a donné le tempo, elle a suivi son programme de travail et publier les textes annoncés aux dates prévues côté conseil la présidence française avait de toute façon rétréci par rapport à 2008 en 2022 le Conseil européen n'était plus présidée par la France, puisqu'il existe dorénavant dorénavant un président permanent du Conseil européen Charles Michel, idem pour le Conseil des Affaires étrangères, présidée depuis le traité de Lisbonne par le haut représentant de l'Union aujourd'hui Josep Borrell dans ce costume étroit, la France a consenti de réels efforts pour favoriser l'obtention de compromis au Conseil, le gouvernement les brandit pêle-mêle, mais il se garde de distinguer les accords politiques obtenu et les initiatives simplement lancé mais loin d'aboutir et il néglige le poids du Parlement européen qui pourrait bien, à l'issue des Trilok délicat qui s'annonce ternir certains résultats déjà hâtivement annoncé venons-en au fond, comme en 2008, la présidence française fut à nouveau bouleversé par une crise d'envergure, cette fois-ci géostratégiques l'Union européenne s'est mobilisé pour répondre à l'agression russe de l'Ukraine, j'y étais il y a quelques jours, avec le président Larché, quelle tristesse mais aussi quelle résilience du peuple ukrainien sous l'impulsion française l'union a réagi vite et bien, et il le fallait pour aider militairement l'Ukraine sanctionner la Russie en 5 paquets accueillir 5 millions de réfugiés ukrainiens leur accorder une protection temporaire et une aide humanitaire réorienter son approvisionnement énergétique, cette crise ukrainienne a-t-elle interférer avec les priorités de la présidence française, paradoxalement, on peut considérer qu'elle a plutôt servi l'ambition française d'amener l'Europe à se penser comme une puissance, elle a en effet donné des arguments à l'impératif de souveraineté stratégique pour lequel la France plaidait depuis longtemps et que refuser d'entendre certains États membres, mais ne nous réjouissons pas trop vite ainsi en matière de défense l'activation de la Facilité européenne pour la paix et l'adoption de la boussole stratégique, le renforcement des investissements européens de la Défense, décidé à Versailles sont autant d'étapes décisives mais le retour en force de l'OTAN et leur équipement militaire accélérée des États profite surtout aux États-Unis. Et rien ne garantit que l'effort d'investissement annoncé à l'industrie militaire européenne, monsieur le président. En matière d'énergie, les importations de charbon et pétrole russes sont bannis, un partage solidaire des installations de stockage et des réserves stratégiques de gaz sont prévues, le développement des énergies renouvelables sera accéléré, mais ceci ne suffira pas à rendre l'Europe souveraine, cela pourrait même la faire entrer dans de nouvelles dépendances déjà par rapport à des fournisseurs alternatifs d'énergie fossile, mais aussi par rapport à la Chine dont l'Europe a besoin pour se doter des batteries électriques et des panneaux photovoltaïques requis pour ses ambitions climatiques en matière spatiale, le volontarisme français accélérer la décision de mettre en place une constellation de connectivité sécurisée européenne, c'est un élément important de souveraineté, mais là aussi, ne sais non pas au triomphalisme, car il y a encore un long chemin à parcourir, technologique et financier et nous espérons que notre lanceur Ariane 6 dans le cadre de la préférence européenne sera prêt et disponible pour la mise en place de cette constellation. Autre avancée valorisé par le gouvernement, les nouveaux outils de régulation au service de la souveraineté numérique les accords sur les textes DSA et DMA qui régule Services et marchés numériques sont aussi une bonne nouvelle pour freiner la la domination pardon des grandes plateformes mais au plan industriel, ne rêvons pas, rien ne dit par exemple que le European Chips acte permettra d'augmenter la production européenne de puces d'effort financier européen pourrait là encore bénéficier à des entreprises étrangères, même si ce matin, nous avons entendu les annonces, porté par la présidence sur les investissements en en France surtout le développement d'écosystèmes industriels européens reste entravées par le statu quo des règles de concurrence européenne qui empêchent toujours les concentrations nécessaires à l'émergence des champions européens. Plus grave que les zones d'ombres sont les angles morts de la présidence française le 1er à mes yeux, c'est la souveraineté alimentaire, il est frappant de n'y trouver aucune allusion dans le bilan publié par le gouvernement sur son semestre de présidence en dépit de nos demandes répétées, en dépit de l'électrochoc du Covid, puis de celui de la guerre en Ukraine, la nouvelle PAC reste redonner reste ordonné à son verdissement et délaissent les objectifs de production et ce malgré le spectre de pénurie alimentaire mondial. 2ème silence inquiétant de la présidence française, la sécurité aux frontières européennes, la France vient de perdre la direction de l'agence la plus puissante de l'Union européenne, l'agence Frontex, son directeur exécutif a démissionné abandonné en rase campagne par notre gouvernement, il ne suffisait pas de des embourber les négociations sur le projet de pacte Asile immigration il aurait aussi fallu affirmer haut et fort que la mission de Frontex et de surveiller les frontières extérieures dans le respect des droits fondamentaux, non pas de contrôler le respect par les États membres des droits fondamentaux, une autre agence européenne s'y emploie déjà. 3ème lacunes de la présidence française, la zone Euro, le débat attendu sur l'évolution du pacte de stabilité et de croissance n'a pas eu lieu, les écarts de Tours et apparaissent, à la faveur des dettes Covid et de l'inflation et menace la cohésion de la zone Euro en outre l'union bancaire ne progresse pas son 3ème, pilier, la garantie des dépôts fait cruellement défaut, je m'inquiète enfin de notre crédibilité sur les marchés dès lors que l'Union n'a toujours pas finalisé les nouvelles ressources propres qui permettront de rembourser le plan de relance européen. 4ème négligence française l'appartenance, c'était pourtant l'un des 3 axes que le gouvernement avait retenu pour sa présidence les urgences du moment ne doivent pas nous détourner de cet impératif qui consiste qui conditionnent consolider l'adhésion populaire au projet européen, spécialement parmi pour pour les jeunes et ce d'autant plus que l'Union entend s'élargir encore, cela passe par une démocratisation de l'Union européenne, à laquelle les parlements nationaux peuvent contribuer au 1er chef c'est précisément sur cette dimension parlementaire que je veux conclure car la présidence française n'a pas été seulement l'affaire du gouvernement, elle a été aussi, elle a aussi mobilisé le Parlement et au 1er chef le Sénat qui a assuré la continuité parlementaire au long du semestre, nous avons oeuvré au renforcement du rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne afin de rendre son fonctionnement plus démocratique après un colloque universitaire organisé ici sur ce thème dès décembre dernier, j'ai porté avec mon homologue de l'Assemblée nationale une redynamisation de la Kosac conférence qui réunit les organes par le du des parlements nationaux, spécialisés dans les affaires de l'Union, nous avons innové en lançant en son sein de groupes de travail, celui que je présidais s'est consacré au rôle des parlements nationaux dans l'Union et au terme de 4 mois de travail intensif entre parlementaires de toute l'Union, il a pu adopter des conclusions le 14 juin dernier parmi les 14 propositions avancées par ce groupe, je souhaite en souligner de, d'une part, la mise en place d'un droit d'initiative commun et indirects des parlements nationaux ou carton Vert, nous proposons un dispositif concret directement applicable sous réserve que la Commission européenne en accepte le principe. Seraient ainsi reconnus aux Parlements nationaux un rôle actif dans la construction européenne, d'autre part, un droit de questionnement écrit des institutions européennes pour les présidents des commissions des Affaires européennes de chacune des 2 chambres, sur le modèle de celui dont disposent les eurodéputés un tel outil nous permettrait de mieux participer au contrôle des politiques européennes, autant de voies d'avenir que nous espérons voir prospérer, Madame la Ministre, sous les prochaines présidences, je vous remercie. Dans la suite du débat, la parole était aux orateurs des groupes et nous commençons par le président Pierre Laurent. Pour. Il va s'exprimer pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le président, Mesdames les Ministres, chers collègues, le choix d'assumer la présidence française en pleine campagne électorale étaient discutables, mais une fois fait, cela a pu, cela aurait pu avoir du sens, il s'était agi d'ouvrir un grand débat démocratique sur l'avenir de l'Union dans un moment historique crucial, mais une fois encore, le débat n'a pas eu lieu la non campagne électorale du président en France et une conférence sur l'avenir de l'Europe demeure et clandestine pour la grande majorité des Européens ont scellé le sort, c'est la guerre, en Ukraine, qui a tout bousculé, diront certains, c'est vrai, l'agression russe a changé la donne, mais elle aurait dû renforcer l'exigence de refondation européenne pour rebâtir la puissance d'avenir que revendiquait le président Macron en ces termes : devant le Parlement européen, je cite, une Europe apte à répondre aux défis climatiques technologiques numériques mais aussi géopolitiques une Europe indépendante, on se qu'elle se donne encore les moyens de décider pour elles-mêmes, de son avenir et de ne pas dépendre des choix des autres grandes puissances mais loin d'une puissance retrouvée par une autonomie stratégique reconstruite, l'Union européenne toujours enfin fracturé sort de cette présidence en puissance passif, c'est-à-dire plus que jamais dépendante de l'action des puissances extérieures, les États-Unis auront ainsi signé sous présidence française, leur grand retour au coeur des choix européens, le président Macron promettait pour l'Europe, autonomie stratégique et reconstruction des souverainetés or avant même le déclenchement de l'agression russe en Ukraine, il était déjà écrit que l'autonomie stratégique promise dans la boussole stratégique ne serait qu'un complément de l'OTAN, 6 mois plus tard, c'est en réalité le document stratégique de l'OTAN, l'OTAN d'ailleurs que vous n'avez même pas cité une seule fois dans votre intervention madame la Ministre, le document stratégique de l'OTAN à Madrid, écrit sous la dictée américaine qui devient de fait la doctrine européenne avec à la clé, entre autres choses d'immenses perspectives de ventes d'armes américaines sur le sol européen face à une guerre qui la menace, au 1er chef l'Europe tous sont sourds tout de son sort à la politique américaine d'idées, elle, par l'obsession de la confrontation avec la Chine, la voix de l'Europe s'aligne au moment où nous aurions au contraire besoin qu'elle s'affirme et qu'elle affirme sa capacité d'initiative propre, neigeait énergétique de l'Europe est lui aussi en cause le gaz illustre par exemple un périlleux transferts de dépendance du gaz russe au gaz naturel américain, c'est un mouvement qui s'était d'ailleurs amorcé avant la guerre, d'Ukraine, entre 2016 et 2021 les importations en Europe de gaz naturel liquéfié ont été multipliées par 20 nous n'arrêterons pas là à 15 milliards de mètres m3 abrogerons l'Europe dès 2022 50 milliards de plus par an jusqu'à la fin de la décennie de quoi raviver les projets d'investissement américain massive dans les terminaux méthaniers, or 80 % de la production américaine est issu du gaz de schiste, un comble au moment où nous parlons d'ambitionner la neutralité carbone en 2050 sur 20 ans le pouvoir de réchauffement de ce gaz et 80 super 80 fois supérieur à celui du CO2 que dire encore de notre souveraineté alimentaire et de l'énième accord de libre-échange qui a été signé avec la Nouvelle-Zélande dans les derniers jours de la présidence française et j'ai une question, Madame la Ministre, le parlement français sera-t-il, à l'instar du CETA uniquement là pour constater les dégâts écologiques et économiques de ces accords de cet accord, sans jamais pouvoir en discuter comme la couche d'ozone, le paquet climat européen commence lui aussi à avoir vraiment beaucoup de trous, s'il continue d'afficher de grandes ambitions, la dimension socialement juste de cette transition ne cesse de s'étioler au fil des discussions ainsi l'adoption, la fin des immatriculations de véhicules thermiques hybrides et l'instauration d'un marché carbone pour le transport routier et le chauffage sont des bombes à retardement sociale et sociétale, dans un contexte de prix de l'essence élevé ce nouveau marché carbone aboutira de fait à une forme de taxe carbone européenne frappant sans distinction, ménages et entreprises risquant d'aggraver les précarité énergétique et les fractures face au droit à la mobilité, en effet, le Fonds social pour le climat qu'il aurait fallu dans ces conditions, massivement renforcé a été finalement plafonné à 50 milliards d'euros 100 co-financement des États la soutenabilité même des mutations de la production et des modes de vie et donc menacée. Dans ces conditions, Madame la Ministre, je vous le demande : que compte faire la France pour demander enfin la révision complète du marché européen de l'électricité une forme d'impôts de l'extérieur qui vient par le gaz et l'électricité quand allons-nous sortir de ce système, responsable d'une inflation particulièrement pénalisante, une fois encore, l'Europe sociale est restée la grande oubliée la directive sur le salaire minimum, car on parle enfin de salaire minimum en Europe, 60 ans après la création de l'Union européenne ne comporte aucune disposition contraignante reste donc risque de rester dans ces conditions, la règle en Europe, les incitations de la directive étant encore extrêmement timide, même si elles sont bienvenues Léon revenus eux continueront de battre des records en toute indécence dans toute l'Europe. Ah oui j'allais oublier, effectivement, vous l'avez cité une autre avancée majeure sociale sous présidence française, après 10 ans de négociations, elle obligera accorder au moins 40 % des postes d'administrateur dans les sociétés cotées en bourse à des dirigeantes, donc l'égalité progresse au CAC 40 c'est une bonne nouvelle, en réalité, l'Europe ne retrouve ni souffle ni ambition pour son avenir, car elle ne conçoit sa souveraineté que comme un repli ainsi vient sous présidence française d'enterrer l'esprit du pacte global pour la migration déposé il y a près de 2 ans par la Commission européenne et qui prônait la notion de solidarité obligatoire. Au contraire, le texte final avalise le recul de nos valeurs d'accueil car les migrations ne sont vus que comme une menace même la crise ukrainienne ne nous aura pas aider à réfléchir au fond sur l'avenir de cette question toute la négociation aura été menée sous la pression du courrier indigne co-signé en octobre dernier par 12 Ministre de l'Intérieur et adressée aux institutions européennes, qui a appelé au rétablissement de mur, financé par le budget de l'UE aux frontières de l'Union, l'accord obtenu reste dominé par celle du partage du fardeau migratoire, la présidence française a subi les événements et aura manqué à lancer les grands débats d'avenir. J'aurais pu certes relever les premières avancées réelles celle-là vers la reconstruction d'une souveraineté numérique au 1er rang desquels les règlements DSA et DMA mais les rêves relation sur Hubert noirci sérieusement le tableau car elle montre au fond qu'on est loin d'en avoir fini de la connivence entre les pouvoirs politique et les puissances d'argent dont les Gafam à ce propos l'Europe numérique ne peut se faire sur le dos des travailleurs des plateformes pourquoi Madame la Ministre, la France traîne les pieds sur le projet directive qui permet enfin de reconnaître la présomption de salariat et de reconnaître les droits attachés à cette présomption de salariat plus fondamentalement, le temps est venu de se préparer, il faut le craindre à une nouvelle crise financière à une récession qui menace, il faut dès lors rouvrir le débat sur la mobilisation des financements sur la mobilisation d'investissements publics massifs alors que, au contraire, nous voyons revenir le refrain de la dette et de la compression des dépenses publiques, qu'est devenu le débat promis sur la révision du pacte de stabilité, quand le Parlement pourra-t-il enfin discuter les soit disant nouvelles règles qu'on nous promet, nous ne pourrons plus longtemps, madame la Ministre, éviter d'affronter des choix politiques, seule à même de dégager les perspectives de financement nécessaires, je vous remercie.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, lors de sa conférence de presse du 9 décembre 2021, le président de la République avait présenté un programme ambitieux pour la présidence française de l'Union européenne fondée autour de 3 ambition une Europe plus souveraine, une Europe plus humaine et une Europe basée sur un modèle sur un nouveau modèle de croissance. Malgré l'éruption de la guerre sur notre vieux continent qui a bouleversé le programme que la France s'était fixé les objectifs fixés lors de la conférence du 9 décembre ont pour la plupart été atteint, nombre d'observateurs avisés qualifie donc cette présidence de réussite car 97 % des objectifs annoncés en décembre ont été atteints je pense premièrement à l'accord, l'accord final sur les textes, Emma et DSA fournissant de nouvelles armes face aux GAFA, ces 2 textes permettront de mieux anticiper les dérives abus et distorsion de concurrence des gars enfin les avancées seriez sont réelles sur de nombreux thèmes tout d'abord, sociaux, avec l'accord trouvé sur la directive relative aux salaires minimaux adéquat ou avec l'accord sur la proportion de femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse au sein de l'UE qui devra atteindre 40 % à l'horizon 2026 avancée également sur le thème de la consommation, avec la mise en place d'un chargeur unique et compatible avec toutes les marques de smartphones liseuses ou casque enfin je salue les accords trouvés à la toute fin de la présidence française sur l'état 5 textes phares du plan climat ayant pour but de réduire de 55 % nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 le tournant qu'a connu votre présidence à partir du 24 février dernier a permis de donner du corps à l'idée française de souveraineté stratégique, l'autre succès à mettre à votre crédit et le maintien de l'union des 27 États membres face à la mise en place des sanctions contre la Russie, les 27 ont fait preuve de solidarité avec l'Ukraine en sanctionnant Moscou à 6 reprises avec des embargos sur le charbon, le gaz et le pétrole, ils ont également acté les livraisons d'armes à Kiev via la Facilité européenne pour la paix, l'Union européenne a offert un refuge aux Ukrainiens fuyant les bombes russes avec l'activation d'un mécanisme d'accueil d'urgence utilisé pour la première fois de prises depuis sa création il y a 20 ans. C'est également dans ce contexte de guerre au port de l'Union européenne que les États membres ont réussi à trouver un accord, le vingt-cinq mars sur leur boussole stratégique en matière de défense d'accord initial a d'ailleurs été musclée au regard des événements auxquels notre continent fait face, l'un des enjeux derrière la définition de cette bouse boussole stratégique a été de parvenir à définir un consensus entre les 27 États de l'UE, tant sur la perception des menaces qui pèsent sur leur sécurité que sur les moyens d'y faire face ensemble. De par leur histoire, les pays européens disposent de culture stratégique différente et non pas nécessairement la même analyse la même analyse, pardon, des menaces et des priorités en matière de sécurité et de défense, la boussole stratégique consiste donc à identifier les priorités sur lesquelles les Européens sont prêts à s'investir collectivement sur les plans géopolitique et opérationnel, ce texte qui sera notre fil conducteur de la politique de sécurité et de défense européenne jusqu'en 2030 et donc une véritable avancée avancée pour un esprit européen de la défense, enfin nous avons accordé à l'à l'Ukraine et à la Moldavie, le statut de Condi dans 2 candidats à l'adhésion à l'UE le 23 juin dans un délai particulièrement rapide signal fort envoyé et à la Russie et à l'Ukraine et son peuple, je me félicite de cette décision, même si personnellement je ne suis pas un adepte de l'élargissement trop rapide, tout en, tout en regrettant qu'il n'ait pas pu être en être de même pour la Géorgie mais je pense que nous en reparlerons

dès le sommet des chefs d'État et de gouvernement de Versailles qui s'est tenu en mars 2022, la question de l'énergie avait été centrale et les États s'étaient engagés à réduire notre dépend dépendance énergétique tout en maintenant l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050 presque 4 mois après ce sommet, les inquiétudes demeurent l'un va l'invasion de l'Ukraine, a un lourd impact sur le orientation des prix énergétiques et l'action perturbatrice de la Russie sur le marché du gaz contribuent également à l'augmentation du prix des denrées alimentaires et des matières premières, les conclusions du dernier Conseil européen sur ce sujet ne sont pas rassurantes de nombreux constats ont été faits et plusieurs pistes pour atténuer la hausse des prix énergétiques ont été étudiés sans que certaines soient définitivement arrêtés alors que les réductions de livraisons de gaz russe au pays de l'Union européenne s'enchaînent, près de 12 États sont désormais touchés par des coupures unilatérales de gaz de la perte de part de la Russie et l'Allemagne restant dans une totale incertitude quant à la réactivation de son gazoduc n'Austruy, nous sommes incapables aujourd'hui de proposer des solutions efficaces et efficientes la seule avancée que nous pouvons saluer à ce stade et la décision du Parlement européen du 6 juillet dernier d'inscrire le nucléaire et le gaz parmi les énergies vertes dans l'Union européenne afin d'y attirer, attirer les investissements publics c'est privé, on nous dit que la commission travaille à un plan d'urgence de réduction de la demande d'énergie sans que celle-ci ne semble être en mesure d'arrêter des décisions dès lors, plusieurs questions s'imposent à nous, quelles pistes seront privilégiés par la France, notamment le 26 juillet prochain lors du sommet des ministres de l'énergie, comment faire pour éviter une fragmentation des nos 27 États sur cette question, quelles actions sont menées pour nous préparer dès maintenant à une réduction, voire à une coupure complète des approvisionnements russes cet hiver, les réductions de livraisons de gaz vers l'Europe, opéré ces dernières semaines par Moscou laisse craindre le pire et doivent nous pousser à nous préparer dès maintenant à une rupture complète de l'approvisionnement en cas d'interruption totale en rationnement pourrait être prononcée dès cet hiver et cela entraînerait une destruction de la demande, aux conséquences désastreuses pour nos économies, dès lors, 2 questions se posent : quel nouveau partenaire, l'Union européenne favorisera-t-elle pour sécuriser ses apports et enfin les objectifs de neutralité carbone sont-ils toujours tenable dans ce contexte, d'autre part, la présidence française de l'Union européenne a enfin vu aboutir la conférence pour l'avenir de l'Europe avec un retard d'un an, crise sanitaire oblige. Cet exercice. Inédit de réflexion et de débat sur l'avenir de l'Europe, largement encouragée par la France et plus particulièrement par le président Macron a abouti à 49 propositions pour rapprocher les institutions européennes des citoyens si lors de la remise du rapport, le 9 mai dernier un élan s'était fait ressentir le sujet n'a été que brièvement abordé au dernier conseil européen, ne laissant pas présager d'évolution rapide, les députés les les députés européens avaient pourtant voté une résolution saluant et approuvant ses conclusions et le travail de cette conférence sur l'avenir de l'Europe avait été saluée par la présidente van der Leyen l'évolution de nos institutions est une nécessité pour répondre aux défis auxquels l'Union européenne est confrontée. Quels leviers allez-vous activez pour soutenir la volonté de mettre fin à la règle de l'unanimité pour certaines décisions prises au sein du Conseil de l'Union européenne, par exemple en matière budgétaire, fiscale oh concernant la paix Ce mode de de votre très lourd peut parfois devenir un frein à l'action de l'Union européenne, l'idée de le remplacer par un système de vote à la majorité qualifiée pour une partie des décisions prises jusqu'ici à l'unanimité sur des domaines précis paraît inéluctable, surtout si l'Union européenne continue continue d'accueillir de nouveaux états membres soyez assurée, Madame la Ministre, que nous restons très attentifs aux suites qui pourront être données à ce sujet, je vous remercie. Merci, cher collègue, et maintenant le tour de parole est à Madame Véronique Guillotin, pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, on se souvient d'une présidence française de l'Union européenne en 2008, chahuté par une profonde crise financière, on se souviendra de celle de 2022 focalisée sur la tragédie ukrainienne, il y a un peu plus de 6 mois, la France avait abordé la présidence de l'Union européenne avec un grand nombre de projets à porter sur plusieurs fronts sécuritaire institutionnels climatique numérique pour le RDSE profondément attachés à la construction communautaire, tout cela allait dans le bon sens, quel bilan peut-on dresser aujourd'hui vous en avez fait le dessin madame la Ministre, et comme vous l'avez expliqué le visage de l'Europe a changé en six mois ce sont bien souvent les crises qui accélère le projet européen et qui renforce la solidarité entre les États membres, bien entendu, on ne peut pas totalement se réjouir de ce constat car s'agissant de la pandémie et de la guerre en Ukraine, le bilan humain est bien trop lourd, néanmoins, à l'évidence une des formules déployés par le président de la République dans son discours de la Sorbonne en 2010 de 2017 prendra tout son prend tout son sens aujourd'hui et je le cite : la la seule voie qui assure notre avenir, c'est la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique on doit en effet reconnaître que la souveraineté de l'Europe, inscrite à l'agenda européen de la présidence française semble prendre corps dans bien des domaines, nous adhérons tout d'abord au renforcement de la souveraineté stratégique de l'Union européenne, une orientation qui peut tout à fait s'accommoder avec les engagements que les États membres ont au sein de l'OTAN, notre groupe, salut les décisions prises au sommet de Versailles le 10 et 11 mars dernier qui donne un nouvel élan à la défense européenne, toutefois, si les États augmentent leurs dépenses militaires, la mise en place de projets capacitaire commun semblent patiner. Dans un autre domaine, la souveraineté énergétique est devenu brutalement un enjeu majeur, la présidence française a fait le voeu d'une meilleure indépendance à l'égard de la Russie, mais il revient désormais à la présidence tchèque de préparer un plan, il serait souhaitable que ce plan ne consiste pas seulement à gérer la pénurie qui se profile la question de la formation du prix du marché de l'électricité ne doit pas être tabou. En outre, ce plan de sécurisation de l'approvisionnement de l'énergie sera-t-il compatible avec l'accord sur le climat que la présidence française a réussi à boucler, disons le, le défi énergétique posé par la guerre en Ukraine et la nécessaire transition écologique pour atteindre la neutralité carbone en 2050 ne font pas nécessairement bon ménage. Je salue en tout cas le plan climat en particulier le principe tant attendu de la taxe carbone aux frontières, qui vise à imposer les normes environnementales de l'Union européenne aux entreprises étrangères exportant sur notre territoire, j'en viens à un autre défi, celui de la souveraineté alimentaire. En dehors des problématiques actuelles liées à l'Ukraine, faut-il rappeler ici dans la chambre des territoires qu'elle passe par le maintien de nos exploitations. Alors que la question des céréales est au 1er plan de l'actualité, l'enjeu agricole semble avoir été délaissés au cours de ces derniers mois. En outre, Bruxelles semble parfois prendre des décisions dans l'impact financier sur le monde agricole lui semble secondaire, je pense en particulier à la proposition de révision de la directive iodé sur les émissions industrielles qui ajoute dans son Champ d'application certaines activités non réglementés jusque là ce qui fait que 180000 185000 exploitations de bovins seraient ainsi concernées contre 20000 aujourd'hui, pour un coût estimé à 2400 euros par exploitation et par an. Bien sûr si les exploitations doivent toutes s'orienter vers des pratiques plus vertueux sur le plan environnemental, elles doivent en retour bénéficier des soutiens nécessaires à leur conversion, j'en profite pour préciser que ces soutiens doivent être plus efficaces et mieux contrôler comme vient de le souligner, le rapport de la Cour des comptes européenne, pointant les fraudes de la PAC. Mes chers collègues, je ne peux pas épuisé tous les chantiers dont s'est emparée la présidence française au cours de ces derniers mois en quelques mots, j'ajoute que le RDS applaudit la directive sur les salaires minimaux ou les 2 lois sur le numérique qui réglemente la concurrence sur les grandes plateformes et limite la diffusion de contenus illicites et ne ou violents. Mais la mesure qui est pas si symbolique que ça d'imposer un chargeur unique mesure à la fois de bon sens, mesures économiques mesures écologiques qui touchent directement les consommateurs et les citoyens, mérite d'être salué. On ne peut en revanche que regretter le véto hongrois sur la taxation minimale international des entreprises, cet épisode rappelle une fois de plus, l'urgence de passer à la majorité qualifiée pour certaines décisions, c'est une nécessité si l'Europe peut s'affirmer davantage en tant que puissance économique. Cette question d'ordre institutionnel va devenir d'autant plus prégnante que se profilent des perspectives d'élargissement de l'Union européenne à cet égard la France restera dans les annales comme le pays qui a ouvert la porte à l'Union européenne, de l'Union européenne à l'Ukraine et à la Moldavie dans ce contexte, c'était bien évidemment un devoir moral, il n'en demeure pas moins que la relance d'un potentiel élargissement devra s'accompagner d'un travail de réflexion sur les règles de fonctionnement de l'Union européenne d'une part, et sur le concept de communauté politique européenne lancée par le président de la République s'il est de nature notamment à rassurer les Balkans occidentaux, il mérite d'être précisée. Enfin, vous le savez, l'Europe du quotidien se construit aussi et j'oserais dire de manière un peu impertinente surtout sur les territoires transfrontaliers, je ne vous rappelle pas les enjeux de mon territoire, à la frontière avec le Luxembourg, sur les questions de fiscalité, de mobilité, de santé, nous aurons sur ces sujets à nous revoir les frontaliers en attendent autant de la part de l'Union européenne que du gouvernement français. Nous passons désormais le flambeau à la Tchéquie, souhaitons qu'elle fasse preuve du même volontarisme que la France pour affirmer la place de le peut être aussi, espérons que Prague puisse faire comprendre à certains de ses partenaires du Groupe de Visegrád où se où se situe leur intérêt: celui d'appartenir à un espace de paix déterminé à le rester, je vous remercie. Merci, cher collègue, le. Tours de parole revient maintenant Didier Marie pour le groupe socialiste. Et que le geste républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, tout d'abord, Madame la Ministre, je vous souhaite la bienvenue au Sénat et vous assure de l'engagement européen sans faille de mon groupe, madame la Ministre, nous sortons de 6 mois de présidence française du Conseil de l'Union Européenne et nous restons quelque peu sur notre faim, malgré des avancées notables sur lesquelles je reviendrai cette présidence que monsieur Macron voulait exceptionnel pour l'Europe, pour la France et peut-être aussi pour sa campagne électorale, l'aura été mais pour une toute autre raison en effet le 24 février la Fédération de Russie, déclenché la guerre que certains n'avaient pas voulu voir venir et agressaient sauvagement d'Ukraine. Cette nouvelle donne géopolitique a confirmé, comme la crise sanitaire avant elle, la capacité des Européens à réagir rapidement, efficacement et en restant unie, peut être même à la surprise de nombreux observateurs extérieurs, les Russes, les premiers cette situation à lever les réticences de certains États membres à l'égard des objectifs stratégiques d'autonomie et de souveraineté européenne devenue centraux et naturel du jour au lendemain, le terrible imprévu de la guerre, a joué un rôle majeur, moteur et a permis des avancées dans de nombreux domaines, paradoxalement, monsieur Poutine aura fait plus pour l'Europe en quelques semaines que les dirigeants européens n'en avait fait ces dernières années, la solidarité des 27 avec l'Ukraine n'a eu aucune difficulté à s'imposer et s'est concrétisée par un soutien humanitaire, économique et militaire massif nous saluons à cet égard la décision de conférer le statut de protection temporaire aux 4 7 millions de réfugiés ukrainiens, tout en s'interrogeant sur les suites qui seront données, si le conflit s'enlise. De même, nous nous félicitons de la mise en oeuvre pour 2 milliards d'euros de la Facilité européenne pour la paix qui a permis de fournir les armes défensives, nécessaires à la résistance ukrainienne, l'unanimité c'est aussi rapidement fait pour décider des citera successifs, de sanctions pour faire pression sur les dirigeants et assécher les sources de financement de l'effort de guerre russe sont, malheureusement, que cela ne produisent à ce jour, les effets escomptés. De même, les orientations de la boussole stratégique ont été adoptées, actant un réinvestissement militaire mais faute d'anticipation, elles le sont sous parapluie américain au sein d'une OTAN renforcée que le président de la République qualifiée pourtant en état de mort cérébrale, reste à savoir qui en sera bénéficiaire, la défense européenne ou seulement les États-Unis et leur industrie d'armement cette recherche de souveraineté et l'autonomie s'est aussi imposé dans le Champ de l'énergie, l'Europe dépendants des hydrocarbures russes s'accordant sur le boycott du charbon et du pétrole mais échouant malheureusement à se mettre d'accord sur un embargo du gaz excusez-moi, la France a fait le travail normal d'une présidence et a pu faire avancer les textes législatifs et endossé le costume de médiateur au nombre des satisfactions, on peut noter comme vous l'avez fait l'accord sur le numérique avec l'adoption des directives DMA DSA la réciprocité de l'accès aux marchés publics dans le commerce international, l'adoption du salaire minimum, l'équilibre femmes-hommes dans les conseils d'administration des grandes entreprises ou encore des progrès sur l'Intelligence artificielle d'autres succès, ont été mis en avant, mais en regardant ces accords de plus près, on reste circonspect, je pense au paquet climat-et au fond social rétréci à l'espace Schengen sur. Les aspects défensifs aux droits sociaux et à d'autres sujets dont parlera mon collègue Jean-Yves Leconte enfin notons les échecs, en particulier celui relatif à la taxation des grandes entreprises à hauteur de 15 % de leurs bénéfices, celui de la réforme du marché électricité toujours indexé sur le cours du gaz, notons que rien n'a été engagée face à la menace de stagflation et rien non plus, aucune feuille de route pour un agenda rural comme le demande la résolution du Sénat initiée par mon ami et collègue Patrice Joly. Quelques mots, madame la ministre, avant de conclure sur l'avenir de l'Europe, nous nous félicitons que l'Ukraine, la Moldavie ait obtenu le statut de candidat à l'UE et que la Géorgie n'ait pas été ignoré. Nous saluons l'initiative à l'égard des Balkans occidentaux les rassurant sur leur avenir européen nous notons avec satisfaction la levée du véto à l'engagement des négociations avec la Macédoine du Nord par le parlement bulgare, même si cela reste à confirmer, cependant, s'il est opportun d'avancer dans le processus d'élargissement à ces pays que les pressions extérieures menace, rappelons qu'il ne peut se réaliser que dans le cadre des accords de Copenhague et tout particulièrement de la primauté de l'État de droit, or à cet égard l'approbation par la Commission et le Conseil du plan de relance de la Pologne sans que toutes les garanties sur l'indépendance de la justice n'ait été donnée inquiète l'unité de l'Europe repose certes sur le dialogue politique, mais avant tout sur le respect de nos valeurs pour ce qui concerne nos relations avec les pays candidats et ceux de notre environnement proche, la proposition du président de la République d'une communauté politique européenne a reçu un accueil allant du glacial au tiède, l'avenir sous présidence tchèque nous dira si cet objectif européen non identifié prospérera pour ma part, je m'interroge sur son périmètre et sur son contenu, plus largement, c'est le fonctionnement même de l'Union qui doit être interrogé, et on ne peut que regretter l'absence de prise en compte des conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe et des appels du Parlement européen pour ouvrir le chantier d'une révision des traités pour une gouvernance renouvelée de l'Union oh les citoyens auraient tout leur rôle à jouer, madame la Ministre de la France a rempli sa mission et il convient de féliciter les diplomates qui ont travaillé mais cette présidence, c'est terminé assez loin des slogans enthousiastes du président Macron décembre 2021 puissance relance appartenance le président parle beaucoup d'Europe ne manque pas d'idées mais il y a encore loin des paroles aux actes cette présidence en demi-teinte aura plus été porté par les événements qu'elle ne les aura provoqué et elle restera malheureusement dans l'histoire comme celle qui aura vu la guerre revenu sur notre continent ces six mois nous aurons aussi rappeler que l'Europe est un collectif, forgé par la culture du dialogue politique, la recherche du consensus et une action résolue fondée sur nos valeurs, liberté, démocratie, justice sociale et responsabilité environnementale, merci. La parole est maintenant Jean-Baptiste Lemoyne, pour le groupe Rassemblement démocrates progressistes et indépendants. monsieur le président de la commission des Affaires européennes, mesdames les ministres, hein, mes chers collègues, si petit moi et, déjà, l'Union européenne n'est plus qu'elle était avant 2022, alors il s'agit pas de lancer un cocorico cocardier pour se faire plaisir, mais je constate que notre Union européenne a beaucoup progressé et par gros temps cette présidence française du Conseil de l'Union européenne, elle marque aussi l'aboutissement d'un certain nombre d'initiatives lancées auparavant par le président de la République, dès 2017 on se souvient, sur ces bancs du discours de la Sorbonne pour une Europe plus souveraine plus protectrice, et puis elle marque aussi l'arrivée à bon port de chantiers lancés ou suivi par de précédentes présidences, c'est là le jeu harmonieux de ses passage de flambeau d'un État membre à l'autre, chaque semestre et dire que certains recommandé que la France passe son tour pour cause d'élections présidentielles, comme le rappelait André Gattolin, mais je veux dire au président, hein, que, en 95, déjà, la France préside alors que des échéances présidentielles importantes avaient lieu, alors oui, le calendrier des événements a été très ramassée, mais le plus important, c'est le fond, la substance que le compte y soit et que des projets majeurs étaient enregistrés, hé bien ce succès, je reprends le terme de Madame la Ministre, historique, hé bien il revient bien au président de la République, épaulé, bien sûr, de l'ensemble de ses ministres de vous-mêmes, Mesdames les Ministres de vos prédécesseurs, Jean-Yves Le Drian, Clément Beaune du secrétaire général de la présidence française, je pense à toutes les équipes animées par Xavier Xavier Lapeyre de Cabanes à à notre représentation permanente naturellement sous l'égide de Philippe Léglise Costa du SGA E de l'ensemble des agents mobilisés au Quai d'Orsay dans les autres ministères de notre haute assemblée aussi vous l'avez rappelé président sans oublier les collectivités locales qui ont mis beaucoup d'engagement et de coeur dans l'accueil des événements, je peux en témoigner, a-t-il personnelle pour les maires des bonnes villes de peau de Dijon, cher François Patriat ou de Montpellier, sans oublier Strasbourg, plus que jamais capitale européenne cher Ludovic. Alors relance puissance appartenant, c'était le triptyque de cette présidence et en effet, si elle a commencé sous le signe de la relance post-Covid on l'a vu très vite l'agression russe sur le Sol d'Ukraine, le retour de la guerre sur le sol européen, hé bien au fait que les thèmes de puissance et d'appartenance, ont été au coeur de l'action conduite par cette présidence française et en européen cela rejoint le fil rouge que le Tir, le président de la République depuis 2017, celui d'une souveraineté d'une indépendance européenne accrue et c'est l'idée tout simplement que nous reprenions le contrôle en européen et non pas, comme ça a été tenté de l'autre côté de la Manche en solitaire et que en européen, nous ne soyons pas des objets de l'histoire qui s'écrit, mais que nous soyons bien des sujets qui maîtrisons notre propre destin et notre avenir, tout cela, c'est le président s'inscrit dans un contexte mondial marqué naturellement par ce conflit en Ukraine par également, on le voit dans l'environnement mondial le barycentre qui se déplace vers le Pacifique sur fond de rivalité sino-américaine et puis par l'urgence climatique qui taraude naturellement encore et toujours nos nos sociétés, hé bien tout au long de cette présidence française, l'Union européenne, ses États se sont affirmés en tant que puissance politique et géopolitique, j'en veux pour preuve l'adoption de la boussole stratégique qui crée cette culture stratégique commune le renforcement des capacités de déploiement rapide de force, le renforcement des investissements de défense acté lors du sommet de Versailles également une meilleure tenue de nos frontières externes, avec la création du Conseil Schengen qui s'est déjà réuni 2 fois et qui permettra, je crois, d'aller toujours plus loin en la matière, en terme de coordination et puis dans ce monde marqué par le retour des empires en quelque sorte, et bien, l'Europe se pense et se projette dans toute sa vaste dimension je pense naturellement aux outre-mer cher Michel Dennemont aux régions ultrapériphériques qui font de l'Europe, hé bien, un continent au monde et qui fait que nous avons un mot à dire, une voix particulière effectivement de ce concert mondial alors que de chemin parcouru depuis la chute du mur de Berlin depuis la réunification de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est et désormais, c'est la poursuite de l'unification du continent européen qui est en marche, je ne peux m'empêcher de penser à l'un des penseurs de cette Europe Denis de Rougemont, qui disait : l'Europe unie n'est pas un expédiant moderne économico-politique, c'est un idéal qu'approuve depuis 1000 ans, les meilleurs esprits, ceux qui ont vu loin les Européens Madame la Ministre de la présidence française, Madame la Ministre, ont vu loin en effet, le statut de candidat à l'adhésion ainsi été accordé par les 27 à l'Ukraine à la Moldavie, vous l'avez rappelé c'était quelques jours après que à Kiev et vous étiez aux côtés du président de la public déjà de ces mots d'encouragement été prononcé dans un délai particulièrement rapide quel temps sur la prendra, nul ne peut le dire, mais le cap est fixé, c'est le plus important, et nous n'oublions pas l'importance des Balkans occidentaux, vous l'avez rappelé, je le sais, chère également au président Richard et comme la géographie commandent que seuls 14 petits kilomètres sépare l'Europe de l'Afrique, nous pouvons également hé bien être fier du partenariat renouvelé avec le continent africain avec ce sommet de Bruxelles en février qui a permis d'aller de l'avant en matière de sécurité d'environnement de santé de migration et puis au-delà avec l'ensemble de nos partenaires, nous avons un certain nombre de défis globaux mondiaux a relevé et très clairement, soit on y arrive ensemble lorsqu'on échoue ensemble, donc on n'a pas le choix, et ça veut dire, par exemple en matière de lutte contre le changement climatique et bien d'être aux avant-postes et par nos propres réglementations aussi de faire évoluer les réglementations des autres ensembles dans le monde et de ce point de vue-là, cette taxe carbone aux frontières, je suis persuadé, hé bien, qu'elle influera sur les réglementations dont se doteront nos partenaires reprendre le contrôle, disais-je, en termes politiques, géopolitiques, mais également en termes économiques énergétique industriel, commercial, l'Europe, à commencer par la construction économique, il serait absurde que voilà aujourd'hui en 2022 elle se fasse dicter sa loi en la matière qu'elle renonce : être une puissance économique et donc c'était très important de forger nos propres stand a d'heures de ne pas être les idiots utiles du village global et de ce point de vue là le fait d'avoir de grands projets industriels européens on pense aux batteries et on en a enclenché de nouveau sous cette présidence française en matière de santé, le fait que nous développions notre indépendance énergétique, alimentaire, le fait que, en matière commerciale, nous soyons pas également les naïfs mais que nous ayons de nouvelles règles et que ces clauses miroirs avec également l'instrument de réciprocité sur les marchés publics qui met de la, de l'équité dans la concurrence, hé bien nous avons progressé et je peux vous dire que longtemps on nous regardait de travers à Bruxelles, hé bien là, les résultats sont là être reprendre le contrôle, c'est également tout simplement s'armer face aux géants du numérique, c'est se prémunir de pratiques déloyales et de ce point de vue là l'acte sur les services numériques l'acte sur les marchés numériques, hé bien permettront justement d'encadrer les activités de réguler et c'est donc un bilan fourni, hé bien, qui s'appuie sur le respect, tant de l'unité européenne que de sa diversité en c'est, c'est notre Maxime notre devise européenne et la présidence française l'illustré de fort belle manière l'unité d'abord qui a été préservé dans toutes les prises de décision, et vous l'avez rappelé, madame la ministre, avec 6 trains de sanctions et puis la diversité donc je note aussi qu'elle était d'ailleurs revendiqué par l'ambassadeur de République tchèque, s'exprimant devant notre assemblée et c'est vrai que nous avons voulu une présidence en langue française, une présidence qui respecte le plurilinguisme, de nombreuses actions ont été conduites à la suite du rapport de Christian Lequesne, elles doivent être poursuivis, nous partons de loin de très loin et ils ont besoin, madame la ministre, de tout votre volontarisme politique pour que ces efforts soient appuyer dans la durée, très bon bilan que le groupe RDPI saluent qui est à l'honneur et au crédit de la France, nous savons pour autant qu'il reste tant et tant à faire que tous nos meilleurs voeux vous accompagnent, Madame la Ministre, ainsi que l'actuelle présidence tchèque et la future présidence suédoise, je vous remercie. Et la parole est au président Claude Malhuret pour le groupe des indépendants.

Monsieur le Président, Madame la Ministre Mesdames les Ministres Monsieur le président de la commission des Affaires européennes, mes chers collègues. Concomitante d'élections présidentielles et législatives, la présidence française du Conseil de l'Union européenne avait tout pour échouer comme beaucoup ne s'était pas privé de le faire remarquer, au point d'en demander le report. Au terme de l'exercice Urszula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, juge le résultat, je cite, exceptionnel, les chancelleries, et l'ensemble de la presse sont du même avis, même si l'air du temps est au dénigrement systématique de toute action politique, il n'y a aucune raison de ne pas le dire clairement, la PFUE s'achève par un succès. Nos diplomates qu'il faut saluer et le gouvernement ont imprimé un rythme effréné, à Bruxelles, capitale des compromis déséquilibre et les décisions chronophage, même si quelques rares dossiers manquent à l'appel désaccord majeur en ont forgé le bilan positif. Les priorités étaient clair climat numérique et social, la directive sur les salaires minimums, coeur de cibles de ces urgences a été atteint, quant au climat, à l'arraché dans les tout derniers jours, la France a su composer et trouver des terrains d'entente pour réduire collectivement nos émissions de gaz à effet de serre la vision de mon groupe et celle d'une écologie libérale de progrès et d'innovation, le travail effectué sur la sobriété énergétique et les réponses industriels associés seront des atouts importants de demain je salue particulièrement les avancées sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, exemple de l'alliance entre le développement économique et les ambitions climatiques

les réseaux antisociaux sont un Far-West où se développe complotisme et M2, l'autre c'est un écosystème de fait que News qui nos démocraties et mes jeunes et moins jeunes, à la merci du cyber harcèlement réguler les contenus avec le DSA, encadrer les pratiques commerciales avec le DMA sur les meilleurs moyens de maîtriser notre espace européen, je fais le voeu que ces textes soient applicables dès la fin de l'année et que l'on continue sans relâche à travailler sur ces sujets. La performance de ces 6 derniers mois, et d'autant plus appréciable que cette présidence a été percuté de plein fouet le 24 février par la guerre en Ukraine, l'idée de réorienter les priorités ayant été, à juste titre, écarté tout a dû être menées de front la sale guerre de Poutine a donc été la toile de fond des 2 tiers de la présidence française, elle aurait pu faire voler l'Union en éclats, elle n'a fait paradoxalement que la renforcer, Poutine voulait diviser l'Europe, il la cimente ridiculiser le temps il a retranché humilier les États-Unis ils ressuscitent Biden après le revers de Kaboul rallier à lui les régimes autoritaires, la Chine s'inquiète la Turquie montre le dans le Kazakhstan, refuse l'envoi de ces soldats, il pensait prendre l'Ukraine en 3 jours, il est embourbé pour longtemps. Le principal succès français et il faut y associer la présidente de la commission a été dans des circonstances difficiles avec certains partenaires à la limite du chantage de parvenir à maintenir l'unité des 27 de décider de sanctions communes de réunir une aide militaire et humanitaire efficace à l'Ukraine et enfin de renforcer la cohésion avec les États-Unis et l'ensemble des démocraties. La prochaine étape sera plus difficile, Poutine le sait : il attend et il espère, elle consiste à relever le défi du long terme quand la guerre va peu à peu affecté l'économie aggraver l'inflation et le coût de la vie, augmenter les dépenses d'énergie. Le défi sera de tenir face aux opinions publiques quand tu la mauvaise petite musique bien sûr renforcé par tous les trolls les bottes et les trash médias de la 5ème colonne des Le Pen des Zemmour et des Mélenchon viendra susurrer que la guerre coûte trop cher et que tout n'est pas noir et blanc et qu'après tout ce n'est pas notre guerre alors que bien sûr elle est seule des naïfs ou des agents de désinformation peuvent croire le contraire. Poutine vient enfin d'avouer lors de la célébration du 300 50ème anniversaire de Pierre Legrand, que la guerre en Ukraine n'a rien à voir avec la supposée menace occidentale que dénoncent depuis des années ses affidés il apporte lui-même la réponse claire et définitive à tous les idiots utiles qui répète depuis des mois que la Russie n'a fait que répondre aux menaces de l'Europe et de l'OTAN, je cite, l'Ukraine fait partie de la propre histoire de la culture et de l'espace spirituel de la Russie après Pierre le Grand et je cite encore : c'est maintenant notre tour de reprendre et renforcer ce qui appartient à la Russie, la guerre en Ukraine n'est rien d'autre qu'une tentative d'annexion ethno-nationalistes comme en témoigne : depuis 2 jours, la délivrance de passeports russes aux Ukrainiens et c'est le fauteur lui-même de cette guerre qui vient de l'annoncer, le masque est tombé. La guerre vient enfin d'apporter de l'eau au moulin du président de la République qui ne cessent depuis 5 ans, de plaider en prêchant jusqu'alors dans le désert pour l'Europe puissance, c'est là encore un des plus grands échecs de Poutine, avoir ouvert les yeux à des centaines de millions d'Européens qui croyait que la guerre était une relique du passé et qu'ils étaient parvenus à la paix perpétuelle de compte alors qu'il n'était qu'en train de préparer leur sortie l'histoire, l'Europe s'est engagée dans son réarmement et à adopter sans ciller la boussole stratégique proposée par Emmanuel Macron espérons que cette leçon sera retenue plus longtemps que toutes celles qui disparaissent au gré d'une actualité qui ne fait plus qu'exacerber les émotions et s'évanouir la mémoire. Il reste que l'Union devra se garder de céder à la tentation d'un gaullisme du pauvre qui n'a rien à voir avec le gaullisme et qui conduirait à prêcher la médiation voir l'équidistance entre Amérique et Russie demain entre Amérique et Chine sans comprendre qu'il y a d'un côté, le camp de la démocratie et de l'autre, celui des dictatures, cette nouvelle guerre froide verse un adversaire chinois à terme beaucoup plus puissant et inquiétant que ne l'était l'Union soviétique sera avec le climat, la menace majeure pour les générations à venir. Contrairement à ce que prétendent les tyranneaux files d'extrême droite et d'extrême gauche, ce ne sont pas les démocraties qui en sont à l'origine, mais les dictatures et les systèmes totalitaires qui portent en eux la guerre comme la nuée porte l'orage prétendre échapper à ce cadre géostratégique où il occupait une position de neutralité, comme une sorte de grande Suisse qui fut trop longtemps la tentation des Européens serait une erreur, même le jour lointain où nous serons enfin réarmer mais ce serait aujourd'hui tout bonnement une incompréhension totale des rapports de force la boussole stratégique et bienvenue, elle ne se conçoit que dans une alliance toujours plus étroite avec les démocraties extra-européenne est un rôle toujours aussi fondamentale de l'OTAN. La réussite de la présidence française du Conseil de l'Union européenne ne lève pas tous les doutes. Bien sûr. L'avenir de l'Union et problématique, les nouveaux clivages politiques se dessine désormais entre pro-européens et populistes, l'avenir de l'Europe est toujours fragile car elle continue de vivre sous un régime perpétuel de crise, les blocages institutionnels persiste, nous avons dû faire face à un Brexit qui nous hante, même après le départ du 1er minister du GATT Brexit dedans, nous vivons avec la guerre en Europe et une crise sanitaire qui n'est pas terminé. Nos prises de décision sont dans plus en plus compliqué nos valeurs sont menacés, de l'extérieur et, hélas, de l'intérieur, la conférence sur l'avenir de l'Europe n'a pas eu l'élan escompté et pour l'heure, la refondation des traités européens semblent bien compliqué mais je suis certain que le désir d'Europe sera plus fort que tout, comme l'espérait dans son essai Europa Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il nous demander de réussir à réaliser le rêve européen, je vous remercie. Madame la Ministre, chers collègues. Mon analyse va différer un peu de celle de notre collègue Maluret mais cela ne vous surprendra pas. Le fait pour la France d'occuper la présidence tournante et semestrielle du Conseil de l'Union européenne est un événement d'autant plus notable qu'il est peu fréquent. On se souvient en effet que la dernière présidence française remonte à 2008. Dans un contexte qui était déjà un contexte de crise. Rappelons au passage que la présidence du Conseil de l'Union Européenne coïncidait à l'époque avec celle du Conseil européen, elle réunissait les chefs d'État et de gouvernement ce qui conférait à Nicolas Sarkozy à l'époque, pendant le semestre, la qualité de président de cette dernière institution telle n'est plus le cas aujourd'hui, depuis le traité de Lisbonne, le Conseil européen dispose désormais d'une présidence permanente, actuellement assurée par le belge Charles Michel. Et ce n'est que par abus de langage ou facilités journalistique qu'on a pu souvent présenté Emmanuel Macron comme président du Conseil européen, voire sans crainte de l'emphase comme président de l'Europe. Il importe également de rappeler la nature véritable de cette présidence du Conseil de l'Union européenne, elle confie essentiellement au ministre concerné un rôle d'animation de modération, et le cas échéant de bons offices. Pour dégager des consensus ou des majorités et fixer la position du Conseil en vue de négociations avec le Parlement, qui dans la plupart des matières et co-législateur. C'est un rôle important certes. Mais c'est de ne pas un rôle décisionnel. Le document de synthèse du bilan de la présidence française que j'ai consulté en préparation de ce débat me semble faire un peu fi de ces réalités institutionnelles et marquée au coin de la forfanterie, voire de l'exagération. Il présente, en effet, les décisions prises par le Conseil européen, notamment en réaction à l'agression de l'Ukraine comme liés à cette présidence. Voir orchestrée par celle-ci, or, comme je viens de l'expliquer, il n'en est rien. Par ailleurs, il met au crédit de l'action de la France, l'ensemble des avancées législatives réalisés pendant le 1er semestre de cette année avec une liste impressionnante de case cochée fais fais fais comme autant de mission accomplie, or cette liste ne comporte aucun dossier traité du de bout en bout par cette présidence certains des dossiers concernés ont pu être menées à terme, sur la base d'un travail au Conseil, déjà bien engagée sous la présidence précédente, d'autres ne sont pas encore conclu et les négociations inter- à leur sujet se poursuivent aujourd'hui sous présidence tchèque. Nos représentants au conseil, appuyés par d'excellents fonctionnaires à Paris et au sein de la représentation permanente à Bruxelles ont certes fait du très bon travail, il y a de véritables succès parmi lesquels je salue particulièrement l'adoption du règlement DSA et DMA en matière numérique, l'adoption de l'instrument de réciprocité sur les marchés publics émis et des avancées importantes en vue de l'adoption d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières il y a cependant certains raccourcis audacieux pour ne pas parler de contre-vérités que je ne peux m'empêcher de relever. Je ne mentionnerait que de non madame la Ministre, la France n'est pas parvenu à favoriser la mise en place de normes de production identique pour les produits fabriqués dans l'Union européenne et les produits importés, le fameux concept de clauses miroirs concocté à Paris pour l'occasion, est considéré par la plupart des experts comme bancal et contestable du point de vue de l'OMC. Il n'a reçu de nos partenaires européens, qu'un accueil Poli pour ne pas dire froid et un rapport récent de la Commission européenne sur le sujet, incite à ne pas avoir des attentes trop importantes pour ce qui concerne sa mise en oeuvre concrète. Non, Madame la Ministre, la politique commerciale n'a pas été réorienté sous l'impulsion de la France, afin notamment de renforcer ses exigences environnementales et sociales dans les accords commerciaux. La volonté de procéder à un tel renforcement est affiché par la Commission européenne depuis des années. Le rappeur longtemps attendu qu'elle vient de publier sur le sujet, ben d'ailleurs dans ce sens. Sa lecture attentive révèle toutefois que des sanctions commerciales pour non respect de ces exigences par nos partenaires ne pourront être envisagées qu'en tout dernier ressort suivant des conditions très difficiles à réunir, et au terme de procédures lourdes et complexes. De plus, ceux-ci ne concernera que les accords commerciaux futurs et pas ceux qui ont déjà été conclus ou sont en attente de conclusion je je pense en particulier au Mercosur. les progrès réels sont donc très limités de manière plus générale, la question des accords commerciaux pose problème, tout le monde convient que la France est parvenue sous la sous sa présidence, a bloqué la conclusion de certains accords, il est toutefois devenu clair au fil des mois que la commission et la déchetterie, ainsi que le groupe des États membres les plus libre-échangiste de l'Union européenne attendait simplement l'horreur, l'annonce de la conclusion d'un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et dramatique pour notre agriculture. Elle a été faite en grande pompe par la présidente de la Commission européenne et la première ministre de la Nouvelle-Zélande le 1er juillet. C'est-à-dire dès le lendemain de la fin de la présidence française. Mieux encore, la nouvelle présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne a inscrit la relance de l'agenda européen des négociations commerciales en tête de ses priorités pour le semestre. Au titre de la concurrence économique internationale, la présidence française n'aura pas non plus été en capacité de lever tous les blocages sur la taxation minimale des multinationales et de convaincre, la Hongrie, de se joindre au consensus européen, nous sommes donc ici réduit littéralement à espérer que le gouvernement américain qui entend dénoncer la convention fiscale qui le lie à Budapest sera plus efficace sur le sujet, que la présidence française. Ceci illustre selon moi toute leur la relativité des pouvoirs qui découle d'une telle présidence. Alors les auto-congratulations sur les réalisations de la présidence française ne saurait en effet nous faire oublier que l'Europe si elle semble désormais avoir davantage conscience d'elle-même de ses intérêts et de la réalité du monde est à la croisée des chemins. Comme je l'ai dit, la France a sans doute fait du bon travail et n'a pas à rougir de son bilan. Cependant, Madame la Ministre, un peu de modestie aurait sans doute été plus raisonnable dans la présentation de ce bilan. Il est vrai que l'humilité n'est pas la qualité première de notre président, je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur Jacques Fernique, pour le groupe Écologie solidarité et territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, c'est 6 mois de présidence française du Conseil de notre Union européenne ont effectivement été lourdement marqué par un tragique imprévu, la guerre russe contre l'Ukraine n'est pas seulement l'attaque contre un pays souverain contre un peuple courageux qui défend ses droits, sa liberté, sa démocratie, elle est aussi le plus grand défi à la sécurité commune en Europe depuis mai 45, une attaque délibérée contre les principes et le mécanisme de coopération et de sécurité en Europe. La réponse solidaire et déterminée de l'Union européenne a pu surprendre ceux qui misaient sur son inertie et sa mollesse, elle se traduit concrètement par des sanctions de l'aide militaire et financière et humanitaire cet imprévu tragique a sans doute contribué à renforcer l'esprit de consensus qui marque le bilan de ce semestre oui tant avec le conseil qu'avec le Parlement, de nombreuses avancées ont été enregistrées pour autant. Il ne faudrait pas Madame la Ministre, que ce débat d'évaluation sans vote auquel le gouvernement nous invite dans les 2 chambres au titre de l'article 50 se tirer 1 de la Constitution, il ne faudrait pas que ce débat gomme les aspérités problématique : les blocages ou les régressions parfois les sujets sur lesquels on peut peiner encore à discerner deux franche d'orientation européenne d'abord je voudrais déploré les insatisfactions con par moment provoquer des absences notables de ministre français, nous savions que la collusion de notre calendrier électoral national avec l'agenda de la présidence française pourrait poser problème, la place laissée vide par des ministres français lors de certains débats thématiques au Parlement européen, concernant directement la PFUE sur des chantiers majeurs : la question de l'état de droit, par exemple, a produit un effet regrettable au moment où justement les gouvernements hongrois ou polonais tente de profiter de la forte tension internationale pour que ces mousses notre vigilance sur la pratique de l'état de droit, dont le président de la République dit pourtant qu'il est notre trésor fondée pour reprendre ses termes sur nos valeurs d'Européens qui font notre unité, notre fierté et notre force par contre avec l'accord sur le paquet climat-juste avant de passer la main, notre pays a joué incontestablement un rôle positif pour faire avancer les dispositifs correspondant au rehaussement de l'ambition climatique européenne, si on peut relever que les objectifs 2030 de progression des renouvelables ou de l'efficacité énergétique, ne sont pas encore assez dans la trajectoire des un degré et demi des accords de Paris il faut surtout dire qu'au-delà de l'affichage d'objectifs le plus compliqué, reste à faire faire bifurquer en conséquence les politiques publiques, avec par exemple la fin des subventions aux fossiles, la suppression des quotas gratuits des grands émetteurs industriels qui ne peut traîner indéfiniment faire en sorte que les territoires comme le Sénat, le demande à chaque occasion, puissent avoir les moyens de décliner efficacement ces politiques climatiques particulièrement sur les enjeux d'adaptation, je voudrais dire combien mon groupe déplore que la France n'est pas appuyé la proposition du Parlement européen pour que les ménages soient exclus du marché carbone des transports routiers et du chauffage des bâtiments. Dire aussi combien mon groupe s'inquiète du rétrécissement du fonds social pour le climat, nous savons l'importance décisive des dispositifs d'accompagnement de réduction des inégalités sociales et territoriales face à ces transitions la gestion difficile des conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine avec le renchérissement des coûts pourrait être l'occasion de hâter la sortie nécessaire de notre dépendance aux énergies fossiles, ce n'est pas l'orientation claire qui se dégage des décisions européennes, il aurait sans du tout, il aurait sans doute fallu pour répondre à la hausse des prix de l'énergie, reprendre la proposition de la Commission européenne de taxer les superprofits des multinationales de l'énergie, la fin à présent programmée des voitures thermiques neuves pour 2000 trente-cinq nous oblige à déployer enfin massivement les stratégies industrielles d'innovation, de reconversion et de formation, stratégie, seuls à même d'éviter le désastre social et économique annoncée si nous n'anticipons pas, si nous n'entendons que ceux qui s'obstinent à chercher à maintenir le plus longtemps possible un modèle industriel dépassé, c'est à mon sens d'ailleurs un un même état d'esprit dépassé qui a hélas permis aux aux tenants du gaz fossile et à ceux du nucléaire, d'obtenir un vote très politique et si peu scientifique pour labelliser durable ces énergies dans le référentiel pour la finance verte, la fameuse taxonomie qui va perdre, de ce fait, une bonne part de sa crédibilité si le pacte Vert et les ambitions européennes pour le climat et la biodiversité, ont besoin du levier de la finance, ils ont également besoin du levier décisif des pratiques agricoles, la présidence française n'a guère fait preuve de volontarisme pour actionner ce levier, bien au contraire, notre gouvernement s'évertue toujours à obtenir une déclinaison nationale à la carte de la politique agricole commune, dans le contexte du drame ukrainien, il pèse pour que soient raboter les ambitions environnementales de la stratégie européenne pour l'agriculture, cette question, on l'a entendu tout à l'heure encore a fait débat au sein de notre Sénat certes la résolution européenne de la majorité va dans votre sens, c'est pour mon groupe une fausse route sur l'accord commercial avec la Nouvelle-Zélande, non, on n'est pas encore dans la nouvelle génération annoncé des accords commerciaux vertueux pour les normes environnementales, le compte n'y est pas si la directive sur le salaire minimum a bien été géré dans les temps et permettra par ce cadre commun de lutter un peu mieux contre le dumping social, mon groupe déplore par contre le rôle de la France sur les travailleurs des plateformes l'actualité toute récente avec l'enquête du Monde et de ses partenaires, a mis en évidence la nécessité d'une loi de séparation des lobbies et de l'État pour la reconnaissance du salariat D'Aubert ou autres Deliveroo pour l'inversion de la charge de la preuve, la France pèse-t-elle vraiment dans le bon sens en Europe non, pour reprendre l'expression de notre collègue Olivier Jacquin elle freine plutôt des 2 pieds pour conclure cette appréciation des 6 mois de présidence française je voudrais insister sur 3 enjeux déterminants pour lesquels l'action de notre gouvernement n'a manifestement pas permis de progresser l'enjeu budgétaire d'abord beaucoup savent qu'il serait contre-productif de revenir aux règles budgétaires que Romano Prodi, qualifié de stupide et que ces années Covid ont achevé de disqualifier qui envisagerait sérieusement de pouvoir mener les investissements de la décarbonation et de l'adaptation dans le carcan du pacte de stabilité, le président de la République envisageait une réforme significative de ces fameux critères : où en est-elle l'enjeu des ressources propres, ensuite, nous savons que l'emprunt commun de la relance s'appuie sur une série de ressources propres à mettre en place, plus que d'autres États membres, la France avait sans doute la carrure pour faire avancer concrètement ces mises en place, l'Union européenne aurait ainsi pu être la première a entériné le projet de taxe sur les multinationales résultant de l'accord de la, de l'OCDE, l'échec face au blocage hongrois vient, hélas, renforcer l'impression qu'on traîne encore et toujours sur ses ressources propres, pourtant indispensable si on ne veut pas que le remboursement futur de la dette européenne se fasse au détriment des programmes européens et du budget existant, enfin, la conférence sur l'avenir de l'Europe et la façon dont des citoyens et des forces vives s'sont investis oblige, même si elle n'a pas eu tout à fait l'écho populaire oblige à sortir du statu quo à bouger pour plus et mieux d'Europe, à l'issue de la présidence française, les conditions sont-elles en place pour que les responsables européens engagent des réponses adaptées à la hauteur des recommandations à la hauteur des suggestions de la conférence, qui nécessite de modifier le cadre fixé par les traités, voilà, voilà, dans ces quelques minutes, notre contribution à ce débat sur cette PFUE si elle vous semble manquer de mesures en pointant davantage des insatisfactions, c'est parce qu'elle est portée soit liaisons assurées par des aspirations fortes au renforcement européen. Merci, cher collègue, et maintenant la parole est à Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, SAMU, me semble-t-il, votre première présence au plateau, Madame la Ministre, je salue aussi votre présence première présence dans, dans, dans l'hémicycle, mes chers collègues. La présidence française de l'Union européenne, ce n'est pas la présidence de l'Europe par le chef de l'État français, mais un rôle de catalyseur pour faire avancer par le Conseil européen sur les propositions de la commission arrivant en première partie de l'année 2022. il était important de faire avancer un certain nombre de dossiers pour que finalement des Trilok puisse aboutir avant la fin du mandat du Parlement européen et de la commission, c'est donc l'intérêt d'avoir à la présidence, un pays qui a une administration qui sait être efficace et comme elle l'a été, effectivement, pendant ces 6 mois, c'est la clé pour obtenir sur des sujets qui sont souvent technique désaccord ou des avancées la partie, la partie politique, bien entendu, nous avons été totalement percuté choquée par l'agression russe contre l'Ukraine, qui n'est pas qu'un événement majeur qui a obligé à s'unir pour faire, pour prendre des sanctions contre la Russie pour accélérer des élargissements pour accueillir les réfugiés qui venait d'Ukraine et pour actionner une Facilité européenne pour de de la défense pour accompagner les forces armées ukrainiennes mais cette agression remet aussi en cause plusieurs de nos fondamentaux si nous concernant, nous parlons d'abord du climat des des défis climatiques qui à lui seul, justifie le renforcement de toutes nos politiques européenne et plus de solidarité européenne le paquet, si son fief Five, bon, il a un peu avancé, mais pas beaucoup, la fin des quotas gratuits a été repoussée, pour permettre l'adoption de mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, mais la question de l'accompagnement de la compétitivité de nos entreprises à l'export, n'est pas encore totalement traiter toutefois au regard de la grille de la guerre en Ukraine, la question de la taxonomie et de la place du gaz dans celle-ci apparaît comme totalement ah d'anachronique par rapport à l'obligation à la nécessite de renforcer notre indépendance énergétique, mais aussi par rapport à ce que veut dire la guerre en Ukraine dans la remise en cause finalement du modèle de développement européen et en particulier du modèle de développement allemand avec le gaz russe depuis plus de plus de 20 ans c'est un fondamental ah fondamentale de l'Allemagne fondamentales de l'Union européenne qui est ainsi remis en cause, aux effets de la crise alimentaire et à la manière dont la PAC devra y répondre concernant les questions d'asile immigration l'approche finalement assez technique graduelle pour essayer de faire avancer le le pacte Asile et immigration proposé en 2020 par la Commission européenne, obtenu des petites avancées mais plutôt sur des textes répressifs, je pense à Eurodac même si la petite avancée qui permet d'intégrer les personnes qui débarquent de sauvetage en mer, pas comme des personnes qui arrivent et qui franchissent de manière illégale, mais de manière spécifique comme personne qui viennent d'un sauvetage en mer est une avancée qui a permis, en particulier à l'Espagne d'accepter cette évolution règlement filtrage sur lequel le Parlement européen aura encore beaucoup à dire, enfin, la déclaration de solidarité reste encore très faible puisque finalement les les pays qui l'ont signé, s'engage aujourd'hui à à peu près 8000 recolle relocalisation, ce qui ne représente pas énormément par rapport aux et d'ailleurs finalement les les accords qui ont été obtenus sur ces 2 textes reste à valider par le Parlement européen et nous savons combien un certain nombre de pays sont plus sur la ligne du Parlement européen, était initialement sur les lignes du Parlement bien et continuer à espérer que le Parlement européen fera évoluer les les acquis actuels il faut aussi espérer, Madame la Ministre, que la la la la, le, le fait d'avoir mis en pneus la la la la protection temporaire pour la première fois pour les réfugiés en provenance d'Ukraine remettra en cause certains de nos fondamentaux en matière de politique d'asile pour la première fois les personnes qui viennent demander la protection en Europe ont la liberté de circulation et ont immédiatement le droit au travail, ces 2 remarques méritent d'être prises en compte, probablement pour faire évoluer la manière dont nous abordons notre politique d'asile en Europe, il faudra en tirer tous les enseignements et ne pas simplement dire qu'il s'agit d'une exception qui ne se reproduira jamais, c'est important pour l'efficacité de notre politique d'asile je pense aussi. à feu. L'Ukraine paye le prix fort depuis 2014 parce qu'elle a choisi la voie européenne les pays des Balkans, choisissent la voie européenne depuis longtemps et l'élargissement n'avance pas. Il est. Heureux, même si c'est malheureusement dans un contexte particulièrement tragique que nous ayons pu au cours de cette présidence affirmé là quand et la candidature à l'Union européenne, de la Moldavie et l'Ukraine et pu dynamiser la candidature de plusieurs pays des Balkans occidentaux ma conviction passe par le fait que cette c'est absolument nécessaire de pouvoir aujourd'hui pour renforcer l'esprit européen de pouvoir répondre à ces peuples qui demande et qui considère l'Union européenne, comme le projet le projet de leur population pour arriver à mieux se développer et améliorer leur gouvernance, mais j'ai 2 inquiétudes : Madame la Ministre de la première sur l'état de droit, la deuxième sur l'économie européenne. Pour avoir un pour tenter d'avoir un accord sur la fiscalité minimum sur les multinationales. Des concessions ont été faites à la Pologne. Madame la ministre, il n'est pas possible de transiger sur l'état de droit, il n'est pas possible de faire, taxation contre-plan de relance sans regarder la manière dont la justice fonctionne dans ces pays, dans des pays qui refusent le parquet européen et qui ne dispose pas d'une justice indépendante, nous ne pouvons pas accepter la mise en oeuvre du plan de relance européen sans aucun sans, sans, sans aucun contrôle, enfin, sur le budget et l'économie européenne, le plan de relance qui finalement consiste à endetter l'Europe pour faire des plans nationaux qui devait être un moment à 1000 Tonia reste aujourd'hui un One shot alors que nous avons parce qu'il faut reconstruire l'Ukraine parce qu'il faut réussir la transition écologique, le besoin de ressources propres et le besoin de transformer ce plan de relance européenne, non pas en un plan pour une fois, mettant une démarche significative et de long terme qui permettra à l'Europe d'avoir une économie forte et d'être attractive, je vous remercie.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, le 9 décembre dernier le président de la République, présenter les priorités de la présidence française de l'Union européenne en abordant l'axe d'une Europe plus souveraine le président mettait en avant la stabilité et la sécurité de notre voisinage il estimait alors qu'on ne pouvait pas bâtir l'Europe de la paix si nous laissions les Balkans occidentaux dans la situation où ils étaient et appelé donc à un réengagement fort de l'Union dans la région, 6 mois plus tard, face à la nouvelle donne géopolitique en Europe, cette affirmation est plus que jamais d'actualité, mais le réengagement promis fait toujours défaut en tant que président du groupe d'amitié France-Balkans occidentaux du Sénat, je ne peux que le regretter, lors du Conseil européen, les 27 chefs d'État et de gouvernement ont accordé le statut de pays candidat à l'Ukraine et à la Moldavie face à l'agression russe, ce geste de solidarité et d'unité européenne était nécessaire. Le Conseil européen a d'ores et déjà annoncé que le chemin vers l'adhésion sera long et à raison, car la priorité est à la fin du conflit militaire à la reconstruction, puis à la mise en oeuvre progressive des acquis européens avant d'envisager toute accession à l'Union européenne, mais cette nouvelle donne a totalement bouleversé la perspective européenne des Balkans occidentaux face à ce bouleversement, quel message a été envoyé à ses États voisins de l'Union européenne, il y a-t-il eu un réengagement, comme l'avait promis le président de la République, malheureusement la réponse européenne fut faible tout juste l'Union européenne, a-t-elle réaffirmé à cette occasion son attachement total à la perspective de l'adhésion des Balkans occidentaux et un une accélération du processus. Ces conclusions du Conseil européen, donne l'impression que la région demeure au milieu du gué il y a pourtant urgence a réengagé clairement la dynamique européenne des Balkans occidentaux urgence car des signes de progrès sont envoyés par les pays des Balkans occidentaux des tensions bilatérales s'apaise, des efforts sont cibles sont opérés, pour se mettre en conformité avec la règle européenne ils doivent être récompensés urgence car l'influence des pays étrangers, comme la Chine, la Russie ou la Turquie sur la religion est grandissante, vous l'avez rappelé : Madame la Ministre, et la frustration et les tensions s'c'est guise face à l'absence de perspective européenne. L'accélération, demandé par le Conseil européen doit se traduire concrètement, Madame la Ministre, la France et les institutions européennes doivent s'engager fermement pour mettre en musique les conclusions du Conseil européen sur les Balkans occidentaux au rang d'une Europe plus souveraine, il est tout aussi essentiel, d'évoquer la question énergétique, les conséquences de la guerre en Ukraine ont confirmé, s'il en était besoin, le caractère fondamentalement stratégique de l'énergie, mais qu'il s'agisse des livraisons alternatives de gaz de pétrole liquéfié des achats communs de gaz ou de la gestion des stocks stratégiques les réponses communes élaboré pendant la présidence française, apparaissent aussi ambitieuse dans leur principe que fragile dans leur mise en oeuvre, en effet, la PFUE n'aura pas permis d'avancées décisives, je pense en particulier à l'organisation du marché de l'électricité à propos duquel le débat a été trop peu a trop à la dépendance persistante à certaines matières premières, équipements qui sont indispensables au développement des énergies renouvelables ou encore au rôle du nucléaire dont la place au sein de la taxonomie verte vient d'être confirmée in-extremis au Parlement européen, mais qui fait toujours l'objet de virulentes attaques alors qu'aucune transition énergétique ne saurait être viable sans l'atome, la PFUE n'aura pas été l'occasion de remettre le nucléaire au centre du jeu énergétique européen si l'Europe sont donc être revenu dans le secteur de l'énergie à davantage de raison, force est de constater qu'il y a là encore du chemin à parcourir, madame la Ministre, la France a un rôle moteur à jouer en la matière, elle doit se faire entendre, je vous remercie. remercie. La parole enfin état notre collègue, Guillaume Chevrollier également pour le groupe des Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a plus de 6 mois, la France avait souhaité faire de l'environnement et du climat, une priorité de sa présidence du Conseil de l'Union européenne. à l'heure du bilan le 1er constat qui s'impose et que notre pays a réussi à aboutir à un accord global sur le paquet climat de remettre l'Europe sur la trajectoire de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030, par rapport à 1990 ce résultat était loin d'être évident compte tenu de la taille du paquet proposé et de son caractère structurant et des positions parfois très divergentes entre États sur le texte, le composant. Sur le fond, on peut par ailleurs se satisfaire globalement des orientations générales du vous avez parlé, Madame la ministre d'avancée majeure qui correspondent pour beaucoup au point d'attention que le Sénat avait mis en exergue dans sa résolution sur le paquet climat et dans le rapport d'information que sa commission de l'aménagement du territoire et développement durable avait consacré à la réforme du marché carbone et à la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières car le Sénat s'est investi sur la PFUE dans nos travaux, nous avions rappelé que la France devait d'une part, maintenir le niveau d'ambition générale du projet proposé par la Commission européenne en cohérence avec l'objectif de réduction des émissions de 55 et nous avions également souligné qu'elle devait, d'autre part, préserver l'acceptabilité sociale de l'ensemble du paquet, cet équilibre est globalement conservées par l'accord trouvé au conseil, notamment par la mise en place d'un fonds social pour le climat, dont la taille est probablement insuffisante pour accompagner à lui seul les ménages, notamment les plus précaires, et aussi les travailleurs mais ce fonds a le mérite d'avoir résisté aux attaques des États frugaux qui n'en voulait pas. Toutefois, le compromis de dernière minute arraché par la présidence française a été obtenue au prix de plusieurs concessions abaissant quelque peu l'ambition du paquet, nous constatons d'ailleurs que la copie rendue par le Parlement européen et plus ambitieuse ses positions correspondent d'ailleurs souvent recommandations exprimées par notre commission sénatoriale lors de ces travaux du printemps dernier. Je pense tout d'abord, au rythme d'extinction des quotas gratuits sur le marché carbone 2035 pour la fin de ces quotas, c'est tard cela retardera d'autant l'entrée en vigueur du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières que nous étions beaucoup à appeler de nos voeux. Le Conseil aurait également pu aller plus loin en intégrant à cette taxe carbone aux frontières d'autres catégories de biens par exemple les produits chimiques organiques, les plastiques ou l'hydrogène comme nous l'avions proposé et, comme le propose aujourd'hui le Parlement européen, constatons également que l'accord au Conseil ne comble pas certains angles morts comme celui des émissions du transport aérien international qui ne sont pas couvertes par le marché carbone mais par un mécanisme Corcia particulièrement peu ambitieux, le Parlement européen s'est aussi saisi du sujet en proposant détendre le marché carbone aux vols internationaux au départ de l'Union européenne, enfin on ne peut évoquer le bilan climat de l'Union européenne, sans évoquer le sujet de notre dépendance énergétique à l'heure où les centrales à charbon réouvre partout en Europe en raison du conflit ukrainien, la possibilité d'une coupure totale du gaz russe, combinée à l'arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires nous font craindre le scénario du pire pour reprendre les propos du gouvernement français, cette crise énergétique menace très sérieusement la compétitivité de nos entreprises, mais aussi l'ensemble de nos compatriotes, particulièrement les plus modestes, à l'heure où les prix de l'essence de l'électricité et du gaz ne cesse de grimper cette crise nous montrer la nécessité de développer une politique européenne cohérente sur l'énergie à la fois sur la production, mais aussi sur la consommation, notamment la lutte contre les passoires thermiques, il ne fait plus aucun doute que si nous voulons atteindre nos objectifs, climat, il nous faudra avant tout atteindre une indépendance énergétique nationale et européenne, une vraie souveraineté énergétique pour ce faire, la tâche reste importante, la 13ème PFUE n'a pas tout réglé, il reste du travail pour renforcer notre honte. Merci, cher collègue, et bien entendu la parole revient à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le président, Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je vous remercie de vos interventions de vos commentaires appréciation est question, j'ai entendu quelques compliments et je vais commencer par y répondre de façon positive, je suis en particulier, très sensible aux remerciements du président Maluret et du sénateur Lemoine je veux vous les retournez chargeant Baptiste par ce que vous avez directement contribué au succès de la PFUE comme Ministre délégué chargé notamment de la francophonie et des petites et moyennes entreprises, ainsi que du commerce extérieur vos anciennes fonctions que vous venez à peine de quitter, vous avez donc fait l'essentiel de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Vous l'avez dit l'union entre entrepris de reprendre le contrôle, une expression que j'ai entendue dans une acception bien différente jusqu'à il y a quelques semaines, de l'autre côté de la Manche et si nous faisons nôtre cette expression c'est de façon plus positive, donc je la fais volontiers mienne en l'appliquant à l'Union européenne, c'est par l'Europe que nous continuerons demain à peser dans le monde que nous pourrons pleinement protéger nos concitoyens définir De Standaard définir de choix énergétique, alimentaire industrielle numérique il y a derrière tout ça une véritable réhabilitation de la politique industrielle et de la politique économique européenne et je vous remercie pâtissent d'avoir porté ce combat dans vos anciennes fonctions. Plusieurs d'entre vous, et notamment les sénateurs Fernique Kern, la sénatrice de Cidrac ainsi que le président Rapin ont évoqué à juste titre, la hausse des prix de l'énergie, comme vous le savez, le gouvernement a mis en place ici en France, un bouclier tarifaire qui gèle les tarifs réglementés du gaz naturel et qui sera prolongée, cela a été annoncé jusqu'à la fin de l'année. La coordination et la solidarité des partenaires européens, à l'échelon européen maintenant seront déterminantes pour nous permettre de nous préparer au mieux à l'hiver prochain le gouvernement, il veillera à la commission reviendra vers nous dès le 20 juillet dès le 20 juillet avec un plan de réduction de la demande d'énergie, là encore, il sera crucial de réagir en européen solidaire, la commission a d'ores et déjà adopté une boîte à outils pour autoriser les aides d'État visant à soutenir les consommateurs et les entreprises, nous poursuivrons nos efforts. J'ai aussi entendu après des commentaires constructifs et quelques compliments. Quelques regrets s'exprimer et je dois également y revenir. Nous serions une Europe passive ou une puissance passive, Monsieur le Sénateur, Laurent. Si vous ne me croyez pas, lorsque j'affirme que cette présidence a été une réussite écoutez les autres Européens, tous les pays européens, tous les pays européens ont dit au contraire que la présidence avait été active avait permis une présidence française du Conseil de l'Union européenne comme il convient de dire en effet réussi et tous les gouvernements, ça veut dire monsieur le sénateur, les gouvernements de droite, de gauche ou du centre, tous nous félicite d'avoir fait progresser l'Europe dans une période au demeurant particulièrement difficile et même dramatique de l'avoir rendue plus forte et plus unie. Certains d'entre vous, mesdames et messieurs les sénateurs ont estimé que nous aurions manqué d'ambition sur la transition écologique, la vérité c'est que nous avons marqué, au contraire, un record d'ambition et de rapidité avec le consensus sur le paquet climat-écoutez là aussi. Le vice-président de la Commission européenne en charge de ces questions, Frans Timmermans, qui a félicité la PFUE en disant même je crois le citer exactement qu'il aurait préféré en tant que socialiste, ne pas avoir à le faire, et pourtant il l'a fait. Sur le plan social, nous aurions obtenu des avancées en trompe l'oeil c'est inexact. Si les avancées obtenues étaient si symbolique que vous semblez parfois le penser les discussions n'aurait pas fait l'objet d'années et d'années de négociations d'années d'années de blocage, j'ai cité que parfois ces textes attendait depuis 10 ans, voire 15 ans, nous sommes parvenus à convaincre, nous sommes parvenus à faire le consensus européen sur ces avancées et c'est une bonne chose, donc je crois que nous devrions nous féliciter de ce qui a été fait et nous retrouver là-dessus, reconnaître la réalité des faits. D'autres parmi vous ont évoqué l'état de droit. Il n'est pas possible de dire que la présidence française ne se serait pas battu suffisamment pour que nos partenaires, certains de nos États respectent l'État droit nous avons mené le combat contre les régressions démocratiques qui apparaissent, c'est vrai, au sein même de notre union, c'est un combat juridique, c'est un combat politique et nous le mènerons d'ailleurs autant qu'il le fera, j'ai bien entendu vos déceptions, monsieur le sénateur, Marie mais la vérité c'est que l'état de droit, a été un fil conducteur tout au long de ce semestre, en mettant à l'ordre du jour, notamment la situation de l'état de droit, en Hongrie, en Pologne, je reviendrai sur ce dernier pays, pour donner quelques précisions en étant la présidence qui a vu l'activation du mécanisme sur la conditionnalité relatives à l'état de droit, cela a été fait en adoptant des conclusions sur la protection des journalistes en finalisant un accord au Conseil sur le financement et sur le statut des partis politiques européens en soutenant une révision de la charte des droits fondamentaux pour défendre le droit à l'avortement, vous m'avez entendu rappeler la proposition du président de la République reprise désormais par le Parlement européen, nous n'avons donc éviter aucun débat, nous nous sommes enfermés dans aucun confort ne l'avons accepté aucune compromission, sous prétexte de faire avancer notre agenda législatif sur la situation en Pologne, cela fait plusieurs années maintenant que la situation de l'état de droit, en Pologne, est suivie avec une attention soutenue par l'Union européenne et en particulier par la France avec, au coeur de nos préoccupations, le constat de défaillance structurelle, notamment celles qui compromettent l'indépendance de la justice. à l'issue de longs échanges et d'une suspension du plan national de reprise et de résilience, ce qu'on appelle le PNR Bruxelles désengagement de la part de la Pologne, ont été obtenus. Des engagements qui seront vérifiés, contrôlés et c'est ainsi que, si la commission a donné dans le principe, son feu Vert au plan national de reprise et de résilience polonais, le 1er juin le 1er juillet la présidente de la commission Madame von der Leyen, indiqué que les progrès réellement effectué était insuffisant pour permettre d'aller de l'avant et donc insuffisant pour débloquer le 1er paiement au titre du PNR donc paiement qui n'a pas eu lieu pour un problème ayant trait à ces questions de justice qui sont vraiment au coeur des difficultés de l'état de droit, en Pologne, la loi ne garantissant pas l'exclusion de toute poursuite disciplinaire contre un juge qui aurait interrogé le niveau d'indépendance d'un autre juge, le dialogue se poursuivra au sein du Conseil, bien sûr, mais aussi dans le cadre de cette procédure que je rappelais fondé sur l'article 7 du traité sur l'Union européenne que nous avons mise en oeuvre et soyez assuré que nous serons vigilants. Monsieur le Président, hein, nous aurions subi un revers avec la démission du directeur français de Frontex, quelles que soient les qualités de Monsieur l'Algérie, permettez-moi de dire qu'il ne faut pas mélanger 2 choses : il y a une situation individuelle que je n'ai pas à commenter, au demeurant, puisqu'elle fait l'objet d'une enquête, enquête qui est toujours en cours et qui a conduit notre compatriote à devoir présenter sa démission, et puis d'autre part, il a le renforcement de l'agence Frontex un renforcement qui est engagé depuis des années, comme la France a toujours et depuis longtemps plaidé en ce sens et qui n'est pas facile parce qu'en effet il y a beaucoup à faire pour renforcer la maîtrise des frontières extérieures de l'Union, je suis fier, au contraire, que sous notre présidence, les réformes et tt accélérer s'agissant du recrutement de corps permanent de garde-frontières et de gardes-côtes c'est fait de l'amélioration des procédures de signalement d'incident grave, c'est fait, ou encore de la montée en puissance en matière de retour vers les pays d'origine, en appui aux États. La réforme du pacte de stabilité de croissance, a également été évoqué par plusieurs d'entre vous, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je peux vous indiquer que la Commission européenne fera prochainement des propositions, ça n'est pas un débat qui a été mis de côté propositions sur la base des orientations qu'elle avait décidé préalablement au sommet de Versailles du mois de mars et professions qui repose sur plusieurs principes auxquels nous souscrivons. D'abord, nous avons besoin d'une politique économique politique économique coordonnée pour contrer les effets de la guerre en Ukraine conforter la stratégie de relance adoptées par l'Union en juillet 2020 et d'étendre ces goulets d'étranglement qui font monter les prix, notamment les prix de de l'énergie. Cette fonction de stabilisation la commission là promet d'ores et déjà en étendant la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance, jusqu'à 2023, nous sommes donc toujours sous l'emprise de ces circonstances exceptionnelles qui ont permis à la commission de détendre cette contrainte, ensuite il faudra élaborer une trajectoire intelligente de désendettement compatible avec l'investissement dans la double transition numérique et climatique et pour cela, il sera très important de tenir compte des situations, des choix de chaque pays, chaque État membre, à l'instar de ce mécanisme d'appropriation qui a permis l'élaboration des plans nationaux de relance et de résilience, donc nous souhaitons nous inscrire dans une approche après l'urgence et après c'est flexibilité qui ont été étendu jusqu'à 2023 nous inscrit dans une approche de moyen terme qui donne à chacun la lisibilité et la prévisibilité nécessaire. L'appartenance à telle était la grande absence de notre présidence si le sénateur rap, hein, monsieur le Président, j'ai entendu vos regrets et je vous remercie de cette question parce que c'est un mot clé qui est au coeur du triptyque qu'a voulu notre présidence, ça va de Pair d'ailleurs avec la volonté de la France, de bâtir une Europe plus souveraine. Pourtant, permettez-moi de dire que les regrets que vous avez exprimé sont presque paradoxaux, au moment où plusieurs peuple ukrainien. Moldavie 1 géorgiens ont exprimé l'aspiration extrêmement forte qui est la leur, d'intégrer l'Union européenne, donc, que le sentiment d'appartenance ne soit pas qu'à l'extérieur de l'Union européenne, mais également à l'intérieur, c'est ce que nous devons encourager, c'est ce que nous avons voulu faire conscient que nous sommes, que l'Europe reste trop souvent une entité lointaine à tort d'ailleurs, mais ce qu'il faut changer, vous avez raison, c'est que nous devons conquérir les coeurs et les esprits, plus encore que nous le faisons, ça a été l'un des axes de notre présidence par les débats citoyens qui ont été voulues par elle est menée pendant un an, l'appartenance, c'est d'abord ressentir la force et la singularité de notre modèle de nos valeurs, de nos convictions, c'est de la démocratie de l'État de droit dont je parlais et des droits fondamentaux, donc à l'extérieur, l'Ukraine nous y appelle à l'intérieur, nous devons encourager le sentiment d'appropriation européen je crois tout de même, pour résumer, que, au cours de ce semestre. face à la guerre en Ukraine, le sentiment d'appartenance de tous les Européens s'est accrue et non pas aurait diminué. Pour poursuivre sur quelques interventions et questions qui ont été faites, monsieur sénateur Laurent je veux répondre à votre question sur l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas un accord mixte c'est un accord signé par l'Union européenne dans le cadre de ses compétences, donc au sens des institutions européennes, ce qui signifie que c'est donc au Parlement européen de se prononcer et il le fera, mais ce que je veux dire sur le fond, également, c'est que c'est un bon d'accord, c'est le plus ambitieux en matière de développement durable, que l'Union européenne et jamais conclu sur le modèle qui nous fait désormais envisager les accords de nouvelle génération, comme intégrant des clauses environnementales et sociales, et ça n'était pas le cas précédemment pour les accords commerciaux il protège nos filières agricoles sensibles et 200 200 Indication géographique le gouvernement s'engage bien sûr à venir vous présenter des enjeux de cet accord, j'en prends l'engagement. Sur la ruralité et plus largement l'attention donnée à la politique agricole, madame la sénatrice Guillotin, vous étiez interrogé notre action a été marqué, là encore par la guerre en Ukraine, c'est inévitable, c'est une réalité qui s'est imposé à tous, elle a permis de conforter 3 objectifs cardinaux je parlerai dans un second temps, de la PAC produire parce qu'alors que les pays du Sud sont exposés à l'insécurité alimentaire, dont la Russie porte l'unique responsabilité par son blocus par la guerre qu'elle mène par les exactions qu'elles continuent de perpétrer notre continent doit plus que jamais être un continent de production et même d'exportation, deuxièmement réduire nos dépendances, on le voit en matière agricole, nous dépendons trop souvent des intrants. Qui viennent d'ailleurs, par exemple, nous dépendons des intrants, de Russie et de Biélorussie, c'est vrai pour les engrais phosphorer, donc nous devons reconquérir là aussi notre autonomie stratégique et troisièmement, contribue à la lutte contre le réchauffement et la préservation de nos écosystèmes et la protection de la diversité, ça reste un impératif de long terme mais qui requiert des actions dès maintenant ces 3 objectifs, ne sont pas incompatibles les uns avec les autres, bien évidemment, pour ce qui concerne la PAC, chacun le sait, le 23 mars donc moins d'un mois ou un mois, disons après le déclenchement de l'invasion en Ukraine, la Commission a autorisé la mise en culture de jachères pour libérer de nouvelles capacités de production, c'est un pas, sans doute faut-il l'encourager et si la guerre de ville s'installer dans la durée, réfléchir à de nouvelles évolutions mais nous avons voulu tout de suite, permettre d'accroître les capacités de production européenne, nous devons parallèlement parce que le marché des céréales et le les marchés alimentaires d'une façon plus générale sont des marchés mondiaux veiller à maintenir le marché ouvert, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait en agissant à l'OMC, le dernier conseil ministériel de lancer le 12 juin a permis d'interdire des restrictions à l'exportation pour déjà le Programme alimentaire mondial, nous agissons aussi au sein du FIDA et en dotant le PAM de moyens supplémentaires, un dernier mot : ces 3 objectifs de production de réduction des dépendances et d'affirmation agro-écologique ne pourront aller ensemble que si nous protégeons nos marchés contre des productions qui n'auraient pas les mêmes niveaux d'exigence sociale et environnementale, et c'est cela les fameuses clauses miroirs sur lesquels la Commission a marqué sa disponibilité avancer, nous en sommes au début, je vous le concède, mais nous avons souhaité que notre présidence pose ce principe des clauses miroirs, Monsieur le Sénateur Cadec parce que la réciprocité des normes est essentiel, c'est un enjeu d'efficacité pour nos propres règles, elles permettent d'assurer que les efforts que l'on demande à nos producteurs ne se traduisent pas pour eux par une perte de Pétiti vitae, croyez-moi, nous suivrons de près ce dossier et les propositions de la commission. J'espère avoir répondu mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs à la plupart de vos observations, pour résumer, croyez bien que certains autres, les autres qu'est la modestie nécessaire à nos fonctions, je dirais même l'humidité, donc je ne tomberai certainement pas dans l'autosatisfaction, monsieur le Président, rap, hein, monsieur le sénateur Cadec en laissant penser que rien n'aurait été fait avant nous et que nous avons tout fait en 6 mois, ça n'est pas cela une présidence une présidence suppose de l'humidité de la persévérance, une vision, nous prenons l'Europe telle que on nous là, confie et nous la rendons à ceux qui nous suivent en meilleur état, si possible, c'est ce que nous avons fait, donc je veux souligner le travail de tous ceux qui nous ont précédés, je le fais volontiers comme de tous ceux qui vont nous suivre, je rappelle aussi que. Tout le travail qui a été accompli salué partout en Europe, il a été possible grâce à votre aide grâce à l'impulsion du président de la République, grâce au soutien de nos forces vives, grâce au soutien aussi de nos citoyens et je m'aperçois monsieur sénateur Marie madame la sénatrice Guillotin, que j'ai oublié de vous répondre sur un point particulier important puisque c'est là aussi, hein, des longs combats de la France, la transposition de l'accord de principe trouvé à l'OCDE sur la taxation du numérique n'a pas pu encore aboutir n'a pas pu aboutir sous notre présidence va vu que l'OCDE vient de se donner elle-même un peu plus de temps, mais le débat que vous avez évoqués et dans lequel le président de la République, vous a promis que nous n'aurions pas de tabou, le débat sur la réforme du fonctionnement d'Union européenne. Peut être sur la sortie de l'unanimité, il devra porter sur la politique étrangère, s'il n'y a pas de tabou mais devra aussi porter sur la fiscalité et là ce sont peut être des partenaires qui seront plus interrogatif que nous, pour notre part, nous souhaitons qu'il porte sur la fiscalité, soyez-en assurés, il y aura donc plein d'autres chantiers, je fais plein de confiance à la présidence tchèque et à celles, au pluriel, qui suivront pour continuer la construction d'une Europe plus souveraine plus unie et qui réponde aux attentes de nos peuples, je vous remercie. Merci madame la ministre, et je vais suspendre la séance pour quelques instants pour permettre le passage au prochain point à l'ordre du jour qui est la proposition de loi sur les contenus terroristes, je reprends la séance dans deux minutes.

La séance est donc reprise l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale a pris un engagement de la procédure accélérée portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire sur ce texte ont été publiées, elles seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. Nous pouvons donc passer à la discussion générale dans laquelle la parole est à Madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Et je crois, nous pouvons souhaiter la bienvenue. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais évidemment tout d'abord vous dire tout le plaisir et l'émotion que je ressens aujourd'hui à intervenir à cette tribune devant cette assemblée que je connais bien, comme vous le savez, j'aurai à coeur que nous puissions travailler ensemble dans un esprit de responsabilité et avec un souci permanent du dialogue depuis 2017, la France a subi 15 attentats terroristes islamistes et à travers ces actes ignobles, c'est notre République et nos valeurs qui ont été visés dans un contexte de menace très élevée, le gouvernement à la demande du président de la République s'est pleinement mobilisé dans la lutte contre la radicalisation et le terrorisme, c'est cet engagement sans faille de nos services qui a permis de déjouer 39 attaques ces 5 dernières années, à la faveur de la diffusion informatique d'une vaste propagande terroriste et de l'émergence de nouveaux moyens de communication électronique les actions terroristes sont ainsi de plus en plus le fait d'individus qui s'inspire des messages de propagande émanant des organisations terroristes, incitant au passage à l'acte en fournissant les tutoriels pour leur réalisation mais qui ne sont pas pour autant entrer en contact visible ou Direct avec des organisations réseau ou groupes terroristes depuis 2017, le gouvernement à oeuvrer avec une très grande détermination au renforcement des dispositifs de lutte contre la menace terroriste, renforcement des moyens humains, budgétaire, juridique, au profit de l'ensemble des services de renseignements des forces de sécurité, les magistrats qui mène un combat sans relâche d'abord les moyens humains et financiers, les services spécialisés en matière de lutte anti-terroriste ont depuis 2017 fait l'objet d'un effort sans précédent, au total 1900 postes supplémentaires ont été créés les Budgets d'investissement et de fonctionnement des services ont également fait l'objet d'un effort inédit, ceux de la DGSI ont par exemple pratiquement doublé entre 2015 et nos jours nous avons également créé le Parquet national antiterroriste aux fins de renforcer la force de frappe judiciaire anti- terroriste. Le cadre légal, a lui aussi également évoluer pour s'adapter, c'était l'objectif de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi Silt eux qui a introduit dans le droit commun, 4 mesures de police administrative issue de l'état d'urgence et qui ont démontré toute leur efficacité et leur pertinence, je pense au périmètre de protection à la fermeture des lieux de culte aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance de visites domiciliaires c'est dans cette même veine que s'est que s'est inscrite la loi du 31 juillet 2021 relative à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement qui a notamment pérenniser ces dispositions de la loi Silt et la technique de l'algorithme en les adaptant à l'évolution de la menace cette même loi a en outre apporté des avancées significatives aux activités des renseignements, extension des techniques de l'algorithme aux ULR expérimentation d'une technique d'interception des communications satellitaires et échange de renseignements entre services, entre parenthèses, exploitation de données brutes issues de techniques de renseignement pour d'autres finalités que celles ayant justifié leur recueil et liberté de partage de renseignements entre les services des 1er et second cercle l'action de l'État se concentre, non seulement sur le terrorisme et la radicalisation lol violentes, mais aussi sur leur terreau l'islamisme et le repli communautaire, nous avons généralisé fin 2019 dans chaque département une cellule départementale de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a porté une stratégie globale de lutte contre le séparatisme et l'islamisme, notamment à travers la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République qui est une étape majeure ces avancées doivent se poursuivre pour mieux appréhender des criminels au profil et aux méthodes qui évolue en adaptant nos outils car la majorité des porteurs de menaces détectées ces 2 dernières années ne sont pas en lien avec des réseaux terroristes structurés mais se radicalise et ça guérisse de manière isolée. à la faveur de la diffusion informatique d'une vaste propagande terroriste et de l'émergence de nouveaux moyens de communication électronique les actions terroristes sont ainsi de plus en plus le fait d'individus qui s'inspire des messages de propagande émanant des organisations terroristes, assistante au passage à l'acte en fournissant les tutoriels pour leur réalisation mais qui ne sont pas pour autant entrer en contact visible ou Direct avec des organisations des réseaux des groupes terroristes, échappant ainsi ainsi à toute capacité de détection par le biais d'une surveillance ciblée. Les enjeux de détection sont donc fondamentaux, raison pour laquelle nous avons engagé d'abord la valorisation du numéro Vert dédiée au recueil de signalement, nous devons d'ailleurs rappelé l'importance de ces signalements, car chacun doit se sentir acteur de la lutte anti-terroriste, deuxièmement, un effort accru sur la détection en ligne d'abord les moyens de Pharos, qui ont été augmentés, puis la pérennisation de la technique de renseignement de traitement automatisé de données de connexion. La circulation d'informations, de haine en ligne ne s'arrêtant pas aux frontières nationales, un règlement de l'Union européenne relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne vise à permettre le retrait des contenus terroristes en ligne en une heure maximum si les plateformes ne retire pas un contenu terroriste dans l'heure, elles doivent payer des sanctions financières allant jusqu'à 4 % de leur chiffre d'affaires pour assurer le bon fonctionnement de ce dispositif des autorité indépendante chargée d'assurer et de contrôler la légalité du retrait des contenus doivent être désignés par chaque État membre, cette proposition de loi initiée en début d'année par la députée Bono-Vandorme que vous avez enrichi en commission viendra donc renforcer notre arsenal en adaptant notre droit national au règlement européen relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne qui constitue un outil décisif contre le terrorisme en Europe, je vous remercie de votre attention. La parole est maintenant au président François Noël Buffet qui remplace notre rapporteur André Reichardt. Merci monsieur le président, effectivement je remplace autre collègue enverra charte qui est empêché pour être là cet après-midi j'ai profite de la circonstance pour saluer quand même un commissaire aux lois qui préside la séance cet après-midi de surcroît. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il me revient de finalement de vous rapportez le le 1er, texte de notre session extraordinaire et je viens de le dire à la place de notre collègue André Reichardt qui a malheureusement empêché ce texte, à certains égards est est un exemple typique d'une pratique régulièrement critiqué sur nos bancs celle en réalité d'une fausse proposition de loi, le texte a été rédigé par les directions centrales des ministères concernés, déposée par les députés du groupe majoritaire à l'époque, puis discuté au Parlement, avec pour conséquence c'est, chacun le sait maintenant, ici, sans étude d'impact ni avis du Conseil d'État, en l'occurrence il nous aurait pourtant été utile d'avoir une estimation du nombre de procédures d'injonction à venir et celle des moyens humains alloués à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, plus connu en réalité sous le nom de Pharos ou à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, plus connu sous l'acronyme comme pour traiter des nouvelles missions qui leur sont dévolues désormais par la proposition de loi, une analyse du Conseil d'État sur la constitutionnalité du dispositif aurait pu également être opportune compte tenu de la position que le Conseil constitutionnel a exprimé, lors de l'examen de la loi du 24 juin 2020 visant, rappelez-vous, à lutter contre les contenus haineux sur Internet, après-midi, il vise à adapter la législation française aux dispositions du règlement européen du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, mais notre marge de manoeuvre en réalité est assez étroite, il faut bien le reconnaître, car défini par le règlement européen lui-même, elle devrait donc faire en réalité consensus je ne reviendrai pas sur ses principaux apports mais je vous les cite tout de même retrait en une heure, possibilité d'émettre des injonctions transfrontalières et de soumettre les fournisseurs de services d'hébergement à des mesures spécifiques, ces dispositifs ne sont pas totalement nouveaux dans notre droit la France étant plus avancé que les autres pays de l'Union européenne en la matière, probablement en raison du fait qu'elle a malheureusement nous avons malheureusement été souvent la cible d'attaques terroristes, mais depuis 2015, les dispositions de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, prévoit une procédure administrative de retrait qui permettent à Pharos, de demander aux éditeurs et aux hébergeurs de retirer des contenus faisant je le site de la provocation ou de l'apologie du terrorisme ou des contenus pédo-pornographiques, s'ils ne le font pas sous 24 heures Pharos alors la possibilité de notifier la liste des adresses électroniques permettant l'accès aux contenus illicites au fournisseur d'accès Internet, afin qu'il les blocs sans délai et au moteur de recherche afin qu'il ait déférence l'articulation en fait avec le droit existant de la nouvelle procédure d'injonction de retrait a suscité quelques réserves de notre rapporteur d'André Reichardt, la proposition de loi, a fait le choix d'un système dual dans lequel les 2 procédures que existeraient, ce qui ne semble pas tout à fait respecter l'esprit du règlement européen qui vise à harmoniser la procédure et les obligations découlant des injonctions de retrait en matière de contenus à caractère terroriste finalement en pratique, il reviendrait à Faro d'articuler ces dispositifs potentiellement concurrents et de décider quelle procédure employée injonction de retrait en une heure ou demande de retrait en 24 heures nous comprenons tout à fait le choix de ne pas désarmer Pharos et de lui conserver la possibilité d'user d'une procédure déjà existantes qui a fait ses preuves en particulier pour continuer à pouvoir pour continuer à pouvoir notifié des déblocages ou des différences ment, enfin, la commission des lois circonstances nous avons souhaité renforcer la cohérence entre les 2 dispositifs en veillant à ce que les autorités concernées, soit les mêmes et en instituant une supervision de Pharos par la personnalité qualifiée de l'art, comme pour l'ensemble des injonctions de retrait, celle-ci pourra ainsi s'assurer que Pharos adopte la même pratique que les autres autorités compétentes européennes et utilisent les injonctions de retrait du règlement européen dans les mêmes cas de figure sans se reporter sur la procédure moins formaliste des dispositions de l'article 6 nous avons également étendu la compétence du suppléant de la personnalité qualifiée, c'est un peu compliqué, qui a été créé par le rapporteur de l'Assemblée nationale pour que ce suppléant puissent également intervenir pour les procédures de l'article 6 tirer hein, y compris d'ailleurs relatives au contenu pédo-pornographiques et ainsi alléger la charge de travail et la personnalité qualifiée reste un dernier sujet sur lequel pour le coup, nous avons un désaccord avec le gouvernement, c'est celui de la procédure juridictionnelle ouverte aux fournisseurs de services d'hébergement et de contenu pour contester les décisions prises par Pharos la personnalité qualifiée et l'art comme dans le cas du règlement européen, la proposition de loi initial ne prévoyait que la première instance en terme de recours j'entends avec une procédure de fond accélérer devant le président du tribunal administratif, nous avons ajouté un appel dans les mêmes délais devant le Conseil d'État, le gouvernement propose une procédure d'appel et classique devant la cour administrative d'appel dans un délai contraint d'un mois, ce point n'est pas dire il en réalité je suis sûr que nous pourrons continuer nos discussions qu'elles seront sans doute fructueuse et de trouver une solution en commission mixte paritaire, avec nos collègues députés, sous réserve des amendements auxquels la Commission a donné un avis favorable, la Commission vous demande donc d'adopter le texte issu de ces travaux, merci.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous allons parler aujourd'hui de prévention. je voudrais juste en cet instant avoir aussi une pensée particulière pour le personnel du centre de déradicalisation, de la prison des femmes de Rennes qui effectue un travail remarquable dans un centre qui est unique en France, le développement d'Internet dans nos sociétés, a multiplié l'accès à l'information, mais le caractère anonyme, simple et accessible à tous, ah malheureusement aussi favoriser l'apparition de nouveaux phénomènes tels que le cyber harcèlement la désinformation massive ou encore l'accès à la pornographie de mineurs dont nous avons ici assez souvent parlé dans la continuité des travaux précédents ayant donné lieu aux lois dites à Avia visant à lutter contre les contenus et ne et le séparatisme, confortant le respect des principes de la République, la proposition de loi que nous examinons aujourd'il vise à accentuer la sécurité de notre cyberespace plus particulièrement à assurer la protection de nos concitoyens face à la diffusion de contenus à caractère terroriste, nous avions déjà les légiférer sur ce sujet après les attentats qui ont endeuillé notre pays en 2015 et l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication peut demander aux éditeurs et aux hébergeurs de retirer des contenus relevant de la provocation ou de l'apologie du terrorisme sous 24 heures mais nous devons aller plus loin en effet le risque terroriste reste une des urgences à laquelle notre pays fait face, les différents attentats et je j'ai une pensée aussi particulière pour Samuel Paty, ainsi que les affaires quotidiennement traités par la cellule anti-terroriste montre l'urgence et l'importance d'améliorer la situation, cette menace qui pèse sur notre pays pèsent aussi sur le reste du monde, il utilise massivement Internet qui ignore toute frontière c'est pourquoi cette lutte ne peut se faire qu'à l'échelle internationale, la menace étant globale, la réponse doit l'être tout autant aussi bien militairement que virtuellement, car le cyberespace est devenue un terrain d'enrôlement si internet permet le meilleur, on sait aussi qu'il peut faciliter le pire par la diffusion de messages de haine, d'incitation au terrorisme de la recherche de cibles et bien d'autres, identifier et retirer ces contenus est un travail long, fastidieux et complexe mais il est indispensable, l'Union européenne nous offrent des moyens d'y faire face, par l'élaboration d'un règlement qui vise à contraindre les services en ligne, à supprimer des contenus à caractère terroriste en moins d'une heure sur injonction d'une autorité administrative, le règlement laisse ceci dit trois marge de manoeuvre aux États membres la désignation des autorités compétentes, le régime de sanctions que nous voulons imposer ainsi que la mise en place des procédures efficaces, il était donc nécessaire d'adapter notre droit interne aux dispositions du règlement européen du 29 avril 2021, c'est pourquoi l'Assemblée nationale a adopté une PPL sur ce thème en février, nous saluons les dispositions à l'issue de l'examen en première lecture à l'Assemblée Nationale, le texte avait été améliorée sur 3 points, comme cela a été rappelé précédemment tout d'abord l'introduction d'un suppléant au cas où l'Arcom qui est l'autorité compétente pour examiner les injonctions de retrait au cas où l'art comme ne puisse donc s'acquitter de ses obligations dans les plus brefs délais, nous souhaitons qu'il puisse y avoir un organisme suppléant, notamment dans le cas d'une notification étrangères de demandes de retrait en France, de plus, les sanctions prévues pourront être appliquées de manière plus dissuasif, c'est-à-dire directement ou en cas d'infraction habituel et non plus systématique uniquement, enfin la possibilité de permettre à l'art comme de recueillir les informations nécessaires pour mettre en place un suivi des obligations administratives qui découle du règlement européen notre commission des lois, le président vient de le rappeler apporter plusieurs modifications important et fort pertinente la semaine dernière et c'est pour moi l'occasion de saluer l'excellent travail dans l'urgence de notre rapporteur André Reichardt, tout d'abord assurer la transmission systématique à l'art comme en cas d'injonction de retrait afin d'obtenir une intervention complètes sur les procédures cité ainsi que de conserver une cohérence globale du traitement notre commission a également retenu l'abaissement de la peine de prison encourue de 3 à un an et l'harmonisation des peines encourues par les fournisseurs de services d'hébergement, le raccourcissement des délais de la suite de la procédure en fixant 72 heures le délai d'un possible appel et en abaissant le délai d'un mois, laissé au Conseil d'État, à compter de la saisie, malgré les regrets pertinent exprimée par le président de la commission des lois, sur ce que nous aurions souhaité voir inclus dans cette proposition de loi, vous l'avez deviné, Madame la Ministre, mes chers collègues, monsieur le Président, que le groupe d'union centriste votera cette proposition de loi dans la version amendée si sagement et si pertinemment par notre commission des lois, je vous remercie. Si beaucoup la parole est maintenant monsieur Jean-Yves Roux pour le RDS. Monsieur le Président, Madame la Ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, Chris cher Samuel Paty tuerie de Buffalo autant donnant ou d'événements dramatiques, associé à une diffusion de masse sur les réseaux sociaux et Internet est tenu ouvert un espace par voir comme en matière de liberté d'expression mais avec comme contrepartie terribles qui vit et faciliter la propagande terroriste les échange de contenu et ne et Viola, certains utilisateurs oublient trop souvent que leurs pseudonymes ne justifie pas d'écarter cinq conséquence, les règles les plus élémentaires, comme l'interdiction de l'incitation à la haine aussi internet ne saurait être n'est-ce pas ceux de l'endroit qui laisserait à des individus la liberté de répandre le réel en toute impunité, il existe bien entendu un arsenal juridique qui permet déjà un contrôle et des sanctions. Et leur mise en oeuvre, justifie qu'il faille mobiliser les plateformes et les supports pour qu'elle agisse avait les pouvoirs publics dans le sens d'une meilleure réglementation et d'un meilleur encadrement permis le retrait ou l'autre législation permet le retrait ou le blocage des contenus à caractère terroriste avait l'article 6 1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, lequel permet ainsi à l'administration de demander aux éditeurs ou aux aux hébergeur de retirer leurs contenus à caractère terroriste, hein, s'appuyant sur des signalements effectués sur la plateforme de signalement Pharos, ce mécanisme est efficace, je me réjouis qu'il soit bien tenu cinq que cela n'empêche d'en intégrer un nouveau telle qu'issue du règlement du 29 avril 2021 et vise à obtenir le retrait de consensus terroriste en ligne pour dans l'bien l'bien entendu, ce dispositif n'est pas neutre du point de vue du respect des libertés fondamentales, le Conseil constitutionnel avait souligné à l'occasion de la loi via comme dans le règlement européen cette loi prévoyait de réduire à une heure, le délai dont disposent les éditeurs, hébergeurs pour retirer les contenus notifié par l'autorité administrative, le Conseil avait considéré que l'atteinte à la liberté d'expression et de communication n'était pas adaptées, nécessaires et proportionnées au but poursuivi, comme chacun sait le groupe RDSE s'est toujours montré favorable au développement de la coopération européenne, nous nous réjouissons donc que sur ce point, le règlement européen est permis dans une certaine mesure de dépasser le verrue verrou constitutionnel pour des raisons certes de hiérarchie des normes, mais aussi par la garantie supplémentaire et qu'il apporte au regard du dispositif censuré de la loi via bien entendu, nous partageons les regrets du rapporteur de procédure pour eux-mêmes objets marqueront un manque de cohérence dans la construction de notre droit, même si nous comprenons aussi qui n'était pas question de faire disparaissent, la procédure initiale, puisque cette dernière a fonctionne mais derrière ce Roger il y en a un autre un tas dispositif aurait pu être pensé avec plus de temps et de recul, par le biais peut-être d'un projet de loi implique trente les analyses souvent éclairé des conseillers d'État, c'est tout particulièrement nécessaire car l'objet de législation touche les jeunes générations qui sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux et sur des réseaux qui se diversifient, il me semble d'ailleurs qu'il serait judicieux d'approfondir nos réflexions quant au dispositif imposer un encadrement encore plus renforcée de l'usage de ces réseaux par les militaires, tant s'agissant de l'accès au compte tenu, notamment, violents ou à caractère sexuel, plus de la collecte de leurs données personnelles et aussi de rechercher comment améliorer les sanctions et l'encadrement de ceux qui partagent les contenus aux mineurs, il n'en demeure pas moins chers collègues, que le groupe RDSE votera en faveur de ce texte. Merci, cher collègue et maintenant là. Parole est à Madame, Esther Benbassa comme sénateur n'appartenant à aucun groupe. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'Europe est sous le coup de la menace terroriste en permanence, il est donc nécessaire pour la France de s'aligner sur la stratégie européenne de lutte contre le terrorisme, notamment contre la propagande en ligne en effet l'espace numérique et le 1er lieu d'endoctrinement ayant travaillé sur la déradicalisation, dans le cadre d'une mission d'information sénatoriale avec Madame Catherine Troendlé je veux affirmer l'importance de la toile, les jeunes sont recrutés via les réseaux sociaux, ils trouvent leur source d'informations sur des sites douteux et communiquent entre eux sur des applications secrète et jeux vidéo, souvenez-vous de la tragédie de Christchurch de la fin, Sina de Samuel Paty qui sont le corollaire de la radicalisation sur internet, il est urgent d'établir un bouclier puissant à l'échelle européenne pour contrer cette spirale numérique, cette proposition de loi est une adaptation aux dispositions du règlement 2021 slash 784 notre législation se doterait alors de nouveaux outils de renforcement du contrôle numérique, ce texte vise aussi aussi à alerter la responsabilité des fournisseurs de services d'hébergement assujettit désormais à un régime de sanctions plus contraignant et dissuasif, bien que l'objet de cette PPL paraissait des plus louables sa substance ne sent pas satisfaire pleinement aux exigences démocratiques garantissant la liberté d'expression, internet est un espace dans les contours échappent encore aux plus aguerris d'entre nous, c'est donc avec la plus grande précaution ou d'une même d'une d'une main tremblante que nous devons intervenir dans la restriction de cette liberté au sein de cet espace si particulier, si dans le dispositif précédent 2 autorités avaient la main sur la procédure dorénavant l'Arcom année la seule exécutrice le délai d'une heure trop court pour saisir un juge, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, participe à une déjudiciarisation déjà en marche, de nombreux exemples nous appelle à la plus grande méfiance envers les moyens mis à disposition par ce texte, les algorithmes ne remplace ni l'esprit humain, ni son jugement, le législateur doit s'attacher à trouver un juste équilibre entre l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information et la protection et la sécurité des utilisateurs d'internet, je voterai pour ce texte, je vous remercie.

Monsieur le président, madame le Ministre, monsieur le président de la commission des lois et et et rapporteur l'espèce, nous apprenons à vivre avec les réseaux sociaux mais les réseaux sociaux évoluent sans cesse, nous avons découvert il y a une dizaine d'années, l'utilisation d'Internet par les islamistes radicaux, nous découvrons depuis peu que d'autres terroristes racistes masculiniste parfois homophobe était tout aussi à l'aise avec les réseaux sociaux, j'en veux pour preuve : le récent acte terroriste commis aux États-Unis, à Buffalo par un suprémaciste blanc, l'auteur a diffuser ses actes en Direct sur la chaîne t'which la vidéo concerné a été retiré en moins de 2 minutes, comme nous le rappeler, France Culture s'est considérablement moins que les dix-sept minutes qu'il avait fallu à Facebook pour retirer une vidéo similaire diffusé par le suprémaciste blanc autoproclamé qui avait tué 51 personnes dans 2 mosquées néo-zélandaise à Christchurch, en 2019, mais ces deux minutes ont suffi pour que certains copie les images concernées et les rediffusent à leur tour le temps réel constitue bel et bien un défi en ce qui concerne le contrôle de la propagation des cours du terroriste en ligne la proposition de loi que nous examinons en séance ce jour concerne ces enjeux, on s'interrogera comme beaucoup de collègues sur tous les bancs sur le véhicule législatif choisi l'adoption du règlement TCO terroriste contiennent Line nécessite l'adaptation de la législation nationale, ne pas le faire, placerait la France en contradiction avec ses obligations et engagements européens. C'est la raison pour laquelle un projet de loi s'imposer le Parlement aurait tiré profit de l'étude d'impact et, surtout, de l'avis du Conseil d'État sur la compatibilité du règlement avec notre ordre constitutionnel espérons en ce début de quinquennat et de législature à l'Assemblée nationale que cette mauvaise habitude qui avait prévalu dans le mandat précédent de l'utilisation abusive des PPL disparaissent des clarifications s'impose quant à la compatibilité entre la définition européenne des contenus à caractère terroriste, moins restrictive que celle qui prévaut aujourd'hui dans le droit français assurant leur appréciation manifeste, peut-on également considéré que la détermination illicite des contenus terroristes ne relève pas de la seule appréciation de l'administration. Dès lors que le règlement européen prévoit le contrôle une personnalité qualifiée désignée au sein d'une autorité administrative indépendante, ainsi que le recours suspensif au juge administratif, l'objectif principal recherché par la présente proposition de loi, la lutte contre le terrorisme et sa propagande n'est pas contestable, son dispositif à vocation à s'insérer dans le cadre du régime de blocage administratif en vigueur dans notre droit interne, si l'hébergeur ou le fournisseur de contenus, refuse de se conformer à l'injonction de retrait du contenu dans l'heure, une demande de blocage pourrait être adressée par l'autorité administrative au fournisseur d'accès à Internet, à l'issue d'un délai de 24 heures conformément à l'article 6 tirer hein en vigueur de la loi pour la confiance de l'économie numérique enfin soulignons à l'instar des considérants préliminaire au réglementés CO que les mesures réglementaires visant à lutter contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne doivent être complétées par des stratégies des États, visant à lutter contre le terrorisme, ces stratégies comprennent : le renforcement de l'éducation aux médias et de l'esprit critique l'élaboration de discours alternatif et de contre-discours et d'autres initiatives visant à réduire l'impact des contenus à caractère terroriste en ligne et la vulnérabilité à l'égard de ces contenus, il peut s'agir aussi que l'investissement dans le travail social des initiatives de déradicalisation et un dialogue avec les communautés touchées afin de parvenir à une prévention durable de la radicalisation dans la société, j'ai entendu et mon groupe l'a entendu les critiques qui s'interroge sur les délais laissés aux fourniture d'accès ainsi que des interrogations quant aux pouvoirs extravagants de certains algorithmes supposés régir les publications des réseaux sociaux oui, les réseaux sociaux sont parfois plus prompt à réagir en cas de non respect du Copyright qu'en cas, une diffusion de contenu supposé, inciter à la violence, j'ai évoqué tout à l'heure, mais j'ai du mal à distinguer de bons ou de mauvais élèves en la matière, vous avez peut-être comme moi, entendu parler des conséquences de l'évolution de la position des juges suprêmes sur l'avortement aux États-Unis Facebook et Instagram censure immédiatement tout poste qui tend à communiquer sur la délivrance de pilules abortives ainsi des utilisateurs ont vu leur poste du type si vous m'envoyez votre adresse je vous enverrai des pilules abortives supprimer sans attente, ils ont été choqués de découvrir que s'ils écrivaient si vous m'envoyez votre adresse je vous enverrai des armes leur communication pouvait rester en ligne sans difficulté mais la suppression des contenus de Christchurch en 2 minutes, devrait nous convaincre, convaincre les plus sceptiques que les réseaux sociaux prennent le terrorisme effectivement au sérieux, je tiens à saluer pour terminer le travail du rapporteur qui a travaillé dans une extrême urgence mais qui a contribué à éclaircir les flou qui pouvait exister en ce qui concerne la compatibilité de ce nouveau dispositif avec ce qui existait déjà en France avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique, je souligne également son souci d'aboutir à un dispositif plus stable que la tristement célèbre sur ces aspects loi Avia en conséquence notre groupe votera en faveur de ce texte telle qu'amendée par notre rapporteur. Eh bien, chers collègues, maintenant la parole est à. Ludovic aïe pour le groupe RDPI. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, il est intéressant de pour notre notre assemblée d'examiner la présente proposition de loi après avoir débattu du bilan de la présidence française de l'Union européenne, dont le volet numérique a été amplement mis en exergue dans la séance, juste avant, notamment par mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne, que je tiens à saluer ici. Largement évoqué, et pour cause : les nouvelles pratiques numériques qui sort de les possibles et peuvent gravement porté atteinte à l'ordre public nous impose d'adapter nos outils de lutte contre le terrorisme, alors nous avons tous malheureusement à l'esprit le rôle de la viralité des contenus lors de l'attentat de Christchurch notamment et de l'assassinat de Monsieur Samuel Paty. C'est indispensable adaptation a été intégré par la France qui se distingue par les outils dont elle s'est dotée pour lutter contre la diffusion des contenus illicites et plus spécifiquement à caractère terroriste. Je pense bien sûr à la commission à la loi pour la confiance dans l'économie numérique au sein de laquelle le législateur a introduit dès 2014 la faculté pour l'autorité administrative de prononcer une demande de retrait des contenus terroristes dans un délai de 24 heures je pense également, et plus récemment en 2021 à la loi, confortant le respect des principes de la République par ces dispositions validées par le Conseil constitutionnel, ce texte a notamment permis de renforcer la lutte contre les sites miroirs en facilitant notamment leur blocage sur décision de l'autorité administrative. Il a également renforcer les obligations de moyens des grandes plateformes dans la lutte contre certains contenus illicites dans la provocation et l'apologie du terrorisme, et a notamment prévu, enfin un pouvoir de sanction de régulateur qui est l'art Cette ambition, la France a porté au niveau de l'Union européenne, dont les travaux ont abouti très récemment en matière de contenu illicite au Digital Services Act dis et plusieurs mois auparavant en matière de contenus à caractère terroriste au règlement dit ici pour terroristes Quentin Online. C'est à ce règlement ici au justement du 29 avril 2021 introduisant une injonction de retrait des contenus à caractère risque dans l'heure, que la proposition de loi soumis à notre approbation aujourd'hui adapte notre droit national. Le texte a été adopté assez largement à l'Assemblée nationale puis par notre commission des lois au Sénat pour plusieurs raisons, je citerai en 1er lieu le fait que le règlement européen s'applique directement par définition de facto dans notre droit interne en l'occurrence, depuis le 7 juin dernier et fait l'objet d'un contrôle restreint de la part du Conseil constitutionnel, le cas échéant. Mais au-delà de ces considérations de forme, il faut je crois nous attacher à rappeler les garanties concrètes que prévoit le règlement, à l'issue de presque 3 années de discussions ainsi que de cette PPL, je n'en citerai là encore que quelques-unes en 1er lieu la gradually es de la procédure d'injonction de retrait des contenus à caractère terroriste en une heure, en effet, l'autorité administrative doit, sauf cas d'urgence faire le retrait au moins 12 heures en amont et en informer l'hébergeur notamment de ses procédures et dans les délais applicables des dérogations à la à l'obligation notamment de retraits sont en outre prévues en cas de force majeur ou d'impossibilité qui ne sont pas imputables à l'hébergeur ensuite via le statut d'hébergeur exposées les obligations de moyens sont proportionnées aux risques d'Exposition, les mesures prises doivent être ciblées en tenant compte de l'importance fondamentale de la liberté d'expression et d'information dans une société ouverte et démocratique. Plus généralement, les contenus à caractère terroriste visé par le règlement, ils sont clairement définies en sont expressément exclus les contenus diffusés au public à des fins éducatives journalistique, artistique ou de recherche ou à des fins de prévention et de lutte contre le terrorisme aussi le règlement impose aux hébergeurs de conserver des données pendant six mois afin de rétablir les contenus en cas d'annulation de l'injonction, par exemple, enfin les voies de recours contre les injonctions de retrait sont clairement définies au sein de la PPL, nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir au cours de l'examen s'agissant des délais de jugement et de modalités d'appel des décisions du tribunal administratif sur lesquels je ne doute pas un instant qu'un accord sera été dans la suite de la navette parlementaire, vous l'aurez compris le groupe RDPI soutient ces dispositions pour leur pertinence pour leur équilibre et leur nécessité dans la lutte contre le terrorisme, il faudra, comme cela a été dit veiller à une bonne articulation dans la pratique des dispositions de la LCN la loi pour la confiance dans l'économie numérique et dans les articles additionnels introduit. L'organisation de ces différentes dispositions marques dans le même temps l'incorporation d'un travail d'ampleur conduit à l'échelon national et européen et je tiens ici à remercier à la fois les membres du gouvernement et du précédent gouvernement pour le travail qu'ils ont pu y apporter pour reprend les termes de notre commissaire européen, Thierry Breton, tout ce qui est interdit offline doit également l'être Online ça signifie bien sûr que l'évolution du droit de l'Union dans un sens favorable progressivement étouffé doit être, doit pouvoir proscrire ce qui est hors ligne doit également être en ligne, pardon, dans le domaine des communications numériques à des fins de protection de l'ordre public, je vous remercie. Merci, cher collègue, et maintenant la parole est à monsieur Franck Menonville pour le groupe, les indépendants.

monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, au cours de cette dernière décennie lors d'attentats terroristes Internet et diverses grandes plateformes ont joué un rôle majeur, ils sont devenus malheureusement des outils essentiels de recrutement d'endoctrinement d'exhibition et de propagande, nous avons tous pu faire ce constat à l'occasion de la diffusion des vidéos de la terrible tuerie de Christian Church en Nouvelle Zélande ou au ou encore de l'odieux attentat de l'enseignant Samuel Paty désignés comme cibles sur les réseaux sociaux. Si ces espaces numériques facilitent la communication il est insupportable que des terroristes puissent y revendiqué leurs actes barbares où y faire l'apologie de leur doctrine nous avons le devoir de responsabiliser efficacement les plateformes sur les contenus qu'elle partage afin de renforcer la protection et la sécurité des concitoyens et d'éviter qu'Internet devienne un espace de non-droit, vous le savez madame la Ministre, c'est un engagement fort de notre groupe et de son président, Claude Malhuret, alors oui, la lutte contre le terrorisme et sa propagande nécessite l'implication de tous les acteurs et notamment des fournisseurs et des hébergeurs de sites aussi : je souscris pleinement aux objectifs à l'objectif poursuivi par la proposition de loi que nous examinons cet après-midi, il vise à adapter la législation française aux dispositions du règlement européen du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, entré en vigueur le 7 juin dernier il harmonise des moyens de lutte contre le terrorisme en ligne au sein de l'Union européenne, il prévoit notamment la possibilité de contraindre les services en ligne, de supprimer des contenus à caractère terroriste en moins d'une heure sur injonction d'une d'une autorité administrative d'application directe en droit français, il nécessite toutefois pour être prélèvement effectif l'adaptation de certaines dispositions et améliorations, améliorant ainsi la coopération européenne l'article unique de la proposition de loi prévoit ainsi de procéder à adaptation de notre droit national par l'ajout de 4 articles à la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ces adaptations, on vise d'une part à habiliter l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'art comme à émettre l'injonction de retrait transfrontalière prévu donc dans dans le règlement européen, elles tendent, d'autre part, a précisé les sanctions pénales applicables à l'encontre des fournisseurs de services d'hébergement par Internet qui ne respecteraient pas donc l'obligation de retrait des cons et des contenus à caractère terroriste par ailleurs des sanctions administratives et pécuniaires sont proposés en cas de non-respect des obligations diligence par les fournisseurs de services d'hébergement par l'Internet, enfin ces adaptations prévoit les voies de recours dont disposent les fournisseurs de services d'hébergement par Internet à l'encontre d'une injonction de retrait, je me félicite donc du travail accompli par la commission des Lois il a permis notamment de renforcer le rôle de l'Arcom toutefois, l'examen de cette proposition de loi appelle plusieurs remarques sur la forme en 1er lieu je regrette le choix du véhicule législatif et notamment cette proposition de loi et non un projet de loi qui nous aurait permis et qui aujourd'hui nous prive d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'État, alors même que les sujets concernés tous nos tous nos libertés fondamentales auxquelles nous sommes tous au sein de cet hémicycle particulièrement attaché, en second lieu, je m'étonne de l'examen de la proposition de loi qui permette d'appliquer le règlement européen interviennent aussi tardivement au Sénat, soit plus d'un mois après son entrée en vigueur, alors Madame la Ministre, mes chers collègues, parce que notre groupe parce que notre détermination donc à combattre le terrorisme doit être totale, il existe une nécessité impérieuse a eu à utiliser tous les leviers et les moyens nécessaires pour y parvenir, donc pour toutes ces raisons, le groupe les indépendants votera en faveur de ce texte telle qu'amendée par notre rapporteur, merci.

Merci madame la ministre, monsieur le rapporteur et président aujourd'hui, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui donc la proposition de loi déposée par nos collègues députés, consacré à la lutte contre les contenus à caractère terroriste sur Internet, comme cela a été rappelé, personne n'aurait évidemment l'idée de remettre en cause l'objectif de ce texte, nous savons ce que représente le partage en ligne des contenus à caractère terroriste partage qui contribue à entretenir la radicalisation et abouti. Dans l'horreur à des actes comme celui de Samuel Paty mais bien d'autres victimes encore nous abordons un aspect technique de cette lutte contre le terrorisme, c'est un prisme primordial important car nous avons aujourd'hui besoin de renforcer les outils indispensables pour combattre ce fléau, l'actualité nous rappelle que la menace est encore présente en France et en Europe, comme d'ailleurs l'illustre le tragique attentat qui a frappé la Norvège le 25 juin dernier au Proche-Orient Daech réorganise au travers de cellules dormantes et reste une menace au quotidien en menant des attaques nombreuses et meurtrière aux portes du continent européen au Sahel, on constate que l'instabilité socio-économique et le vide sécuritaire les groupes djihadistes toujours présent, l'idéologie du terrorisme islamiste, a pour objectif de remettre en cause nos libertés, nos valeurs républicaines, notre modèle de société, notre sécurité, il est en effet de notre responsabilité de prendre des mesures pour garantir la sécurité de nos citoyens et éviter le prosélytisme, la mesure phare de ce texte, consistant à pouvoir contraindre les entreprises du Net à supprimer des contenus à caractère terroriste, en l'espace d'une heure après injonction d'une autorité administrative est une mesure forte cependant aller à l'instar de notre rapporteur, nous ne comprenons pas le choix qui a été fait par l'Assemblée d'ajouter les nouveaux dispositifs européens à ceux déjà existants dans notre pays, il en résulte que ce sont les autorités compétentes qui devront d'elles-mêmes en assurer la coordination alors que nous faisons tous unanimement le constat citoyen comme législateur des dangers de la complexité des normes et des procédures pour notre vie démocratique, nous nous apprêtons à examiner un texte qui, une fois de plus, conduit à un enchevêtre ment de mécanismes administratifs, nous regrettons donc ce manque de cohérence et par voie de conséquence d'intelligibilité qui écorne la confiance des citoyens comme celle des acteurs économiques, nous tenons également à souligner que pour garantir l'efficacité du dispositif, il reviendra à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication d'adopter la même pratique que les autres autorités européennes et d'utiliser les injonctions de retrait du règlement européen dans les même cas de figure parmi les améliorations apportées au texte en commission, nous saluons les dispositions visant à alléger la charge de la personne des qualifiés par l'extension des compétences de son suppléant, ainsi que l'instauration de délai de recours plus contraint, il y a tout le d'espérer que les apports sénatoriaux seront maintenus dans le texte de la commission mixte paritaire, s'agissant de la question de constitutionnalité pointée du doigt, il nous semble que les garanties prévues par le règlement, comme la présente proposition de loi qui n'existait pas, ce qui a été dit dans la loi Avia permettent d'écarter ses risques d'inconstitutionnalité pour conclure, je tiens à remercier et avoir une pensée pour notre rapporteur Richard qui a travaillé la qualité de son travail malgré des délais très contraints, il lui a fallu évidemment beaucoup composé, je lui souhaite également un bon rétablissement à mon collègue pour l'ensemble de ces raisons, notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi telle qu'amendée par notre commission des lois, je vous remercie.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous avons l'agenda législatif de cette session extraordinaire par l'étude de textes sur la prévention de la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, nous ne le savons que trop la haine prolifèrent en ligne et nous devons nous doter d'un arsenal le plus efficace possible pour limiter cette propagande terroriste, ses méthodes de recrutement ayant pour but de nuire à notre République, le terrorisme, tu es Internet demeure le terreau fertile, permettant à la fois la diffusion de certaines idéologies macabre, le recrutement et le financement des terroristes, il est donc essentiel de se doter d'outils de droit freinant cette utilisation d'Internet, nous avons hélas du recul sur les enjeux et problématiques liées au contenu terroristes en ligne le règlement européen qui nous est demandé de facilité par l'adaptation de notre droit est le fruit d'une réflexion sereine, loin d'un mode caricatural ou je cite un de nos anciens présidents quand on consulte des images de jihadistes en état djihadistes heureusement ce règlement distincte de manière sensée la diffusion de certains de ses conclut à des fins journalistiques pédagogique artistique plus resterait plus équilibrée dans la définition des contenus nécessitant d'être retirés garantissant la possibilité de mettre lire des contenus dans le cadre du débat public, par exemple, il constitue un outil majeur est nécessaire pour notre législation, toutefois, la loi qui nous est proposé aujourd'hui quand il y a des limites, certaines tout d'abord le choix du une PPL, privant le contrôle a priori du Conseil d'État ne semble pas le plus sécurisant sur l'évaluation des conséquences notamment sur les libertés publiques les individuels, cette crête s'exprime au regard de la censure, qui a déjà pu exercer le Conseil constitutionnel sur des mesures proche contenues dans la loi dite Avia, ce dernier rappeler en trente que la détermination du caractère illicite des contenus à caractère terroriste ne devait pas être soumise à la seule appréciation de l'administration, le choix de l'Arcom, désigné depuis la loi sur le séparatisme comme l'opérateur pour traiter la haine en ligne démontre une cohérence mais suscite de nombreuses interrogations, comme a pu le rappeler plusieurs fois mes collègues ici présentes au Mado su et Monique de Marco dans leurs travaux de la commission culture, l'Arcom se voit confier de plus en plus de responsabilités, mais les moyens humains et financiers suivent-t-il, je sais que nous entrons dans un quinquennat sauce d'impôts ni accroissement de dettes aussi je suis impatient de voir comment à constant du gouvernement va faire pour doter l'Arcom des moyens nécessaires pour mener à bien cette nouvelle mission en nombre d'agents, mais aussi dans la formation adaptée nécessaire si j'insiste sur ce point, c'est que le drame de Samuel Paty a démontré que le circuit de signalements existe fonctionne bien mais que le manque de personnel, engrange des délais de traitement qui ont la funeste conséquences que nous connaissons tous, nous serons donc très vigilants lors du projet de loi de finances, à la rentrée reste trois autres points majeurs : d'abord l'urgence du délai d'une heure représente pour de nombreuses associations de protection des libertés risquent au-delà des erreurs techniques inhérentes à des procédures automatisées dans la sélection des contenus à supprimer mis en avant par la Quadrature du Net, de nombreuses ONG craignent de voir la mise en place de filtres de téléchargement, qui permettrait à l'hébergeur d'interdire à un utilisateur de poster du contenu ensuite la subjectivité des éditeur ou hébergeur dans l'évaluation du contenu, ces opérateurs privés en des démarches à géométrie variable selon les sujets qu'ils posent, devoir être retiré, comme l'a très bien dit Jérôme Durain nous avons vu récemment lorsque mettent la maison mère de Facebook n'a pu répondre aux différences de traitement entre plusieurs postes possiblement litigieux en effet l'associatif de presse rapporte que le journaliste ayant publié 2 annonces proposant soit une pilule abortive soit une arme à feu, a vu son 1er poste supprimé dans la minute, alors que l'autre est resté à toucher enfin l'aspect transfrontalier des demandes de retrait au vu de l'arrivée au pouvoir du régime aux valeurs parfois très éloignées de celles de notre pays au sein même de l'Union européenne, le règlement pour lequel nous adoptons, nous adaptons nos droits aujourd'hui permet des demandes transfrontalière de retraits de contenus qui pourraient être litigieuse comment sans contrôle d'un juge judiciaire, garantir la liberté d'expression sur notre territoire, face à des gouvernements parfois totalitaire caractérisant de manière caricaturale leurs oppositions comme des terroristes, il n'existe parfois que trop peu de garanties sur l'autorité compétente désignés par chaque pays membre, notamment en terme d'indépendance, certes, la procédure prévoit un droit de regard de l'Autorité nationale du pays sollicités mais la coopération entre pays à la réciprocité de leurs actions pourrait poser problème, ces inquiétudes chers collègues sont réelles, elle ne sort pas fantasmer, elle s'impose dans une réflexion globale et apaisée de la recherche qui est celle de notre assemblée d'un équilibre entre une lutte juste ferme et efficace contre la dissémination de contenus terroristes sur Internet et la protection de la liberté d'expression, cette protection, nous sommes constitutionnellement revenir au juge judiciaire hélas écarter dans les dispositifs étudier aussi toutes ses réserves nous empêche de soutenir pleinement la démarche de loi présentée écologie solidarité et territoires en responsabilité, hé bien conscient de la nécessité du besoin d'agir rapidement contre l'expansion du terrorisme via la lutte contre les contenus Internet ne s'opposera pas à cette loi et s'abstiendra. Si beaucoup et maintenant la parole est à monsieur Pierre Ouzoulias pour le CRCE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la première ministre au nom du gouvernement a pris à cette tribune, l'engagement de changer sa méthode de travail avec le Parlement, et singulièrement avec le Sénat, qu'elle souhaite devenir, je la cite une forte, une force de co-construction Madame la Ministre, vous avez la redoutable responsabilité de nous montrer pratiquement, comment le gouvernement va mettre en oeuvre cette nouvelle méthode, je ne suis pas sûr que cette proposition de loi, soit le meilleur choix pour inaugurer ses nouvelles pratiques législatif en effet la proposition de loi que vous nous soumettez a été adopté par l'Assemblée nationale le 16 février dernier son principal objet est d'adapter le droit national français ou dispositions du règlement adopté le 29 avril 2021 mais déjà appliquée dans l'Union européenne depuis le 7 juin 2022 il est singulier voir quelque peu cavalier et tout le monde debout, a dit d'utiliser une proposition de loi pour transposer les dispositions d'un règlement européen, cette méthode n'est pas respectueuse des droits du Parlement car elle le prive d'une étude d'impact et de l'avis du Conseil d'État, alors même que les juridictions administratives seraient fortement sollicités par les procédures qu'elle met en oeuvre il y a pire cette proposition reprend bon nombre des dispositifs de la loi du 24 juin 2020, visant à lutter contre les contenus et ne sur Internet, dite loi Avia et notamment sa mesure principale, obligeant le retrait des contenus et ne en moins d'une heure, le Sénat s'était fermement opposé et le rapporteur pour la commission des lois, le sénateur Christophe André Frassa avait très justement montrer que cette injonction à les renforcer le pouvoir des grandes plateformes du numérique en leur donnant un droit de censure il s'est écrié, je le cite, ce n'est pas à elle d'exercer la police de la liberté d'expression, le groupe des Républicains du Sénat avait saisi le Conseil constitutionnel sur ce texte, les sages ont censuré la quasi-totalité de ses articles, en considérant que le délai d'une heure, imposer aux hébergeurs à la liberté d'expression et de communication, une atteinte excessive, je cite son argument qui est décisif pour la présente proposition de loi l'engagement d'un recours contre la demande de retrait n'est pas suspensif et le de l'est du heure à l'éditeur ou l'hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible visés ne lui permet pas d'obtenir une décision du juge, avant d'être contraint de le retirer, nous avons, dès lors, le sentiment pénible d'examiner un texte dont la mesure principale, a déjà été censuré par le Conseil constitutionnel, vous allez nous expliquer que le règlement européen apporte aux auteurs des contenus des garanties que la loi Avia ne ferait pas par problème, je vous répondrai que les procédures de recours instituée par le règlement, peuvent être engagées après leur suppression, alors que le Conseil constitutionnel considère qu'elles doivent pouvoir l'être avant tout se passe donc comme si vous considériez, Madame la Ministre, que le règlement européen est supérieur en droit à la décision du conseil constitutionnel français, c'est un renversement total de doctrine pour lequel vous nous devez des explications, mais ce n'est pas tout : la présente proposition de loi porte transposition d'un règlement élaboré dans le cadre de la directive européenne du jus, du 8 juin 2000 relative à la société de l'information et au commerce électronique, or cette directive est très prochainement rendue obsolète par l'adoption par le Parlement européen le 5 juillet 2022 des versions définitives des de règlement sur les services numériques et sur les marchés numériques, les DSA et DMA, ces 2 textes devraient être validée par le Conseil de l'Union européenne en juillet et septembre et seront donc en vigueur avant la fin de cette année, ils introduisent dans le droit européen des nouveaux régimes pour les fournisseurs des services débarquement, les contrôleurs d'accès et tous les acteurs du numérique, enfin, l'article 14 du premier met en place des mécanismes de signalement et de retrait des contenus les sites beaucoup plus respectueux de la liberté d'expression que votre texte plutôt que de nous demander d'examiner un texte qui sera caduc avant la fin de l'année, il aurait été plus intéressant d'engager avec le Sénat, dans une démarche de co-construction, une réflexion sur l'éventuelle transposition de ces de règlements majeur pour cette raison, nous voterons contre ce texte, merci. Ah si chers collègues, la discussion générale est ainsi close et nous passons à la discussion du texte de la commission. De Paris. Madame Mercier a demandé la parole sur le l'article unique. Merci, merci, monsieur le président, Monsieur le président de la la commission des lois, madame la ministre, évidemment, je me félicite qu'on puisse retirer en une heure des contenus à visée terroriste ou pédo-pornographiques peut dans il y a une loi qui a été voté ici, à l'unanimité le 20 juillet 2020 et aujourd'hui, malgré la bonne volonté de l'art comme la bonne volonté de la CNIL, il est toujours possible pour des enfants de visionner des films pornographiques, destinés aux adultes, on ne peut pas jouer d'argent quand on est un mineur sur le Net, on peut toujours être traumatisés par des films pornographiques, encore aujourd'hui, je me demande juste jusqu'à quand nos enfants devront se protéger eux-mêmes. Monsieur Julia se demande la parole également. Oui, monsieur le président, je suis obligée de m'exprimer sur le premier article parce que c'est le seul je sollicite des réponses de votre part, madame le Ministre il y a, il y a 2 questions fondamentales que que je vous ai posé et c'est des questions de de droit bien évidemment dans cet hémicycle, nous sommes tous d'accord pour engager tous les moyens possibles pour contrer le le terrorisme mais est-ce que vous pouvez nous garantir ici maintenant que ce que nous allons voter et conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, moi je retiens de de l'argument qui a été développé ici, c'est que les collègues considèrent que

des retraits des contenus, je pense que là il y a une une différence vous savez de toute façon la loi le elle va sans doute retourner à l'Assemblée nationale, je doute qu'elle ne soit pas à un moment donné, conduite, elle aussi, devant le Conseil constitutionnel, donc il serait mieux ici de de s'entendre sur ce qu'il est possible de faire et par ailleurs sur les les 2 directives dont votre collègue Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères nous a dit très justement que c'était de pas de géant vers la réforme du numérique, il faudrait que vous nous disiez si ils seront compatibles avec ce que vous souhaitez que nous votions maintenant. merci monsieur le président avec le règlement qui est stabilisé qu'a aucune contradiction avec le texte. La discussion appelle maintenant le premier amendement. Pour La ministre va présenter le 1er amendement, il va donc pouvoir présenter l'explication souhaité présenter l'amendement de la mer, Donc l'amendement numéro 1 qui modifie l'article 6 1 de la loi qui désigne les autorités nationales compétentes pour mettre en oeuvre les procédures prévues par le règlement TCO jusqu'à présent, le grand de de cet article disposait simplement que la personnalité qualifiée de l'Arcom était l'autorité compétente au sens de l'article 4 du règlement pour examiner, soit d'office, soit à la demande des fournisseurs de services, les injonctions issus d'autorités étrangères, avec possibilité de les confirmer aussi opposés, or le sénateur Richard a très judicieusement conseillère considéré qu'il fallait prévoir un mécanisme semblable en droit national lorsque l'injonction émanait de l'Autorité nationale et s'adressait un fournisseur installé en France simplement votre commission des lois a inscrit cette précision dans un grand de bis de l'article 6 1 4 E dont nous discuterons tout à l'heure alors que cet article ne traite que de questions contentieuses, il nous semble donc plus simple et plus lisible d'inscrire à cet article 6 à hein que cette personnalité qualifiée de l'Arcom reçoivent d'une part, copie des injonctions de l'Office et mise en application de l'article 3 du règlement et, d'autre part qu'elle constitue l'autorité compétente mentionnés à l'article 4 du règlement, ce que la rédaction de la PPL prévoyait depuis le début, c'est le sens de la rédaction qui vous est soumis au grand de de l'Arctique six hein, si vous le adoptiez, je vous proposerai dans quelques instants, de procéder à la correction symétrique à l'article 6 1 4 pour ne conserver dans ce second article que la partie de l'amendement du sénateur Richert qui entend ouvrir à la personnalité qualifiée de l'art, comme la possibilité de déférer à la juridiction administrative une injonction de retrait émanant de l'Office. C'est un avis défavorable de la commission, en réalité, c'est un problème d'organisation de l'article et de logistique, la difficulté c'est que si sur le principe de cet amendement, il y a pas de désaccord de fond majeur, il est lié à l'amendement numéro 3 que l'on verra tout à l'heure et abondamment sur lequel nous avons un avis très défavorable puisque cet amendement supprime la procédure de recours devant le Conseil d'État que n'aura que la commission a établi donc c'est un avis défavorable sur l'amendement numéro un. je mets aux voix l'amendement s'il n'y a pas de d'autres demandes de parole. Qui est donc favorable à l'amendement. Qui y est opposé. L'amendement n'est donc pas adoptée, nous passons à l'amendement numéro 2 que la ministre présente. L'amendement numéro 2 modifie l'article 6 1 3 de la proposition de loi cet article donne à l'art comme un pouvoir de mise en demeure des fournisseurs de respecter les obligations prévues par le règlement TCO le grand de de l'article et le pouvoir de les sanctionner lorsqu'il ne défère pas assez mises en demeure, grand trois de cet article, toutefois, le 1er supprime dans le grand de de l'Arctique 6 1 3 qui liste les obligations pour lesquels l'Arcom peut mettre en demeure les fournisseurs de les respecter, celle qui a trait aux mesures spécifiques, en effet, le règlement prévoit déjà que l'art comme peut enjoindre l'hébergeur exposés à des contenus à caractère terroriste à mettre en oeuvre des mesures spécifiques supplémentaires lorsqu'elle considère que les mesures qui lui a présenté, afin de protéger ces services contre la défini la diffusion de contenus terroristes ne sont pas suffisantes, c'est ce que prévoit le paragraphe 6 de l'article 5 du règlement TCO en effet la jonction prévue par le règlement constitue une mise en demeure dans la méconnaissance peut faire l'objet de sanctions, il serait donc cohérent de maintenir parmi ces mesures spécifiques, la référence au 6 de l'article 5 du règlement relative à la mise en demeure, dans ce grand de de l'article, si c'est un 3 de la loi, car cela aboutirait à contraindre l'Arcom à devoir mettre le fournisseur en demeure de respecter une mise en demeure, avant de pouvoir éventuellement la le sanctionner, je pense que vous seriez d'accord avec moi qu'une telle mécanique de double mise en demeure ne serait ni pertinente ni efficace et certainement pas cohérente avec le but recherché par le règlement TCO, c'est pourquoi je vous propose de supprimer cette référence au grand de de l'article, mais de le remettre au grand trois c'est le sens du deuxième du présent amendement afin qu'il soit clair que la méconnaissance de l'injonction à prendre des mesures spécifiques supplémentaires peut donner lieu à l'enclenchement de poursuites. L'avis de la commission, monsieur le président. Alors je voudrais lever un suspense insoutenable, nous sommes favorables à cet amendement car il faut effectivement éviter cette double possibilité d'injonction merci.

du DSA, donc il sera adopté et qui rentrera en vigueur avant la fin de l'année, change radicalement toute la procédure et renverse la charge de la preuve, c'est-à-dire que ce sera bientôt au fournisseur d'accès d'envoyer aux autorités régulatrices l'art comme en France, toute une série de de pièces qui lui permettront de justifier le retrait des contenus et c'est pour cette raison là d'ailleurs que le délai d'une heure ne tient plus, c'est que le le fournisseur a l'obligation de de présenter l'identité de l'individu, son l'adresse électronique son courrier électronique et une déclaration de l'individu ou l'entité soumettant la notification de de bonne foi et on est en train de discuter sur un système donc là, dans la logique même sera complètement obsolète avant de la la fin de l'année pour un nouveau dispositif que je trouve beaucoup plus intéressant, qui est de renverser la charge de la preuve et de mettre systématiquement à la charge de l'hébergeur, tous les moyens de de

Madame la Ministre. donc je ne vois pas l'intérêt de de vous répondre sur les questions que vous posez, puisque, apparemment, les choses sont assez claires, à mon sens. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 2 du gouvernement qui a reçu l'avis favorable de la commission, quels sont ceux qui y sont favorables, celles et ceux, pardon. Quels sont ceux qui sont opposés. Et donc adopté et nous passons à l'amendement L'amendement trois a trait à la procédure contentieuse applicable aux décisions de retrait ou essentiellement rédactionnel et il vise d'une part à fusionner au sein d'un alinéa unique les dispositions identiques identiques relative au recours ouvert aux fournisseurs de services d'hébergement aux fournisseurs de contenus et à la personnalité qualifiée à l'encontre des injonctions de retrait, deuxièmement à uniformiser l'office du juge, en supprimant les termes reformation aux alinéas 34 et 38 en faveur des termes annulation qui nous semble plus explicite, troisièmement à supprimer la procédure d'appel devant le Conseil d'État pour les décisions rendues, où on a, en application des grandes et grand trois pour rétablir une voie d'appel de droit commun devant les cours administratives d'appel s'agissant d'appels interjetés à l'encontre de décisions de fond encadrant toutefois le délai en encadrant pardon toutefois le délais de jugement à un mois à compter de la date de la saisine de la juridiction, quatrièmement, supprimer la mention de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort s'agissant des décisions de l'art, comme cette règle de compétence étant de nature réglementaire. L'avis de la commission, monsieur le président, la commission émet un avis défavorable car elle supprime la procédure à bref délai que nous instaurons devant le Conseil d'État, ce n'est pas une lubie de la commission, c'est le souci d'une efficacité supplémentaire, c'est-à-dire qu'en la circonstance et sur ce type de matière, il faut aller très vite et purger le plus vite possible toutes les capacités de recours ou les ou les éléments qui doivent être tranchées, évidemment, pour savoir si on maintient la communiquer, on maintient donc à partir de là, si on rentre dans une procédure devant la cour d'appel assez classique, ça va durer, ça a duré trop longtemps, donc on s'adapte en fait aux circonstances de la cause et c'est la raison pour laquelle ne se la commission est très attaché à son recours à bref délai devant le Conseil d'État afin de purger j'allais presque dire : tous les éléments de cette procédure, merci donc défavorable. Madame la Ministre. 321 1 du code de justice administrative selon laquelle je cite les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'État, en effet, même si j'entends que ces injonctions de retraits de contenus sur Internet peuvent porter atteinte à la liberté de communication, cela ne me paraît pas devoir conduire à déroger à cette règle de compétences, sauf à considérer que que telle devait être le cas de toutes les contentieux des mesures de police administrative qui, dans leur majorité, car c'est leur objet porte atteinte à une liberté fondamentale, or le contentieux d'appel de ces décisions relèvent invariablement des cours administratives d'appel, y compris pour des décisions tout aussi graves en termes d'atteinte à une liberté fondamentale sans que le droit au recours effectif soit pour autant méconnu, il en est ainsi des interdictions de manifestations de réunion des expulsions d'étrangers ou encore des décisions restreignant la liberté de circulation, le Conseil d'État est en principe un juge de cassation et les dérogations exceptionnelles doivent le rester, sauf à remettre en cause la cohérence de l'organisation au sein de l'ordre administratif. on va pas rentrer dans la discussion trop technique maintenant, mais le recours devant la cour administrative d'appel le délai que vous reposer, vous avez d'un mois, donc c'est vrai qu'il est plus court que le délai habituel sauf que la décision de la cour administrative d'appel peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, donc on repart encore dans les délais, donc l'idée c'est de compresser au maximum quand tout de la matière, mais l'avis est défavorable, j'imagine que la réflexion de la CMP nous aidera peut-être à progresser, merci. Je peux donc mettre voir l'amendement numéro 3 présenté par le gouvernement et ce faisant l'objet d'un avis défavorable de la commission, quels sont ceux qui y sont favorables. quels sont ceux qui sont opposés, il y en a un petit peu plus et donc il n'est pas adopté. L'amendement numéro 4 du gouvernement, Madame la Ministre. L'amendement numéro 4 a pour objet de compléter le dernier alinéa de cet article unique afin de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles Wallis et Futuna sur mention expresse d'application, les dispositions de ce règlement afin de donner plein effet à l'application de ce règlement dans les pays et territoires d'outre-mer où le règlement de 2021 784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 21 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère ruisseau en ligne n'est pas applicable en vertu de du du droit de l'Union, il convient donc de prévoir explicitement une telle application. La ville de la Commission, monsieur l'amendement utile : avis favorable de la commission. Favorable. S'il n'y S'il n'y a pas d'observation, je propose de voter sur cet amendement du gouvernement, objet d'un accord d'un avis favorable de la commission, quelles sont les collègues qui sont pour. Voilà, il y en a-t-il contre. Point et donc cet amendement est adopté et il nous n'avons plus qu'à voter sur l'article unique. Composants constituant l'ensemble de la proposition de loi et ce vote sur l'article vaudra vote sur l'ensemble de la proposition. Y a-t-il des demandes d'explications de vote Madame Mercier monsieur Sido monsieur Julia. Merci monsieur le président, madame la présidente, monsieur le le rapporteur dame la ministre, mes chers collègues, bien évidemment, notre groupe va voter ce texte, mais si je puis dire, Madame la Ministre, vous savez comme moi qu'il est contre nature que des enfants soient exposés à des images qui sont violentes, pour eux, la loi du 20 juillet 2020, a été voté avec l'avis favorable du gouvernement, donc j'aimerais vraiment connaître la position du gouvernement. Ensuite, monsieur sinon. Oui, c'est l'ancien rapporteur de la loi sur la confiance dans les cuisines, l'économie numérique qui prend la parole, c'était dans les années 2 au début des années 2000, ça fait un certain temps et les choses ont bien évolué, ce que je voulais dire que ces ces textes sont très compliqué et, finalement, ça aurait dû être ça a été dit, un projet de loi, alors on a trouvé un député pour que ce soit une PPL, ça ne passe pas devant le Conseil d'État, mais en plus les quatre amendements qui ont été le présenter discuter proviennent du gouvernement, donc le gouvernement, une deuxième fois, corrige son texte sans passer devant le Conseil d'État, moi je trouve que ce genre de ce ce genre de méthode il faut l'abandonner c'est fini c'est plus de c'est pas la vraie législation le rapporteur et président de la commission l'a dit, cela a été fait en urgence et puis voilà que le rapporteur est empêcher et par conséquent c'est vraiment traiter la question des

je ne comprends pas votre argumentaire, madame la ministre, et permettez-moi d'y d'y revenir, à la fin, vous nous dites que la présente loi n'est que la transposition d'un règlement qui serait conforme aux de règlements qui vont venir dès sa DNA or juste avant vous, la ministre des Affaires européennes, enfin de l'Europe et des Affaires étrangères nous dit très justement que les de règlements des ça a des nerfs sont des pas de géant change radicalement radicalement la réglementation qui touche le numérique, comment on peut penser maintenant que le règlement sur le commerce de 2000, dont vous nous dites que cette la loi que nous votons et placé comme une transposition, comment on peut considérer que ce règlement sera encore compatible avec les deux de règlement des ça DNA, c'est absolument pas possible, donc ce que je crains, cercle, chers collègues, c'est que le gouvernement ne soit obligé de revenir vers nous, avant la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine pour que alors j'espère cette fois-ci que ça sera un projet de loi est pas une proposition, mais que nous puissions adapté une nouvelle fois le droit français aux changements radicaux qui vont être apportés par les 2 règlements des ça et DNA je leur nous nouveau trop contre parce que moi j'ai j'ai une passion absolue pour la mythologie grecque et j'adore Pénélope mais faire et défaire ce ça ça ça ça fait perdre souvent du merci monsieur le président. d'une proposition de loi, il n'y a pas de saisine du Conseil d'État, ni d'étude d'impact, on peut, on peut le regretter, mais c'est le modèle qui est déposé aujourd'hui, messieurs les sénateurs et donc cette PPL, elle vise à adapter notre droit à un règlement européen qui s'impose à nous et donc l'étude d'impact n'a pas lieu d'être, mais vous le savez aussi bien que moi, je crois, si nébuleux.

263825 signalements en 2021, dont plus de 7800 liés au terrorisme, le doublement des effectifs entre décembre 2000 20 juillet 2021 passant de 24 à 52 dont 14 gendarmes a permis de faire évoluer le fonctionnement et l'organisation de la plateforme, il me semble que c'est des chiffres que vous aviez réclamé la prise en compte, je citerai aussi la prise en compte des signalements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la création d'une cellule spécialisée dans le traitement des contenus discriminatoires, la cellule spécialisée dans le traitement des demandes administratives visant les contenus pédo-pornographique pédo-pornographique et terroriste chargé et c'est là Madame Mercier, je réponds à votre question, chargé des actions de détection proactive des contenus illicites enfin une brigade judiciaire chargé d'accentuer la judiciarisation des contenus illicites voilà ce que je voulais vous dire mesdames et messieurs les sénateurs, en conclusion de cette séance cet après-midi. je vais donc mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne sur l'ensemble sur l'article unique donc, quels sont ceux qui sont favorables. Voilà. Y a-t-il des voix contre. Et les abstentions. l'article unique et la proposition de loi sont donc adopté, chers collègues, je vais lever la séance, la prochaine séance, c'est demain mercredi, mercredi 13 juillet à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement, la séance est levée.